Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 17 mai a été publié sur le site internet du Sénat, il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé le procès verbal est d'autres. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons appris avec beaucoup d'émotion. Le terrible accident qui a eu lieu dimanche matin dans le nord près de Villeneuve un chocs entre véhicules a entraîné la mort d'une policière et de de policiers en mission dans le cadre de leurs fonctions au commissariat de Roubaix ils étaient âgés de 24 et 25 ans. C'est avec la même émotion que nous avons appris la violente agression au couteau. Lundi 22 mai au CHU de Reims d'une secrétaire médicale, grièvement blessée et d'une infirmière malheureusement décédé cette nuit. Au nom du Sénat tout entier. Je souhaite leur rendre hommage et présenter à leur famille nos condoléances les plus attristées. Je vous propose d'observer un instant de recueillement.

Je vous remercie. J'ai le regret également de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Madelin qui fut sénateur d'Ille-et-Vilaine. De 1980 à 1998. L'ordre du jour appelle à présent, les explications de vote, des groupes et le vote par scrutin public solennel sur la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France présenté par messieurs Laurent Duplomb Pierre Louvot Serge Méry You et plusieurs de leurs collègues. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que ce scrutin s'effectuera depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc chers collègues à vous assurer que vous disposez dès à présent de votre carte de vote et vérifier que celle-ci fonctionnent correctement. En l'insérant dans votre terminal de vote. Vous pourrez vous rapprocher des initiés si vous avez des difficultés ou si vous avez perdu la dite carte. Avant de passer au vote. Je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote. Un peu de silence, pour que nous puissions entamer l'explication de vote. 7 minutes pour chaque groupe, 3 minutes pour les non inscrits. La parole est à présent à monsieur Laurent Duplomb des républicains pour sept minutes, chers collègues. Madame la présidente. Madame la présidente de la Commission. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il va de soins que sur ces bancs. Nous ne proposons pas tous les mêmes solutions et que nous n'avons pas tous la même vision de l'agriculture française. Les débats de la semaine dernière l'ont du reste montré. Sur plusieurs articles les positions. Était clairement antagonistes avec des, des propositions de suppression d'articles. Mais je crois en la liberté d'opinion et dans la vertu et dans les vertus de la confrontation des idées, je crois qu'il est bon et sain que ces divergences et plus s'exprimer. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous a manqué. Sur les 6 dernières années avec la prétention d'un pouvoir omniscient à dépasser tout clivage. Je veux donc ici. Saluer la courtoisie républicaine dans laquelle ces débats se sont tenus. Malgré ces désaccords marqués et en dépit d'une offensive médiatique injuste qui a qualifié ce texte je cite de de profonde régression consumériste et environnementale de cheval de Troie de l'auto de l'agro-industrie ou encore de lettres au Père Noël de la FNSEA. À rebours de ses caricatures. Je crois que nous avons su montrer l'exemple. Le monde agricole et la la ruralité nous serons reconnaissants d'avoir discuté jusqu'à tard dans la nuit de leurs problèmes de charges de normes et des impasses techniques auxquelles ils font face avec des arguments et des chiffres sérieux tiré de la réalité et de leur quotidien. À défaut d'un vote humaniste unanime sur les propositions. Il est dommage que nous ne nous entendions pas sur le diagnostic vécue au quotidien par les agriculteurs. Si les constats de la désindustrialisation de la France ou de sa dépendance énergétique sont aujourd'hui bien admis, je regrette qu'une forme de déni et empêcher certains d'y voir aussi clair pour notre agriculture sur ces bancs ou ailleurs certains pêche encore par une naïveté trop coupable et certains sont peut être frappée de cécité idéologique. Risque de black-out cet hiver. Rupture d'approvisionnement en composants industriels critique et même en paracétamol. Nous connaissons le même glissement aujourd'hui dans le domaine agricole. L'histoire pourrait ressembler, comme l'a écrit Géraldine Hausner un conte pour enfant dans lequel les habitants d'un pays comblé par la nature croulant sous c'est bien fait en seraient curieusement. À se persuader que les richesses les entourant était le fruit, non pas 2 siècles de la bord des générations précédentes du climat ou de la géographie. Mais de leur propre vertu et qui à force de s'aveugler sur eux-mêmes en viendrait à détruire leur trésor. La recommandation d'hier de la Cour des comptes, de réduire le cheptel de vaches françaises et la preuve de cet aveuglement. Et cette technocratie abrutissante sera capable après cette injonction contradictoire de s'étonner de la hausse croissante du déficit de la balance commerciale sans faire le lien Direct avec notre excédent positif des produits laitiers. Le message de la Cour des comptes me rappelle cette phrase de Tocqueville cet état se veut si bienveillant envers ses concitoyens qu'il entend se substituer à eux dans l'organisation de leur propre vie. Ira-t-il jusqu'à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d'eux-mêmes le plus grand soin d'un bon gouvernement, Monsieur le Ministre, devrait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. Est-ce vraiment à la Cour des comptes de s'occuper de savoir ce que les Français doivent manger alors qu'elle est incapable. Alors qu'elle est incapable depuis des années d'inverser la spirale de la dette du déficit public et de l'appauvrissement progressif de la France. Le diagnostic du déclassement de la France de la ferme France existe depuis au moins quatre ans et le rapport que j'ai présenté en 2009 le rapport présenté en 2022 avec Pierre et Serge Mir mais Riou n'est que la démonstration à une échelle plus fine avec cinq produit emblématique de l'érosion continue de nos parts de marché notamment au sein de l'Union européenne et de la baisse tendancielle de nos taux À ce stade, je voudrais saluer le courage de Serge Merriot qui a su et compris à travers les auditions et les visites à la, à quel point notre agriculture était mal en point et qui n'a rien cédé à l'intimidation de l'écologisme dogmatique. Par son courage il a démontré que nous sommes pas à la solde de quiconque. Comme l'écrit le président du FC que choisir qui d'ailleurs ferait mieux de rester dans le cadre de ses prérogatives en s'occupant du pouvoir d'achat des Français et tout particulièrement de celui des 16% de Français qui aujourd'hui à cause de l'inflation et du tout monter en gamme déclare ne plus manger à leur faim. Oui, cette proposition de loi et le remède que nous voulons appliquer, je ne me réjouis de son caractère jusqu'au bout transpartisan. Venant en À la suite. Car si l'adoption aujourd'hui de ce texte est en soi une très bonne nouvelle pour le monde agricole, il serait bien dommage de s'arrêter en si bon chemin. Peut-on considérer que la proposition de loi adoptée en première lecture au Sénat. Notre s'est achevée où notre tâche accomplie. Non. Certains journalistes ont vu dans cette dans ce texte la simple tentative de la part de la droite sénatoriale de déplacer le débat de décaler le Champ de ce qui est acceptable ou ne l'est pas du du dicible et de l'indicible. Je réponds très clairement à ceux-ci. Ce n'est pas la fenêtre d'Overton que nous avons ouverte mais les yeux devant la réalité. Comme je l'ai rappelé la semaine dernière. Il ne faut pas avoir peur et vous n'avez pas eu peur par vos votes la semaine dernière vous avez prouvé dans votre grande majorité que vous non plus vous n'avez pas peur. J'appelle les parlementaires de tous bords et notamment de l'Assemblée nationale à faire de même, ainsi que le ministre de l'agriculture dont le soutien n'a pas été à toutes les épreuves, la semaine dernière, hormis peut-être sur le Livret A ou les peint ou l'épandage par drônes car il va. Car il va falloir trouver une traduction concrète aux propositions que dans sa grande majorité, et dans son non moins grande sagesse, le Sénat s'apprête à adopter. Inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Hein. Injection dans une loi d'orientation et d'avenir attendu pour l'Automne, l'avenir nous le dira. Mais soyez sûrs. Je ne lâcherai rien et nous ne lâcherons rien pour que ce texte poursuive son chemin, celui de l'espoir, celui de la fierté retrouvée votants pour que notre agriculture reste fier pour que l'agriculture française. Villiers et continue de vivre.

En attendant la venue de Monsieur Pierre Med via du groupe les indépendants. Je voudrais saluer la délégation il y a EDF de Nouvelle Aquitaine, une délégation importante qui est venu à notre rencontre maire. Monsieur Manuel, vous avez 7 minutes. Madame la présidente, madame la présidente de commission. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis 2019, la France ne produit plus qu'elle consomme. Cette situation inédite totalement indigne de notre potentiel de production agricole ne peut que nous questionner. Comment en est-on arrivé à une telle opération. Au pays de Sully, est-il normal de voir nos agriculteurs. Stigmatiser. Continuellement. Est-il normal de subir l'intégrisme écologique qui nous empêchent de profiter des dernières innovations agro-technologique. Est-il normal de livrer en pâture aux agriculteurs, aux agité du bocal incompétente des réseaux sociaux qui dans un délire utopiste nous éloignent des réalités économiques et terrienne de cette noble profession. Est-il normal de décider des sur-transpositions de directives qui ne font que pénaliser nos réacteur français face à la concurrence européenne. Est-il normal enfin de devoir toujours, bataillé pour faire admettre des mesures évidentes de bon sens. Face à la guerre en Ukraine qui a bouleversé les marchés agricoles mondiaux. Face au réchauffement climatique et à la diminution des surfaces cultivables dans le monde. Et face aux prévisions démographiques actuelles notre agriculture doit absolument prendre un nouveau virage. Après la révolution d'après-guerre avec remembrement et mécanisation nous allons devoir relever un nouveau défi. Produire plus et mieux, alors que le stress hydrique sécheresse et catastrophes naturelles ne font que s'accentuer. Trop souvent la presse et les médias n'écoute que les détracteurs notre modèle agricole et ne relaie que les commentaires des marchands de peur et de sensationnel. Il est facile de s'émouvoir des contrats signés avec les autres continents, comme le CETA ou dans le cadre du Mercosur sans en connaître le contenu exact. Le danger, comme l'a souligné, Monsieur le Ministre ne vient pas toujours des autres continents. Si je prends l'exemple des production bovine ou maraîchères. Nos principaux concurrents sont aux portes dans notre pays. L'Europe doit se doter à court terme d'un cadre législatif harmoniser. Si nous voulons peser de tout notre poids sur les marchés mondiaux, préalable indispensable à la survie de notre production agricole nationale et européenne. J'en viens maintenant plus précisément. Compte tenu de cette proposition de loi. Dans le titre au premier, il paraît évident que la recherche de compétitivité de la ferme France et des investissements que nous devons lui consacrer chante une priorité absolue. Un des premiers amendements d'ailleurs que nous avons soutenu consacrent la souveraineté alimentaire comme l'intérêt fondamental. De la nation. De même, nous pouvons que nous féliciter de la constitution de fonds spécial de soutien à la compétitivité des secteurs agricoles en difficulté. L'investissement, la modernisation le produire local et la réorganisation des filières doivent nous permettre de relancer la productivité de la ferme France. Notre agriculture pourra ainsi retrouver la place qui était la sienne dans notre balance commerciale extérieure. Je tiens d'ailleurs tout particulièrement à saluer certaines mesures inscrites dans le titre de notamment la création du livret Grimm et la mise en place de crédit d'impôt pour les investissements en agriculture qui permettront de réduire les coûts de production et de faire progresser la compétitivité prix seule possibilité de réussir la modernisation indispensable de nos exploitations. Nous ne pouvons plus nous en tenir aux discours rétrograde de certaines organisations comme la Confédération paysanne ou les adeptes de l'agriculture de grand-papa. Ces sondes de trembler devant des exploitations de dimension plus importante car seule la rentabilité de ces structures permettra l'attractivité et l'attrait de la profession. Trop d'agriculteurs sont isolés peu soutenu et renonce hélas dans de nombreux cas à projet d'installation et d'évolution. Par ailleurs, je tiens à évoquer la dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Elle était encore un bel exemple des effets délétères du refus du progrès et du modernisme. Ce système permet pourtant dépendra moins de produits et représente une sécurité indispensable notamment dans les zones collinaires. Les instituts comme line raillé ou encore les écoles d'agriculture et d'agronomie ne cesse de nous montrer tout le bénéfice des évolutions scientifiques et technologiques. Des progrès qui semble être ignorée par beaucoup, par exemple la surveillance satellitaire des cultures permet dépendent beaucoup moins de produits phytopharmaceutiques. En ne traitant que les gens ne fait c'était. Au cours de nos débats. Nous sommes particulièrement revenu sur le cas de Lanxess et son rôle. Cette agence donc j'ai envié par bien des pays, il a eu, dans cet hémicycle de vives discussions sur ses prérogatives et ses missions. Pour rappel, cet agent d'expertise scientifique. Évalue tous les risques sanitaires alimentaires et environnementaux. Elle est allongée ne du concept révolutionnaire à l'époque de phyto-pharmacovigilance. En tant que rapporteur pour avis de l'examen du projet de loi Egalim hein. J'avais loué le caractère indispensable cette agence et demander à ce qu'aucune interdiction en matière de produits phytos ne se fasse sans l'avis de la MCS. En cas de litige qui liait discussion avec le ministre sur le rapport bénéfice risque me paraît judicieux. Mais je suis beaucoup plus partagés sur le Rwanda, véto. De même, il serait nécessaire d'augmenter les crédits alloués à la duchesse. Afin de débloquer plusieurs dossiers d'autorisation de mise sur le marché de nouvelles Start-Up qui présentent des molécules pourtant très novatrices, notamment dans le domaine des biocontrôle. Nous replongeant dans l'éternel débat des produits phytopharmaceutiques. Il a eu de grosses erreurs commises dans le passé. Mais nous progressons constitutionnellement en terme de qualité et d'objectivité des expertises. S'imaginer aujourd'hui comme certains que l'on peut vider complètement la trousse à pharmacie relève de l'idéologie pure et du fantasme. Il y aura toujours des attaques bactériennes, fongiques ou d'insectes sur nos cultures. Et quand on voit la taille actuelle des parcelles ainsi que leur proximité. On imagine aisément les conséquences des attaques sans réaction cibler notre part nous avons hélas vécu un bel exemple avec les attaques dans le Sud-Ouest et le reste du pays, de la pyrale du buis. Pour conclure, mes chers collègues. Cessons de polémiquer autour de blocage est purement idéologique dans la profession a trop souffert ces dernières décennies. Ce texte contient plusieurs mesures de bon sens nécessaire à la modernisation de notre agriculture. Nous ont rapidement d'autres débats sur des sujets primordiaux comme celui de l'eau. Le Sénat en tant que fin connaisseur des territoires et des sujets agricoles devra jouer à plein son rôle de créateur de solutions seul intérêt de l'agriculture française, donc il y a une notre action pour ces raisons le groupe les indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. Merci cher collègue. La parole est à présent. Aux sénateurs, Joël Labbé, du groupe des écologistes cherchent. Vous avez 7 minutes.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure. J'ai entendu mais de les deux premiers orateurs. Je vois que nos avis sont divergents particulièrement divergent. Choc de régression. Cheval de Troie de l'agro-industrie. Proposition de loi d'un autre temps, ces mots sont sont ceux des associations paysannes environnementales de consommateurs pour décrire les reculs inacceptables portées par ce texte qui a choqué à juste titre l'ensemble des acteurs qui travaille depuis des années à construire un modèle agricole et alimentaire plus durable et plus équitable. En effet les reculs portées par ce texte sont nombreux. Et nous continuons de les dénoncer. Je citerai la remise en cause de Lanxess et la proposition de mise en balance. du niveau de, de santé et d'environnement avec celui des enjeux économiques pour le retrait des pesticides, nous paraissent particulièrement graves. L'autorisation des pantalons de pesticides par drone malgré les risques sanitaires pointées par l'ne c'est également un recul majeur. Le recul sur la séparation entre la vente et le Conseil sur les pesticides envoie un très mauvais signal sur la nécessité de développer un conseil indépendant auprès des agriculteurs pour la réduction parce que c'est le but et la sortie de l'usage de ces produits. De même, plutôt que de faire appel au volontarisme des acteurs pour appliquer la loi Egalim, restauration collective, l'article 11 acte là aussi un retour en arrière en repoussant l'échéance et en abaissant l'exigence de qualité. Sur l'eau. Madame la rapporteur le texte de façon très inquiétante priorisent le stockage pour les pour l'irrigation en le considérant d'intérêt général majeur sans réflexion sur le partage de cette ressource. Il propose aussi de soutenir massivement et sans conditionnalité l'investissement agricole enfin dans un contexte de tension sociale ce texte propose dans une proposition de loi agricole de réformer, Pôle Emploi et le cumul RSA revenu d'activité au détriment des droits sociaux. Les solutions proposées ne répondent pas aux questions cruciales du revenu des agriculteurs et de la hausse des importations de produits alimentaires se lancer dans la course au moins disant. Ne permettra pas de construire notre souveraineté alimentaire. Cela accélère notre dépendance à des intrants issu d'importation et dont les coûts explosent et affaibli les écosystèmes. Alors que les agriculteurs dépendent des sols des pollinisateurs du cycle de l'eau du climat. Les solutions se situent dans la régulation des marchés, la sortie des accords de libre-échange. Et dans une répartition équitable de la valeur. Elle réside aussi dans un rééquilibrage des aides PAC inégalement distribuées au détriment des filières pour lesquelles les importations augmentent. Il s'agit également de mener avec volontarisme politique de relocalisation de l'alimentation. Pour cela il nous faut construire un accès de tous, toutes et tous à une alimentation de qualité. On ne peut que déplorer l'abandon du chèque alimentaire durable et qui devait être un 1er pas vers un droit à la, à une alimentation de qualité et locales droit pour tous bénéfique pour les agriculteurs et pour nos concitoyens. En cette période d'explosion de la précarité. Nous continuerons de défendre une sécurité sociale de l'alimentation afin de conjuguer droit à une alimentation durable et rémunération équitable des agriculteurs. Car le modèle agro-écologique basée sur des pratiques agronomiques permettant de se passer d'un conjugué avec des politiques alimentaires forte permettront, nous en sommes convaincus de réussir le défi de la transition. Mais pour cela il faut un accompagnement fort des alternatives alors que seul 1% de la dépense publique agricole contribue à la sortie des pesticides. Il faut aussi soutenir l'agriculture biologique pour laquelle ce projet de loi n'a pas une seule ligne. La transition se doit pourtant d'être accompagné et organisé le directeur de l'INRAE affirmait en audition au Sénat l'importance de l'anticipation, plutôt que d'attendre l'arrivée de contrat extérieur. Il a insisté aussi sur la stabilité et la cohérence des politiques publiques. Pour les rails. Après un travail scientifique, la sortie des produits phytosanitaires à l'horizon 2050 est possible. Pour cela on a besoin de recherche et des moyens de la recherche. On a appris par le directeur de l'INRA et que le budget. De recherche de Bayer, un des piliers du funeste fit Eh bien le budget de Bayer est 4 fois supérieur à celui de l'INRAE. C'est dire si on doit faire des efforts. Avec ce texte qui fait l'impasse sur les enjeux environnementaux et sanitaires à venir et revient sur le droit existant. C'est tout le contraire qui est proposé, mais malgré tout les propositions que nous contribuons à porter bien que caricaturer dans les débats portent parfois leurs fruits. Ah si nous alertons à chaque texte budgétaire sur l'application de la loi Egalim. Les annonces récentes du gouvernement, Monsieur le Ministre semble aller dans le bon sens. Idem pour le soutien à l'agriculture biologique sur lequel en lien avec les filières nous alertons depuis des mois les financements annoncés sont nécessaires. Même s'il reste tardif est encore insuffisant. Ainsi, alors que nous assistons avec regret et dépit au vote positif de ce texte auquel nous nous opposons fermement. Nous serons vigilants et combatifs. Pour que les débats de la loi d'orientation et d'avenir agricole permettent de construire de véritables solutions pour notre agriculture. Nous voterons contre. Farouchement contre ce texte. Pour les cales minutes pour les quelques minutes. Pour les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous parler. Et du plan tout à l'heure il avait il avait tous les droits. Je voudrais vous parler des projets des des projets alimentaires territoriaux obtenu de force dans dans la loi d'avenir agricole 2014 partout où ils sont en place, ils jouent parfaitement le rôle est un voeu pieux. Serait de voir l'ensemble du territoire français. Couvert de projets alimentaires territoriaux allant. Vers la souveraine souveraineté alimentaire des territoires. Allant aussi vers une rémunération plus juste des agriculteurs. Le respect de la biodiversité, le respect du climat. Alors vous me direz, je vous entends mais là ce sont des utopies et je vous répondrez. C'est l'utopie qui nous sauvera la vie. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent. Un autre collègue sénatrice Madame, Patricia Schillinger pour sept minutes, chers collègues. La seule femme de l'après-midi. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. La semaine dernière nous avons achevé tard dans la nuit l'examen de cette proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France sur laquelle nous sommes invités à nous prononcer. Du rapport de l'Automne dernier a aujourd'hui le chemin parcouru est positif et aujourd'hui nous nous accordons sur la nécessité de ne pas céder à l'opposition stérile entre les différents modèles à la condamnation en bloc de la stratégie de montée en gamme ou à la caricature d'une agriculture dite productivité. Productivité, ce dont nous sommes loin de la France. Le défi que doit se. Lever notre modèle agricole n'est pas anodin, il s'agit de restaurer la puissance agricole de la France que plusieurs décennies de déclin ont abîmé. Alors que la planète entière subit d'ores et déjà les conséquences du dérèglement climatique, l'adaptation de ce dernier. Et aux évolutions de la disponibilité de la ressource en eau, le renouvellement des générations et la préservation de notre souveraineté alimentaire sont 3 priorités qui se rejoignent et sont chacune vital pour notre agriculture. La loi d'orientation agricole dont les concertations se déroulent encore sera une nouvelle occasion d'aborder ces sujets sur lesquels il nous faudra trouver un consensus. De nombreux producteurs français ont fait le choix du bio ou d'une activité sous le signe de qualité synonyme de valeur ajoutée de prix plus rémunérateurs et de conquête de nouveaux marchés. Les jeunes agriculteurs installés ou en devenir ont souvent la volonté de participer au changement de paradigme que nous connaissons, nous devons les accompagner car leur réussite sera notre réussite. C'est le sens de l'annonce du ministre-la semaine dernière du renforcement du plan de soutien à l'agriculture biologique avec la mobilisation de 60 millions pour résoudre les difficultés urgente une nouvelle campagne de communication et surtout l'engagement de l'État de respecter d'ici la fin de l'année, l'objectif de 50% des produits sous signe de qualité et durable et de 20% minimum de produits biologiques en restauration collective, dans chaque établissement relevant de lui. Sur ce dernier point, nous saluons la volonté d'exemplarité de l'État. Pour autant, il n'est pas question de neutre de ne traiter et de n'. Que l'agriculture biologique. tous les agriculteurs ont leur métier à coeur et la volonté de nourrir du mieux qu'ils peuvent les Français c'est pour les soutenir que nous souhaitons les accompagner dans leur adaptation et leur anticipation des conséquences du dérèglement climatique. Notre objectif est clair, poser des Paz durable à la puissance agricole et à la souveraineté alimentaire de la France du XXIe siècle. C'est le sens de notre engagement depuis 6 ans aux côtés du gouvernement et de notre action pour que les transitions nécessaires s'engage rapidement de manière pragmatique et efficace sur le fond du texte. Nous sommes convaincus que certains articles pourront être intégrées dans la loi d'orientation d'avenir agricole. L'article 9 qui permet une meilleure reconnaissance des externalités positives de l'agriculture en matière de stockage du carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'article 16 qui renforce les péter GE et il y a introduit des concertations concourant ainsi à la nécessité de créer du consensus sur la gestion de l'eau. Par ailleurs, je me réjouis de la rédaction finale de l'article 8 concernant l'épandage des produits phytopharmaceutiques par drone. En effet, je rappelle que le dispositif que nous a proposé Madame la rapporteure et très bien cadré, seuls les surfaces agricoles, avec une pente supérieure ou égale à 30% et l'agriculture de précision peuvent bénéficier de l'expérimentation. Une évaluation de l'c'est c'est toujours prévu et peut déboucher sur la possibilité d'ouvrir une dérogation pour 5 ans offrant potentiellement une décennie à la filière pour exploiter son potentiel en matière d'exploiter de réduction d'usage et de produits phytosanitaires coffre cette technologie. Nous avons trouvé un équilibre qui permet de préserver l'innovation au service de la transition et de la compétitivité de notre agriculture. Cependant il suce 10 des points de blocage. L'article 15, par exemple, nous considérons comme primordial d'adapter. Et nos modes de production et l'aménagement de nos territoires aux conséquences dures dérèglement climatique sur la disponibilité de l'eau des ouvrages de stockage de l'eau auront une importance majeure pour remplir ces 2 objectifs, tout comme la réutilisation d'eaux non conventionnelles et l'adaptation du système des productions mais chaque projet différent et c'est à chaque territoire de s'organiser ainsi la déclaration d'intérêt général majeur prévu à l'article 15 nous nous apparaît disproportionnée et fermant la porte à la concertation locale sur un autre plan, nous pourrions également évoqué les mesures liées au travail et à la fiscalité qui bien que nous apparaissent intéressante et pour certaines d'entre elles pertinentes. Relève de la loi de finances ou de la loi de travail je pense particulièrement à la pérennisation du TO-DE à laquelle nous sommes attachés pour offrir aux agriculteurs une meilleure visibilité sur une sur un dispositif qui fonctionne, mes chers collègues. Si cette proposition de loi pose des débats que nous retrouvons dans la loi d'orientation et d'avenir agricole ainsi que dans les projets de loi travail et les projets de loi finances elle pose également des questions qui renvoient à notre rapport à l'agriculture et à la nature la compétitivité de l'agriculture n'est pas un gros mot, la préservation de l'environnement non plus la souveraineté alimentaire de demain nécessitera que nous ayons pris aujourd'hui des décisions qui préserveront les qualité de nos sols de nos savoir-faire et de nos produits. Le groupe RDPI adopte sur ce texte, une position de liberté individuelle de vote. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent à monsieur Jean-Claude Tissot du groupe socialiste. Comme pour sept minutes,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente, rapporteur. Mes chers collègues. Dès 8h de débats que nous avons consacré à cette proposition de loi auront permis de clarifier les positions et les divergences entre la droite sénatoriale et l'ensemble des groupes de gauche. Pour des enjeux aussi importante, l'agriculture et l'alimentation. Il est toutefois regrettable d'avoir dû débattre sur un temps parlementaire si court. Sans étude d'impact pour des dispositions majeures et surtout avec de nombreuses imprécisions de définition sur des thèmes centraux de ce texte. De la discussion générale nous avions parfaitement compris la stratégie de la majorité sénatoriale qui cherchant à prendre ses marques pour la future et doit a souhaité imposer un certain nombre de concepts dans le débat de notre politique agricole. À ce titre il est malheureux que la grande majorité des dispositions de ces dispositions de loi ne soient que des retours en arrière sur des législations des rapports adoptés ici même face à tout cela, Monsieur le Ministre, vous avez pris le parti dans un 1er temps de défense et propositions de loi de manière vigoureuse lors de la discussion générale avant d'adopter une approche bien plus modéré lors des débats. J'en veux pour preuve les avis favorables que vous avez exprimé de sur de nombreux amendements de suppression de mon groupe aux articles 6 7 11 13 15 17 et 22. Nous saurons nous souvenir de ses positions lors de l'examen de la LOA. Toutefois, lors des débats. Monsieur le Ministre, vous avez appelé à de nombreuses reprises à ne pas tomber dans la caricature vis-à-vis cette proposition de loi en vous tournant principalement. Vers la gauche de cet hémicycle la relecture des comptes rendus de séance prouve pourtant que les interventions caricatural ou simpliste ne se trouvait pourtant pas de ce côté-là les nombreuses interruptions lors de la présentation de la question préalable en sont de bons exemples présentés défendre une autre vision de l'agriculture ce n'est pas mes chers collègues. Une caricature mais simplement. Un avis. Pour un débat politique sur laquelle avec nos compétences et nos expériences nous apportons des approches techniques et concrètes pour nous aussi. Le mot compétitivité n'est pas un gros mot et nous l'avons clairement mise en avant en démontrant que les exploitations agro-écologiques peuvent être parfaitement compétitive et rentable, tout en préservant la santé de l'agriculteur et son environnement immédiat. Il est donc totalement anormal qu'un texte qui aborde au sens large. Notre modèle agricole décide de ne pas s'intéresser à toute une part de notre agriculture en ne citant un aucune reprise des notions d'agriculture biologique et agroécologie. Les maigres ça joue que nous avons obtenu que ce soit sur la durée dit durabilité au sein démission du commissaire à la compétitivité ou à la demande d'un rapport sur les paiements pour services environnementaux sont des premiers pas mais ils ne viennent pas contrebalancer la teneur générale du texte, une nouvelle fois nous rappelons notre opposition aux mesures fiscales proposées qui ne bénéficieront pas agriculteurs les plus en difficulté, ni à ceux qui débutent dans le métier si nous souhaitons favoriser l'installation d'un d'agriculteurs et ainsi permettre une inversion de la courbe du nombre d'exploitations réfléchissons davantage au renforcement des mesures ciblées et limitées dans le temps, comme l'a dit, j'y a plutôt carrée aussi des plafonds pour des agriculteurs qui ont déjà la chance de mettre des sommes importantes de côté. Sur la question des aides publiques. Il est dommage Monsieur le Ministre, chers collègues du plomb que nous n'ayant pas eu davantage de débats et d'échanges au Parlement sur le PSN. Plan stratégique national de la PAC qui vient d'entrer en vigueur. Sortir de la réflexion uniquement centrés sur des aides à l'hectare pourrait être un axe d'évolution intéressant pour poursuivre. Nous sommes au sein du groupe socialiste opposé avec vigueur à l'ensemble des articles qui réécrivent allègrement le droit du travail. Sans aucune caricature. Nous avons parfaitement conscience des besoins spécifiques en main d'Oeuvres d'un secteur comme l'agriculture, que ce soit sur la temporalité ou les compétences. C'est la raison pour laquelle nous avons une nouvelle fois soutenu la pérennisation des dispositif TODE et proposer son élargissement aux États arf entreprise des 3 agricoles forestier et ruraux toutefois l'ajout de la notion de secteurs prioritaires en tension dans l'émission pour l'emploi, la généralisation du cumul RSA emploi ou encore la création d'une exonération au sein du dispositif bonus Banu bonus malus sur les contrats courts nous paraissent complètement à contresens des attentes des agriculteurs et des salariés du secteur. Les agriculteurs souhaitent avoir une main oeuvre formée et disponible dans les territoires et pour cela, c'est la question de la formation agricole, qui doit être au coeur du débat et non pas une nouvelle précarisation du marché du travail ou les travailleurs seraient la variable d'ajustement d'un secteur intensif. L'absence d'opposition de la part du gouvernement sur ces articles qui s'est arrangé derrière un avis de sagesse est à ce titre particulièrement inquiétant. Espérons que le futur projet de loi travail tant annoncée ne soit pas de cette teneur à ce titre nous regrettons profondément. Monsieur le ministre. Publication en catimini le 13 mai d'un décret redéfinissant le statut d'agriculteurs actifs. C'est une porte ouverte à mon sens un autre sens à la Financière réalisation sans limite de l'agriculture à une prise en main de nos exploitations par des investisseurs extérieurs aux intérêts bien éloignée des paysans.

Permet de revenir sur ces dispositions ou tout du moins de les adoucir ce n'est malheureusement pas le cas au contraire sur l'article 8, la pérennisation de l'usage de drone en agriculture. À l'issue de l'expérimentation prévue a été adopté sur ces sujets. Monsieur le Ministre, vous avez adopté les propositions des positions différentes en soutenant l'article 8 tout en vous opposant aux articles 13 et 18 alors que le gouvernement commence à réfléchir à des solutions pour adopter la France pour adapter la France à une température de plus 4 degrés en 2100, il serait peut-être bon de tenir un discours plus cohérent sur un secteur qui représente 21% des émissions de gaz à effet de serre mais qui est aussi la première victime du changement climatique. Sur la question de l'eau, je l'avais dit en discussion générale mais nous avons mais nous considérons que traiter ce sujet de cette manière, c'est simplement mettent de l'huile sur le feu dans sa portée sans apporter de solution concrète à la problématique du stockage déclaré d'intérêt général majeur, un projet de stockage d'eau par principe et réduire parallèlement les contentieux ne font que prouver votre vision idéologique de l'eau que vous souhaitez privatisé que pour quelques-uns, il s'agit pourtant d'un bien commun que nous devrions défendre collectivement notre souveraineté alimentaire passera aussi par le partage de l'eau. Non non non non. En cohérence avec notre position pendant les débats avec mes collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain. Nous nous opposerons évidemment à cette proposition de loi, nous aussi, nous souhaitons apporter répondre nous souhaitons répondre et aider les 16% de Français qui déclare ne pas manger à leur faim mais nous ne pouvons pas nous résoudre à leur fournir des aliments de faible qualité qui ne sont que des bombes à retardement sanitaire produit par des agriculteurs étranglés par le marché, au contraire, nous prenons une restructuration de notre modèle agricole avec une véritable répartition de la valeur et un accompagnement des pouvoirs publics à la hauteur des transitions nécessaires la compétitivité de l'agriculture française passera par ceux-là. Je vous remercie. remercie. La parole est à présent. Un notre collègue monsieur le sénateur, Fabien Gay du groupe communiste. Vous avez 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier les auteurs de cette proposition de loi. Car si nous ne partageons quasiment rien pour ne pas dire aucune des propositions qui sont faites et du projet de société qui est défendu, ce texte a au moins une vertu. Celle de nous faire parler de cette France rurale. Agricole des paysannes et des paysans si souvent ignorés méprisés voire conspué et qui se sent légitimement incompris. Alors que nos paysans remplit chaque jour une mission d'intérêt général, celle de nous nourrir. Qu'ils sont en première ligne face au changement climatique et qu'ils sont les seuls ouvriers et artisans du vivant. Il ne décide pourtant pas des prix à la vente et sont obligés de survivre pour nous nourrir. Ils sont souvent voire toujours les premiers sacrifiés par les gouvernements successifs dans les traités de libre-échange alors qu'au contraire, il nous faudrait un débat sur le droit à l'alimentation de qualité pour toutes et tous, au moment où il existe déjà une alimentation à 2 vitesses, non il ne faut pas opposer agriculture conventionnelle et biologique. La première qui reste d'une grande qualité nourri la majorité de la nation et pourtant sans cesse stigmatisé oui nos paysans sont pris dans des saisons injonctions contradictoires entre produire toujours plus, toujours mieux toujours moins cher, et toujours en concurrence avec des pays qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales. C'est donc tout le logiciel qu'il faut changer car on ne soigne pas le libéralisme par l'ultra-libéralisme, au contraire, nous devons aider. Accompagner leur transition pas contre eux, mais avec eux et les aider à sortir progressivement des schémas l'agrobusiness et des produits phytosanitaires. Qui ont d'abord des effets néfastes pour eux et ensuite pour les consommateurs. À l'inverse, l'agriculture biologique ne doit plus être moqué ou raillé m'aider encourager. Pour que celle-ci peut-être puisse être accessible à toutes et tous et devienne demain la norme. Oui, il faudra s'attaquer enfin à la puissance des centrales d'achat et des agro-industriels qui font des marges pour rémunérer les agriculteurs à des prix qui dépassent leurs coûts de production et de l'autre côté de la chaîne. Augmenter les salaires des consommateurs pour qu'ils puissent acheter des produits de meilleure qualité. Ces grands enjeux, chers collègues, nous ne pensons pas les atteindre avec des recettes qui ont prouvé leur, il ne fait qu'inciter économique et social et leur nocivité écologique non continuer à appauvrir les sols avec des insecticides et pesticides n'est pas une vision de long terme et ce n'est pas l'utilisation de drônes pour aller plus vite, plus loin et plus fort dans l'épandage qui réglera quoi que ce soit. Non, rejeté la ville Lanxess n'est pas sérieux. Car si elle avait existé, il y a 40 ans, nous aurions certainement interdit le chlordécone aux Antilles bien avant non conditionner le versement du RSA à 15 ou 20h de travail agricole ou obligé hein de travailleurs privés d'emploi à accepter un travail saisonnier ne peut pas être l'horizon de la future entité France travail. Pensez-vous vraiment résoudre la question du départ à la retraite de la moitié des exploitants agricoles d'ici 10 ans avec ses solutions. D'un autre temps en faisant l'économie d'une réflexion sur les conditions de travail, les salaires, le sens du travail. La formation au lycée agricole les aides à apporter à l'installation de nouveaux agriculteurs ou encore la lutte contre l'accaparement des Terres agricoles par des financiers. Enfin, au moment où déjà au mois de mai 4 villages sont privés d'eau. L'an dernier 100 au coeur l'été et alors que nous avons vécu des méga-feux l'été dernier. Non ce n'est pas sérieux d'autoriser toutes les bassines, qu'elle soit méga de retenue ou de pompage. Oui, l'eau doit être reconnue comme un bien commun est sorti du secteur marchand. Enfin. Nous devrions nous rassembler pour refuser les accords de libre-, échange, non pas que nous ne voulons plus commercer, Monsieur le Ministre, mais nous voulons nouer des partenariats et des coopérations là où ces accords pousse à la concurrence et au moins-disant social et environnemental. Alors maintenant, le gouvernement dit nous voulons être exemplaires avec les clauses miroirs et refuser les produits qui ne respectent pas nos normes, nous en avons un bel exemple très concret. Pas plus tard que l'an dernier avec l'accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande. Si vous allez sur le site du ministère de la transition écologique. Vous pourrez lire que la France s'est dotée d'une stratégie pour mettre un terme à l'impact de ces importations sur la déforestation, c'est sur le site internet. Ensuite, dans la réalité c'est autre chose et ça ne pose aucun problème de signer des accords avec la Nouvelle Zélande 1er importateur mondial de tourteaux en Palm une monoculture, qui déforeste les forêts d'Asie du Sud-Est et tout ça sous la présidence française de l'Union européenne. C'est un dumping environnemental. Ou concrètement tolère et même pire on encourage ailleurs ce Colombien interdit chez nous. Toujours sur ses accords avec la Nouvelle-Zélande. Nous allons avoir des milliers de tonnes de viande brevet à l'atrazine et 10 Flubber Vérone des produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne depuis 2003 et 2021. Classé cancérigène et produits nos six. Voilà donc ce qui est pour l'instant les clauses miroirs, Monsieur le Ministre. À l'heure pour nous faire avaler c'est traité antisociaux et climaticide. Le seul effet de ces accords de libre-échange sur nos territoires en puisse d'organiser le dumping économique ces 2 pressurisé nos filières agricoles qui elles doivent respecter les normes qui sont nécessaires et nous pouvons être fiers. Mais qui les rendent moins compétitifs que n'importe quel produit cancérigène. Ce sont là des enjeux structurants pour notre agriculture est un enjeu démocratique car il y a bien un scandale c'est que le CETA s'applique à 90% sans justification du CETA ni de l'ensemble du Parlement. La dernière invention, la Commission européenne. Ce sont ces accords nouvelle génération qui ont des impacts sur nos services publics sur nos barrières tarifaires et non tarifaires. Et le Parlement est tenu à l'écart de ces négociations top tout comme il est empêché de voter sur le CETA par ce gouvernement, qui refuse toujours de l'inscrire à l'heure du jour du Sénat. Alors dans le calme. Je vous fais une dernière proposition, puisque ce projet sur le bureau du Sénat et qu'une sommes tous opposés alors vous reprenant le dans une niche jaloux et votons contre selon un double effet, premièrement, redonner du pouvoir au parlement si souvent piétinée par ce gouvernement, et deuxièmement nous rendre un grand service aux agriculteurs en faisant tomber ce traité et en ouvrant une nouvelle ère pour nos relations commerciales. Nous y sommes prêts. Alors chiche. Pour le reste, nous voterons contre ce projet de loi. Cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue monsieur le sénateur Pierre Louÿs au pour le groupe Union sans. Triste. Et vous avez 7 minutes. Chers collègue vidange. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Après la réalisation du rapport d'information sur la compétitivité de la ferme France. Que nous avons réalisé avec mes collègues Serge mais Riou et Laurent Duplomb. Il nous a semblé nécessaire de. D'aller vers une loi d'aller vers une loi tout simplement pour essayer de réparer un peu l'agriculture qui est dans une situation alarmante. Je tiens à saluer le travail de la qualité et plusieurs heures de débats sur le texte en commission. Madame. La rapporteure. Ce projet de loi été déjà amélioré déjà amendé. On a reçu même lors du débat ici dans cette assemblée. Écoutez le ministre de l'Agriculture. Moi je dirai à Laurent Duplomb. Il y a toujours moyen de voir une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Je pense que le ministre a été plutôt dans le bon sens même. Il a quelques réserves. Et je veux saluer son travail de collaboration, mon cher Laurent. Madame la présidente, par tout le travail, les rapports éclairé sur cette proposition de loi perfectionné au sein. De de la commission des des affaires économiques. Nous. Nous vous avez permis d'apporter une proposition de loi qui est qui a bien évolué. Cependant, je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Qui font tant débat étant de critiques. On nous dit qu'on revient sur le cadre normatif. On nous dit qu'. Il ne faut pas. S'occuper des lois européennes mais faire des sur-surtranspositions. Je crois qu'un des mals principaux de notre agriculture. C'est effectivement le cadre normatif, ce sont les. Transposition qui ont été faites avec beaucoup d'anticipation. Et je crois que les agriculteurs sont un peu comme les entreprises françaises. Ils n'en peuvent plus de cette réglementation, à n'en plus finir. Même le président de la République dit, il faut réduire le débat préalable aux travaux à deux ans et non pas partir à trois, quatre, six ans, 10 ans pour avoir un bâtiment d'élevage ou pour réaliser une retenue colinéaire. Je crois que fait fureur réglementation tous les agriculteurs sont atteints. J'ai eu l'occasion, j'ai dans ma famille des producteurs bio. Je puis vous dire que les producteurs bio en arboriculture n'en peuvent plus de cette sur-. Transposition parce que quand il pleut il faut protéger. Avec des produits bio. La production, hé bien ils ont été interdits par une loi. Scélérate, on veut toujours en faire plus. Dans l'imbécilité. Ces producteurs n'en peuvent plus, ils n'avaient pas le droit de traiter donc il devait fait disparaître leur production. Et je crois que c'est un peu ça, tout le débat, il y a quand même des exemples sur cette terre. Ou on s'imagine. Qu'avec les méthodes où il y avait un million d'habitants, un milliard d'habitants, on peut nourrir 8 milliards d'habitants. Le Sri Lanka a été cité en exemple par vous tous ou à là quelques années. Ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, la production annuelle avait diminué de moitié. Et un tiers du pays subissait la famine. Revenons aux réalités. Si ça ne vous dérange pas. Et pourtant. Et pourtant. Je crois pouvoir vous dire que je suis très favorable à une évolution. Vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Avec des nouvelles méthodes, mais les nouvelles méthodes ne sont pas forcément de copier ce qui se faisait au XIXe siècle. Les nouvelles méthodes. Vous voulez réfuter. l'évolution de l'agriculture viendra de l'évolution des technologies. De l'évolution de la Résistance variétale. Tout cela vous ne voulaient pas en entendre parler. Et je crois que c'est véritablement le problème d'aujourd'hui. 2ème problème qui a été critiquée, le volet fiscal. Le volet fiscal. Et pour tous les producteurs, les producteurs bio comme les autres parce que chacun a besoin d'investir pour trouver les nouvelles méthodes de production Ils ont une. Des recettes tellement insuffisante qu'ils ne peuvent plus investir et c'est essentiellement le problème. Et l'idée. D'avoir une épargne. Qu'on consacrée aux agriculteurs, je l'espère permettra de rapprocher. Les agriculteurs de l'ensemble des habitants du pays. Je crois qu'il faut également encourager l'innovation. La productivité la production de l'environnement. Pourquoi vouloir être systématiquement contre la productivité. Pourquoi vouloir être systématiquement contre l'utilisation de l'eau. Alors que. Depuis 10 ans, ces gouvernements, 20 ans même ces gouvernements s'acharne à ben les rivières à sec et vider les nappes par siphonage et aujourd'hui. On a mis le feu. On crie au feu. Eh bien je crois que il faut aussi un peu moins de doctrine et un peu plus de réalité si nous voulons pas fait l'été prochain à boire de l'eau pour tous les habitants français et toute l'agriculture. Un petit mot des salariés agricoles. J'entends bien qu'il ne faut pas remettre au travail. L'ensemble des salariés. Et pourtant. Vous avez la mémoire courte, je voudrais vous citer l'international ouvriers et paysans. Nous sommes le grand parti des travailleurs l'appartient. La terre n'appartient qu'aux hommes. Loi vif ira loger ailleurs. nous vous proposons tout simplement de donner l'occasion aux oisifs de revenir au travail et à participer à la nourriture de la nation. Enfin. Et je vais essayer de faire did. D'une manière plus générale. Cette passion qui nous anime tous dans ce débat, ce texte témoigne de l'importance que l'Assemblée accorde à l'agriculture et à la compétitivité de la compétitivité de l'agriculture et je salue tous. Tous ceux qui y ont participé. Merci à vous. Merci cher collègue. La parole est à présent à monsieur Jean Louis Masson pour 3 minutes au titre du des non inscrits.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Aussi bien pour des raisons de forme que de fond. Je suis assez réservé sur cette proposition de loi. Sur la forme, tout d'abord, j'ai constaté que le site du Sénat qui a pourtant un caractère officiel présente cette proposition comme étant transpartisane. Certes, dans les médias cette terminologie est à la mode. Cependant si on utilise la terminologie de manière officielle sur le site du Sénat. Encore faut-il qu'alors tous les sénateurs aient été traités sur un pied d'égalité en ayant eu la possibilité de s'y associer. Or je constate que sur les 175 signataires de cette proposition. 166. Soit la quasi-totalité appartiennent aux 2 groupes LR et Union centriste. À titre personnel, je n'avais par exemple pas été informé de cette démarche abusivement qualifié de transpartisane. En réalité, c'est donc une proposition de loi plus partisane que transpartisane. Par ailleurs. La procédure du scrutin public solennel est en général utilisé pour les projets de loi très important et je suis sûr pluri-qu'une simple proposition de loi faussement qualifiés de transpartisane on bénéficie. Certes, dans quelques mois, nous aurons des élections sénatoriales et ceci explique peut-être cela. Sur le fond maintenant. Cette proposition juxtapose des mesures ponctuelles, je reconnais bien volontiers que certaines sont assez intéressantes. D'autres ont par contre un caractère un peu politicien. Ainsi, quand on veut étouffer une affaire on crée une commission. De même, quand on veut créer du vent médiatique on désigne un haut-commissaire. C'est sans doute pour cela. Pour ce vent médiatique que l'article 1er de la proposition crée un Haut commissaire auprès du ministre de l'Agriculture. Ce haut commissaire sera-t-il un magicien qui va régler tous les problèmes de l'agriculture. De plus, à quoi sert le ministre de l'Agriculture. S'il faut encore lui adjoindre au commissaire. Monsieur le Ministre, à votre place je serais très inquiet. Vous allez vous retrouver au chômage. Donc il est temps Monsieur le Ministre, de réfléchir un petit peu à quoi va servir ce haut commissaire et je m'inquiète pour vous Monsieur le Ministre, vous voyez. La parole est donc à présent au sénateur Henri Cabanel pour le groupe RDSE. Mon cher collègue, vous avez 7 minutes de temps de parole. Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Madame la présidente de la commission et madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous voici réunis une fois encore, je n'ose veux dire une fois de plus pour parler d'agriculture. Une fois posé le constat amer de son déclin. Ce texte, analyse les causes et qui sont multifactorielles charge excessive surtransposition. Coût de l'innovation. Avec une absence de politique transversale depuis très longtemps.

La santé publique, la valeur partagée, la protection de l'environnement, le foncier, la préservation de la ressource ou le maintien de métier dans le délocalisable la transmission l'adéquation à l'évolution des goûts échoué des consommateurs la sauvegarde des paysages tous ces enjeux mérite d'être étudiée dans leur interconnexion. Les dissocier, comme cela a été fait conduit inévitablement à des politiques morcelé qui. Effectivement font oublier la compétitivité. En face, c'est le cas au niveau syndical mais aussi au niveau politique on oppose souvent l'écologie à l'économie. Dont débat trop souvent cliver en témoigne. Je suis convaincu que c'est une erreur, les politiques agricoles ne doivent pas être conçu par le petit bout de la lorgnette. En effet, le constat de réchauffement climatique. L'annonce de milliers d'espèces d'oiseaux disparus ou menacés nous oblige à revoir nos modes de production et de consommation. Concernant la rareté de l'eau, la situation de virer une très tendue dans nos territoires du sud. Les communes sont régulièrement ravitaillés en eau potable. Le, les préfets ont déjà pris à ce jour des arrêtés pour limiter certains usages, on ne peut l'ignorer. Il faut raisonner globalement la gestion de l'eau hein. Sachant que l'agriculture n'a besoin car et est source de vie, y compris l'agriculture bio. Le triptyque santé économie et environnement doit être au coeur de nos argumentations. Il a d'autres, ils doivent être prises en considération. Ensemble, nous avons un devoir moral envers les générations futures. C'est complexe mais possible et caricaturé modère un modèle qualitatif a le limitant à dénicher lui faisant peser le poids du déclin agricole n'est pas entendable. Je suis persuadé qu'il y a la place pour toute forme d'agriculture à condition que celle-ci soit sincère et répondent aux enjeux. Quand je pars de sincérité, je pense au bio qui a suscité un engouement face aux et à des et à l'évolution de la PAC qui s'est le bio traverse aujourd'hui la même crise que l'agriculture conventionnelle et de nombreux agriculteurs pensent à revenir à leur ancien mode de production. Car leur leur sur le le seul fil ici et le volet économique. Ce serait une erreur. Si l'on a une Pierre, les 2 autres indissociable d'jeu que sur la santé, l'environnement, les gouvernants ne doivent votre soutenir cette filière, le temps de la crise conjoncturelle. Je l'avais dit précédemment, et cela avait pu choquer mais les organisations professionnelles doivent également se soutirer et se solidariser. En France, dans le secteur du lait par exemple que je connais bien, il n'y a pas de stratégie nationale seul par bassins viticoles et même certaines appellations de même territoire se concurrence entre elles dans un contexte de crise ne pouvons-nous encore nous offrir ce luxe. Ne pouvons-nous pas mettre autour d'une table comme l'ont fait nos voisins espagnols et italiens pour élaborer des stratégies communes et offensive. Enfin, s'agissant du partage. Comment peut-on imaginer en prenant en contre un, un corps pardon. L'exemple de la filière viticole vaine. Ce qui se se Van la sortie de caves à 75 centimes le litre et se retrouve à 5 euros le verre de quel centilitres dans nos restaurants. Cherchez l'erreur. Et cet exemple homo pour plusieurs filières agricoles. Tout le monde doit gagner de l'argent à condition que la valeur soit partagé et ce n'est évidemment pas le cas, qu'on mange. Ce texte va-t-il améliorer cette problématique. J'ai l'impression que le morse que le que le morcellement dans les politiques agricoles largement critiqué et reproduit ici et que les auteurs ont fait des propositions. Avec le seul la compétitivité et donc essentiellement de l'économie. Où sont les autres enjeux pour détailler le texte le RDSE se réjouit de plusieurs avancées, notamment sur les clauses miroirs la transposition, la création de livret Agri le diagnostic agricoles sur les exploitations. Inutile de vous dire ma satisfaction concernant l'article 8 bis préconisant un rapport de bilan exhaustif relatifs au PSE. Hein pour services environnementaux avec mon collègue Franck Montaugé, nous avons cessé d'expliquer depuis 2016 les services rendus par les agriculteurs stockage du carbone, lutte contre les incendies via le pastoralisme, ouverture des espaces maintiennent des paysages. Ceux-ci doivent être prises en compte et. À l'inverse je déplore l'article hein. Je ne comprends ni la volonté ni l'asile nécessité d'avoir défendu la création d'un Haut Commissariat à la compétitivité des filières agricoles, alors que ce même texte du doigt la complexité administrative et prône la simplification on vient rajouter une couche au ministère de l'Agriculture au conseil général de l'agriculture et au Sham droit et culture. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Cela signifie-t-il que ces structures n'ont pas de vision prospective. Pas d'objectif sur la compatible. si c'est cela, c'est grave car c'est le coeur même de leur mission, établir des évaluations et des stratégies. De même à l'article je me choque car il revient sur la loi Egalim a déclaré en décalant l'échéance de 2022 à 2025 sur les produits de qualité durable domaine % de bio alors que nous n'avons pas assez de recul. La solution ne serait-elle pas plutôt la relance des projets alimentaires territoriaux qui structuraient la demande et l'offre locale autour de ces objectifs de qualité. Dans l'Hérault par exemple, un des départements précurseur, ces objectifs sont presque gagné grâce au 10 AT dont. Départemental. Ah au fait je m'étonne de l'article 18 qui réhabilite le conseil et la vente de produits phyto-sitôt pharmaceutique. Qu'un peu temps qu'être à la fois juge et partie. Pour toutes ces raisons je m'abstiendrai comme la grande majorité de mon groupe. Ce texte, nous le savons et politique puisque la loi d'orientation agricole se profile, c'est autant qu'elle prenne en compte tous les enjeux et je répète tous les enjeux. La bataille se jouera pour penser des actions cohérentes qui répondent. Enfin je l'espère, je vous remercie. public solennel sur la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France. Je vous invite à insérer des à présent votre votre carte de vote dans le terminal. Et Ali laisser jusqu'à la fin du vote qui va être ouvert dans quelques instants. Le vote est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Pas de problème a soulever parfait. Le scrutin est donc clos.

Voici le résultat du scrutin numéro 280 ans sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Nombre de votants, 332. Nombre de suffrages exprimés, 304 pour l'adoption de 10 contre 94. Le. Sénat vient donc d'adopter la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France. La parole est à monsieur Marc Fesneau Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté plaît. La parole est au ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, chers collègues. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs.

qui a permis d'éclairer un peu les débats et de préparer cette pépé. Alors on a eu des débats. On n'a pas toujours été d'accord, Monsieur Duplomb. À vrai dire c'est le la vertu démocratique mais vous dire je trouve bien qu'on a eu ce débat parce que sur le sujet agricole. On a souvent trop de non-dits et pas assez de choses qui soient mises sur la table et explicite et parfois on a cru qu'il y avait des tas de consensus et à la vérité, il y a besoin de dire un certain nombre de choses. La 2ème, chose que je voulais dire tu rassurez-vous je ne serai pas long c'est qu'on a besoin de. Pour avancer sur l'agriculture de science et pas de posture de respect et pas de mise au ban de progrès et pas de crainte du progrès. Je ne vois pas pourquoi le secteur agricole serait le seul qu'on priverait des moyens du progrès technologique et technique. C'est quand même assez original de trouver que alors que le monde agricole a été le 1er à bénéficier du progrès technique, on va lui à chaque fois qu'il y a un progrès technique sur les variétés. Sur les drônes sur autre on lui dise non. Vous, vous n'avez pas le droit au progrès technique quelque chose d'assez offensant, je le dis au passage. Deuxièmement, on a besoin. Troisièmement, on a besoin de solutions et pas d'injection de de. D'injonction. Et trois, on a, on a besoin de réel et pas de posture et sur le réel. La vérité m'oblige à dire. Que la ferme France. Elle a perdu en compétitivité en souveraineté. Alors on peut toujours aller chercher les causes à l'extérieur des frontières. Le sénateur. C'est un débat que nous avons ensemble à évoquer la question du libre-échange mais ça n'expliquera jamais pourquoi nous sommes le seul pays d'Europe où quasiment le seul pays d'Europe qui a perdu en souveraineté. Donc on a besoin de réfléchir au fait que pourquoi pourquoi la France elle même a perdu en souveraineté et pourquoi elle a perdu en compétitivité et c'est en cela que c'était intéressant sur ce sur ce point sur ce débat. Alors on a avancé. Moi je crois ces dernières années. Pas que sous les gouvernements depuis 2017 mais je pense que la loi Egalim a est un jalon important sur la question de la rémunération. La question des AT qui c'est ce sénateur la qui auquel vous tenez comme moi c'est profondément. Il y a quatre Il y en avait 20 en 2019 et c'était une loi de 2014, on a quand même progressé, reconnaissons qu'on a pu progresser sur un certain nombre de sujets et sur un certain nombre de plans de souveraineté, enfin je voudrais dire une chose, c'est qu'on a besoin aussi de dire attention au discours que nous tenons sur l'agriculture et j'ai trouvé qu'ici au Sénat, nous avons essayé de ne pas être. Dans la caricature du sujet agricole attention au discours que nous tenons vis-à-vis des agriculteurs. On a besoin des agriculteurs d'abord pour nous nourrir et ça n'est pas un chemin qui est derrière nous. L'idée que nous avons résolu notre problème pour la nuit des temps est une erreur et une une erreur funeste. Tant d'un point de vue j'ai végétal que d'un point de vue animale En France comme jusqu'à la rue Cambon. On a besoin de souveraineté alimentaire, on a besoin de souveraineté alimentaire, y compris d'un point de vue de l'élevage. Parce que tant qu'on importe des produits d'élevage qui viennent de l'extérieur de nos frontières. On ne me fera pas croire qu'on a besoin d'en rabattre sur cette question de production et on a besoin de dire aux éleveurs qu'on a besoin de on a besoin d'eux pour nous nourrir mais on n'a pas besoin de, que pour nous nourrir parce qu'on a besoin d'eux pour maintenir les prix Rist qui est du carbone. On a besoin d'eux pour maintenir les on a besoin d'eux pour entretenir les paysages. On a besoin de, pour lutter contre l'incendie. Donc l'ensemble des fonctions et des aménité comme on dit, on a besoin de leur dire et de cesser cette permanente chasse qu'on fait

de la place que nous entendons redonner à l'élevage et d'arrêter en permanence sept l'autre stratégie mortifère qui est la stratégie. Non pas de la baisse de la consommation mais de la baisse de la souveraineté. Parce que c'est ça ce qui se passe et quand vous regardez la cour c'est ça ce qui se passait donc je suis très heureux. Monsieur le sénateur du plomb parce que c'est plutôt avec vous qu'on avait changé, mais avec vous tous. Dans cette soirée. Avec vous tous ces sénateur vous inquiétez pas, j'ai bien noté que vous étiez là. Vous allez pas vous plaindre. Pour une fois ce n'pas vous que je regarde. Sinon vous avez le sentiment que c'est vous que j'attaque mais j'ai trouvé utile que nous ayons ce débat mais nous avons besoin. Nous avons besoin sur ce débat agricole de regarder lucidement. La situation de l'agriculture française. Et donc il faut arrêter de dire que tout va bien. Et donc on a besoin de reconquérir cette souveraineté et nous sommes collectivement. Et nous sommes collectivement en échec de cette question de la souveraineté, donc on a besoin de regarder. Ça avec lucidité sans injonction et c'était bien l'objet de ce texte, il y aura d'autres itérations d'initiative parlementaire évidemment d'initiative gouvernementale au travers du projet de loi d'orientation et c'est à ce rendez-vous là que nous devons être à la fois pour les agriculteurs et les agricultrices. Pour l'agriculture mais aussi parce que la souveraineté alimentaire c'est aussi important que d'autres formes de souveraineté énergétique industrielle ou militaire. Merci à toutes et à tous. Merci, monsieur le Ministre. Je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

Chers collègues, la séance est reprise. La parole est à madame Brigitte de VISA pour une mise au point, au sujet d'un vote. Oui madame la présidente. Merci de me donner la parole effectivement sur le scrutin public qui vient d'avoir lieu sur la ferme France je voulais voter pour donc. Acte est donné de votre mise au point le figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés entre 1933 et 1945 la procédure accélérée a été engagée Bonjour, madame la Ministre, dans la discussion générale. La parole est à vous. Donc je vous cède la parole.

Madame la présidente. Madame la rapporteure chers Béatrice Gosselin mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Il y a 80 ans. En Europe. Le pouvoir nazi et les autorités de collaboration ont confisqués aux juifs leur bien avant de s'en prendre à leur vie ou de les contraindre à la clandestinité à l'exil. Il y a 80 ans en France même, il a été décidé que les possession des juifs pouvait leur être enlevés. Souvenirs, objets du quotidien. Livre. Autant de biens spoliés et pillé par centaines de milliers qui n'ont pu être retrouvés et rendus. Les Oeuvres et objets d'art non pas échapper à ce destin. D'abord par la main de l'Allemagne nazie puis avec la complicité active de l'État français. Par le biais de son Commissariat général aux questions juives. Les galeries d'art ont été à réaliser. Les biens des professionnels et des particuliers ont été spoliés. Dans d'autres cas, les familles persécute. N'ont eu d'autre choix que de fuir en vendant sous la contrainte leur bien pour financer leur survie ou leur exil forcé. Derrière chaque oeuvre. Il y a une histoire familiale. Derrière chaque spoliation. Il y a un drame humain. À chaque restitution. C'est un acte de justice qui est rendue. Ce chemin de justice. Nous devons continuer à le tracé. Alors que les derniers témoins de la Shoah sont encore parmi nous. Plus pour longtemps et que l'antisémitisme n'appartient toujours pas au passé. En 1995, le discours du président Chirac au Vélodrome d'Hiver, a reconnu la complicité de la France dans la déportation et l'assassinat des Juifs de France. Au cours de l'occupation du pays par les nazis. En 1997, la mission Mattéoli a levé le voile sur le sujet longtemps oubliée des spoliations des juifs de France en dénombrant les avoirs en déshérence dans les banques et les compagnies d'assurance et en dressant un bilan des Oeuvres spoliées encore à la garde des musées nationaux. Ces recherches ont permis de rappeler que les spoliations participait de l'horreur du génocide puisqu'elle procédait de la même volonté de priver les victimes de leur individualité. Je voudrais si dire quelques-uns de leurs noms. Hugo Simon et Gertrud Simon. Contraint de laisser derrière eux leurs biens pour fuir au Brésil, loin de toute l'existence qu'ils avaient reconstruite après leur première exil d'Allemagne en 1933. 80 ans plus tard, lorsque leur arrière petit fils Raphaël Cardoso s'est vu restituer le tableau nu dans un paysage de Max Pechstein, il a prononcé ces mots. Notre souhait est que cet objet Servent à raconter l'histoire de nos aïeux et de tout ce que l'Europe a perdu au nom du délire de la pureté raciale. Nous désirons aussi que cette restitution puisse ouvrir une voie plus saines pour les relations entre les institutions culturelles et les familles spoliées. Le mot allemand pour la réparation, disait-il videur marron qui veut littéralement dire rendre bon de nouveau exprime parfaitement l'esprit que. De ce que nous pouvons réussir quand nous nous consacrons ensemble à réparer l'irréparable. Nos races Tiznit déporté et assassiné en 1942 avec sa mère, comme son mari et son fils qui vend pour presque rien, c'est bien à des faux amis qui travailleront sa confiance sans parvenir pour autant à échapper au sort tragique qui l'attend. L'année dernière grâce à la loi portée par Roselyne Bachelot, que le Parlement a adopté à l'unanimité nous avons restitué à ses ayants droit rosier sous les arbres tableaux de Gustav Klimt dont elle avait dû se séparer pour tenter en vain de fuir l'Autriche en 1938 années de l'Anschluss. Mathilde Javal dont l'appartement parisien et pillé et dont les biens sont ensuite dispersés. Si plusieurs de ses biens ont été rapatriés en France après la guerre, ce n'est que plus de 70 ans plus tard que le lien a été fait entre elle et 2 de ses tableaux. Contacté par des généalogistes une de leurs ayants droit Marion a découvert en 2018. Ces tableaux et à travers eux le souvenir d'une famille qu'elle avait toujours recherché. C'est en contemplant ensemble ces Oeuvres au musée du Louvre que les descendants d'Adolf et Mathilde Javal se sont rencontrés pour la première fois. Gertrude et Hugo Simon nos racines et Hasni Mathilde avale et tout c'est non. Tous ces destins qui reste aujourd'hui encore anonyme. Ces destins. Nous devons sans relâche continuer à en chercher les traces. Cela signifie conduire les investigations nécessaires jusque dans les collections publiques ou cet héritage injustement spoliés et souvent méconnu. On estime à au moins 100.000 le nombre d'Oeuvres d'objets d'art d'instruments de musique spoliées aux juifs pour la seule France, aux côtés de millions de livres. Si beaucoup ont été restitués dans l'immédiat. Après-guerre d'autres n'ont pas retrouvé leurs légitimes propriétaires, certains sont passés de main en main jusqu'à se retrouver dans les collections nationales. réaliser piller spolier les biens culturels des juifs, c'était essayer d'effacer non seulement les être que l'on brise mais aussi leur héritage que l'on vole leur histoire, leur individualité leur postérité. Les réduire à un numéro sans voix. Sans bagage sans droit. Rien ne peut les ramener. Rien ne peut. Inverser le cours de l'histoire. Mais nous pouvons rendre possible la restitution de leurs biens culturels à leur famille à leurs ayants droit. Nous le devons aux victimes d'hier et à leurs héritiers d'aujourd'hui pour leur rendre un fragment d'histoire familiale pour que ce qui est juste ne soit plus un combat législatif sans fin. Mais en droit. La tâche est immense ardue car les spoliateurs sont aussi des dissimulateurs démêler cet écheveau de semblants dissiper les simulacres qui ont été forgé pour masquer l'origine d'une oeuvre volée exige non seulement une intense détermination mais aussi la mobilisation d'une somme d'informations de connaissance. D'une grande complexité pour déterminer les cas de vente forcée d'échanges suspects de saisie pillage d'aryanisation et parvenir à retracer l'itinéraire tortueux de ses Oeuvres. Ce que le législateur va permettre aujourd'hui. C'est l'historien qui l'a construit. Ces dernières décennies, de nombreuses études conduites en Europe et surtout en France et en Allemagne, ont mis au jour numérisé et mis en partage des sources d'archives qui permettent de lutter contre l'oubli. Nul ne peut désormais ignorer ces ressources. Je veux saluer dans cette enceinte, le travail de Madame Corinne Bouchoux sénatrice du Maine et Loire qui avec son rapport sur les Oeuvres culturelles spoliés a formulé en 2013 des propositions pour relancer le travail d'enquête. À l'occasion de la commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv en 2018, le Premier Ministre s'était engagé à faire mieux en matière de recherche et de restitution des Oeuvres d'art spoliées aux familles juives. À cet effet, nous avons créé en 2019, la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au sein du ministère de la culture pour piloter animé cette politique publique de recherche de réparation et de mémoire. Je veux ici remercier personnellement David Zivie et son équipe dont l'expertise et l'engagement mis au service des musées contribue justement à faire mieux. Longtemps, ces recherches se sont concentrées sur les Oeuvres récupérées par les alliés qui n'ont pu malgré bien des efforts, être restitués à des propriétaires restait inconnu. Elles ont été siglés et inventorié MNR pour Musées Nationaux récupération et confiés à la garde des musées en attente de leur légitime propriétaire ses Oeuvres lorsqu'elles sont spoliés peuvent être restituées de droit sans loi spécifique car elles ne sont jamais entrer dans nos collections publiques. Mais depuis la création de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés. Les recherches ont été étendues à d'autres types d'Oeuvres. Entrer en toute légalité dans les collections parfois bien des années, voire même des décennies après la guerre. Dans 2 cas sur 3, aujourd'hui 2 cas sur 3, c'est à l'initiative du ministère de la culture que les Oeuvres spoliées sont identifiés et restitués aux descendants. Ces restitutions ont tissé un lien entre les chercheurs et experts d'hier et ceux d'aujourd'hui, je pense avec émotion, notamment à l'héroïque Rose Valland qui attachée bénévole au musée du Jeu de Paume à inventorier clandestinement les Oeuvres spoliées qui étaient entreposées pendant l'occupation. Aujourd'hui c'est une nouvelle génération d'historiens qui s'engage avec détermination dans les recherches dans les recherches de provenance. Car il s'agit bien désormais d'expertiser les collections sur une toute autre échelle. Et de déceler les origines douteuses parmi les Oeuvres entrer dans les collections publiques depuis 1933. Ce chantier, les professionnels de l'art sont désormais prêts à le conduire et le ministère de la culture ne cessent de l'encourager ses préoccupations figurent aujourd'hui dans la formation initiale des conservateurs et des commissaires priseurs à l'École du Louvre à l'Institut national du Patrimoine et depuis 2022 dans un nouveau diplôme de l'université Paris Nanterre spécialisé dans la recherche de provenance. Pour autant, lorsque ces longues et difficiles recherches aboutissent lorsqu'une oeuvre spoliée et repéré comme tels dans les collections publiques lorsqu'on a identifié les propriétaires lorsque toutes les parties s'accordent sur le principe de la restitution, il reste impossible de la restituer sans passer par une loi spécifique pour déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Or, cette loi ne peut intervenir qu'après une certaine attente au terme d'un processus législatif nécessairement long. Prenons un exemple, celui de Georges Bernheim ce galeriste d'avant-guerre merveilleux découvreurs des grands artistes modernes. Dont les biens furent spoliés pendant l'occupation en 2018 l'un de ses tableaux volés a été retrouvée dans les collections du musée Utrillo Valadon de la ville de Sannois. Toutes les parties prenantes était d'accord pour le restituer la ville de Sannois qui en était propriétaire l'ACI vs la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. Le ministère de la Culture les ayants droit bien sûr mais pour que l'oeuvre soit restituée. Il a fallu attendre 4 ans. 4 ans pour qu'une loi d'espèces présenté par Roselyne Bachelot dont je veux saluer la détermination soit votée. Aujourd'hui, dans la lignée de la politique volontariste que nous menons depuis plusieurs années nous souhaitons par cette loi offrir un horizon légales, claires et juste aux démarches de restitution afin que les Oeuvres spoliées conservés dans les collections publiques puissent être restitués sans délai supplémentaire sans perdre des années à chaque fois. Toutes les collections publiques seront concernés, qu'elle soit dans des musées nationaux relevant du ministère de la culture dans des musées territoriaux des établissements publics non muséaux, qui détiennent des collections ou encore dans les bibliothèques. Avec cette loi lorsqu'après enquête, la spoliation aura été reconnu par la commission consultative indépendante et par le propriétaire public quel qu'il soit la restitution de l'oeuvre se fera de droit. Pour l'État, un décret simple de la Première ministre suffira pour les collectivités. Une décision de l'organe délibérant. La commission consultative chargée d'apprécier l'existence et les circonstances de la spoliation sera la Commission pour pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation la ACI vs. La CIV est qui a prouvé depuis sa création son expertise sa légitimité. C'est en effet l'organe aujourd'hui, spécialisée dans l'appréciation des faits de spoliation. Elle examine les faits de vols de pillages d'aryanisation ainsi que les ventes contrainte et peu recommander à la Première ministre des mesures de réparation. Si ces faits constituent des spoliations antisémites. Si cette loi traite du passé des biens déjà entré dans les collections. Elle s'impose par voie de conséquence aux futures acquisitions lorsqu'il ne sera pas possible de déterminer avec certitude la trajectoire d'une oeuvre acquise pendant la période 1933 1945. Celle-ci ne devra pas entrer dans les collections publiques. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Ce projet de loi et le premier depuis la Libération qui reconnaît la spoliation spécifique subies par les juifs en France et partout, du fait de l'Allemagne nazie et des diverses autorités qui lui ont été liées. En vous proposant aujourd'hui d'ajouter 4 articles dans le code du patrimoine. Je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre du rapport que nous entretenons avec notre histoire. Dans le sens de la justice dans le sens de la vérité historique. Sous l'impulsion des chercheurs et sous réserve de l'avis de la CIV s chaque bien culturels précédemment spoliés est entrée par la suite dans les collections publiques pourra être restitués aux ayants droit de son propriétaire originel grâce à cette loi cadre. Nous élargissons le Champ de compétence de la CIV S pour qu'elle puisse traiter des dossiers de spoliations antisémites intervenu entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et non pas seulement pendant l'occupation. Quel que soit le lieu de spoliation parce que même volé à l'étranger des Oeuvres spoliées peuvent se trouver aujourd'hui dans une collection publique française. Telle est désormais la portée de cette nouvelle ambition qui nous engage et nous oblige. L'année de la mission Mattéoli. En 1997, Patrick Modiano écrivez dans Dora Bruder. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière, ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés et quel gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à voulait montrer ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres exister. En écrivant ce livre, je lance des appels comme des signaux de phares. Dont je doute, malheureusement, qu'il puisse éclairer la nuit. Chercheurs, historiens association descendants des familles généalogiste élu. Ils ont été nombreux à entendre ces appels et nous ont aidé à éclairer la nuit. Rien ne saurait réparer la tragédie de la Shoah. Rien ne saurait rendre aux familles les objets du quotidien massivement spoliés et pillé qu'il est matériellement impossible de restituer à des hommes, des femmes, des enfants, que l'État français a livré en collaborant avec le régime nazi. Mais il est de notre responsabilité. De faire tout ce qui est en notre pouvoir pour opposer la justice à la cruauté au cynisme à l'ignominie. Ce chemin de justice a été ouvert par les résistants. Dans le maquis à Londres en Afrique du Nord, mais aussi dans nos musées ouverts par Rose Valland ouvert par tous ceux, toutes celles qui se sont battus pour rendre les restitutions possible. Avec cette loi, nous rendons hommage à leur engagement et nous nous en montrons digne je vous remercie. Merci madame la ministre. La parole est à présent à madame Béatrice Gosselin, rapporteur de la commission de la culture de l'éducation et de la communication et vous avez 10 minutes, chers collègues. Madame Madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues. Certains moments législatif sont empreints d'une seule annuités et d'une émotion particulière. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en état. Si le rôle du législateur n'est pas d'écrire l'histoire, il peut être de sa responsabilité de faire en sorte de panser certaines plaies du passé. Les spoliations de biens culturels font partie des crimes de la Shoah, pour lesquels nous conservons une dette imprescriptible pour reprendre les mots prononcés par le président de la République Jacques Chirac en 1995. Elles ne peuvent être dissociées. De la politique d'extermination des juifs d'Europe mises en oeuvre par le régime nazi et ses complices. Une politique à laquelle le régime de Vichy a pris toute sa part. En privant ces personnes de leurs Oeuvres et objets d'art de leurs livres ou de leurs instruments de l'Unédic, c'est bien leur dignité, leur culture, leur histoire et leur identité qui leur a été retirée. Même si ces crimes sont irréparables. Nous pouvons nous devons même. Faire oeuvre de justice et d'humanité en corrigeant ce qui peut l'être. En visant à faciliter la restitution des biens culturels spoliés conservés dans nos collections votre projet. Madame la Ministre, ils contribuent de manière indiscutable. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la première loi de restitution des biens spoliés que nous avions votée l'an dernier. Nous avions alors unanimement souscrit à la nécessité de lever Linda ni un l'inaliénabilité à la fois par devoir vis-à-vis des victimes, mais aussi par nécessité pour nos collections tant que nous sommes tous d'accord que c'est bien n'y ont pas leur place. C'est pourquoi la commission accueille très favorablement le principe d'une loi cadre. Nous sommes en effet convaincu que le devoir de mémoire et de réparation nous commande d'accélérer le rythme des restitutions avant que la mémoire des familles de victimes ne s'estompe ou que les recherches s'avère impossible. La France doit prendre des mesures fortes pour garantir que soient trouvées des solutions justes et équitables au spoliation de biens culturels confisqués par les nazis. Conformément aux principes de Washington. Adoptée en 1998. De ce point de vue l'adoption d'une loi cadre nous paraît préférable au vote d'une multitude de loi d'espèces. D'abord parce que c'est un vrai symbole de notre engagement à aller plus loin sur le chemin de réparation des spoliations antisémites. Mais aussi parce que c'est une réponse de long terme global fiables et transparentes aux problèmes soulevés par ces spoliations sans nécessiter d'autorisation au cas par cas du Parlement. Nous voulons aussi croire que les perspectives plus tangible de restitution offerte par une loi cadre contribueront à mieux sensibiliser des acteurs culturels à l'enjeu des spoliations et à intensifier les recherches proactive aujourd'hui trop modeste. Nous sommes conscients. Que la complexité et la lourdeur de la procédure parlementaire peuvent aujourd'hui découragé certains établissements de s'investir dans ses recherches dans la mesure où ils n'ont pas la certitude qu'elles aboutiront à une restitution au moins à brève échéance. J'en viens maintenant contenu du projet de loi. Le texte crée une procédure administrative permettant à l'État et ou aux collectivités territoriales. Par dérogation au principe d'inaliénabilité de restituer des biens culturels appartenant à leur collection qui se révélerait spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés entre 1933 et 1945 et après l'avis de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations la CV la CIV. Sur l'existence de la spoliation et des circonstances. Cette procédure nous paraissent satisfaisantes à plusieurs titres. Déjà la réduction garantie que la restitution s'impose aux personnes publiques lorsqu'il est établi que le bien a fait l'objet d'une spoliation ensuite le périmètre de la procédure est suffisamment large pour qu'elle soit applicable à tous les types de biens culturels relevant du domaine public, y compris le mobilier, les livres et des instruments de musique mais aussi aux différentes formes de spoliation liées à des persécutions antisémites, quelle que soit la personne responsable et le lieu de leur perpétration. Enfin, le recours à la fille PS nous apparaît comme une comme une garantie d'un examen scientifique et impartiale des cas. Son Son expertise en matière de caractérisation des spoliations et reconnue et sa compétence en matière de biens culturels est désormais assurée depuis la réforme survenu en 2018. Il nous paraît donc opportun que son avis ne revêtent d'un caractère simple afin de responsabilité davantage les collectivités publiques et de conférer une plus grande dimension symbolique à la décision de de restitution. Le risque que son avis ne soit pas suivi semble de toute façon assez faible. L'une des innovations de ce projet de loi et la possibilité offerte aux parties de conclure un accord amiable sur des modalités de réparation, autre que la restitution. Une fois le principe de celle-ci obtenue par les victimes par exemple le maintien du bien dans la collection publique en contrepartie d'une compensation financière. Cette disposition est évidemment avantageuse pour la préservation des collections publiques comme l'a montré la transaction conclue par le musée, la branche de Brive-la-Gaillarde avec les héritiers d'un propriétaire. Propriétaire allemand spoliés. Elle pourrait aussi intéresser des familles de victimes en leur garantissant que demeure d'anciens lieux accessibles au public une trace mémorielle de la spoliation dont elles ont été via victime. qu'elles constituent une solution qu'elle constitue une solution juste et équitable, au même titre que la restitution. Puisqu'elle ne pourra en aucune manière être imposé et qu'elle préserve la reconnaissance de la spoliation et s'juste admis indemnisation. Il reste que sa mise en oeuvre pourrait néanmoins se heurter à une problématique financière compte tenu de la faiblesse des crédits d'acquisitions dont disposent actuellement les établissements. Ce qui soulève la question des moyens qui seront déployés pour garantir la bonne application de cette loi Madame la Ministre je reviendrai tout à l'heure. Un mot avant sur l'article 2 qui autorise les propriétaires des musées privés ayant reçu l'appellation Musée de France a restitué après la avis de la CEI vs les biens spoliés de leurs collections acquis pardon ou leg ou avec le concours financier d'une collectivité publique dans la mesure où ils sont en principe incessibles sauf à un autre musée de France. La commission est favorable à cette disposition. Non seulement elle permet de lever les obstacles juridiques qui pourraient bloquer la restitution de certains biens spoliés par des musées privés mais elle pourrait inciter les propriétaires de ces établissements engager des recherches sur la provenance de leurs collections. La commission a d'ailleurs adopté 2 amendements visant à il été là sa bonne application. Car c'est bien la mise en oeuvre du texte qui préoccupent notre commission. Si le projet de loi créé l'impulsion qui nous faisait défaut en facilitant la perspective des restitutions, il reste encore un immense travail à fournir pour que celles-ci puissent intervenir. Nous sommes convaincus que cette réforme ne pourra se passe effectuée à moyens constants, sans que les espoirs suscités par ce projet de loi soit immanquablement déçu. Malgré des progrès ces dernières années, l'engagement de la France en termes humains et financiers restent modestes en comparaison de plusieurs de nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne, dont l'État fédéral et les Länder ont consacré depuis 15 ans, plus de 40 millions d'euros en matière de notre recherche de provenance sur les biens spoliés. Si la mise en oeuvre du projet de loi nécessitera à coup sûr de renforcer les effectifs de la. Et de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés de votre ministère. Elle exige également d'intensifier le travail de recherche de provenance tant celui apparaît comme la clé de voûte des restitutions à venir. Il s'agit évidemment d'un travail titanesque complexe et chronophage qui requiert un personnel qualifié disponible. Nous ne pourrons pas y parvenir sans enrichir encore l'offre de formation en matière de recherche de provenance ni sans donner aux établissements de nouveaux moyens pour recruter des, des des chercheurs de provenance quitte éventuellement à envisager des recrutements mutualisés. Mais maintenant que l'obstacle législatif hors institution est en passe d'être levés. Nous ne saurions rester au milieu du gué. Même si le travail de recherche de provenance ne débouchera pas toujours sur une restitution tant l'éducateur l'identification des biens et des ayants droit s'avère parfois complexes. Elle constitue une exigence pour mieux rendre compte de l'histoire des spoliations et retracer le parcours des biens spoliés. le parcours des Oeuvres conservées dans nos collections pardon la médiation des biens spoliés fait partie intégrante de la politique de réparation. Elle est une autre manière de rendre aux victimes. Une part de leur vie, de leur histoire et de leur identité. Dans le cas où la restitution s'avère impossible, je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à présent à monsieur Jean-Pierre de col du groupe des indépendants et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. La question de la provenance des Oeuvres d'art exposée dans les bus dans les collections publiques est aujourd'hui un sujet majeur pour les musées français. Elle engage une profonde réflexion sur notre rapport à l'histoire à la politique mémorielle et la formation de notre Patrimoine culturel, nous sommes face à un vaste débat de société. Et celui-ci nous engage relativement. Au cours des décennies précédentes, l'humain était au coeur de la politique française de réparation des spoliations. L'heure était au recueille les témoignages et des récits transmis par les ultimes témoins du passé commissaire priseur fonctionnaire de l'administration conservateur de musée marchand d'art. Aujourd'hui, les biens culturels incarne l'histoire et sont porteurs de mémoire pour les générations à venir. Nous parlementaires avant le devoir de participer à la formalisation de la politique française de restitution, grâce à ce projet de loi. Au cours de la seconde guerre mondiale la déportation des juifs de France est accompagné du pillage méthodique de l'ensemble de leurs biens, notamment culturels. Dès l'été 1990, de nombreux domiciles de familles juives ont été vidés du sol au plafond de leur mobilier de leurs Oeuvres d'art de leurs instruments de musique. À Paris, première place mondiale du marché de l'art. Pas moins de 40.000 appartements ont été pillés. Les Oeuvres spoliées ont d'abord été stockés à l'ambassade d'Allemagne à Paris puis au Louvre et enfin au musée du Jeu de Paume. À partir du mois de novembre 1940. En France, on estime à 100.000 les Oeuvres volés ou vendus sous la contrainte. Un nombre sans doute sous-évalué. Il est en effet calculé en s'appuyant sur les signalements réalisé après la guerre par les familles. Toutes ne se sont pas manifestés. Après la guerre, 60.000 de ses Oeuvres sont revenus en France dont une grande partie a été rapidement restitués au propriétaire. Certains biens ont été vendus tandis que d'autres ont été confiées aux musées français. Oublié quelques années le sujet de la restitution des Oeuvres spoliées est revenue sur le devant de la scène, au milieu des années 1990, depuis une vingtaine d'années, le nombre le restitution augmente peu à peu. À l'image de la Vierge à l'enfant de la Vierge de pitié et de la scène de bataille siège de Carthage par Scipion Émilien rendu en avril dernier à leurs ayants droit. Malheureusement. Certaines Oeuvres n'ont pas encore retrouvé la propriétaire et patiente dans les salles d'Exposition de nos musées. Commence alors le rôle des historiens spécialisés leur longues enquêtes sont le travail de toute une vie. Il s'appuie sur un faisceau d'indices hétéroclite les archives nazies, les services administratifs de l'État collaborateurs les généalogistes les marques apparentes sur les Oeuvres elles-mêmes. Les prescriptions par les familles lésées. Je voudrais toutefois salué la mémoire de Rose Valland, attachée de conservation à Paris pendant l'Occupation figurative de la résistance à l'a pris de grands risques pour archiver l'ensemble des Oeuvres spoliées et conserver au sein du musée du Jeu de paume. Nous lui devons une grande partie des restitutions d'après-guerre. Aujourd'hui encore, nous devons affronter ce passé. Pour les Oeuvres qui appartiennent tous aux collections publiques, seule une loi spécifique peut autoriser leur sortie du domaine public en raison de leur caractère inaliénable. Pour faciliter la restitution et éviter de légiférer au cas par cas. Il est essentiel de prévoir une loi-cadre permettant d'aller plus vite, nous pouvons nous féliciter que ce sujet soit l'une des priorités du ministère de la culture. Ce texte pose également la question de l'après-restitution. Aucune compensation n'est prévue après la restitution de l'oeuvre. Les musées vont devoir se réinventer pour continuer à servir leurs murs les Oeuvres rendus aux familles. L'art numérique peut être une piste de réflexion intéressante. Je suis également favorable au fait d'encourager les familles volontaires à permettre au public d'accéder périodiquement aux biens culturels restituer ces différents sujets nourriront je l'espère de prochains débats. Mes chers collègues. L'historien Philippe des raids écrivez dans l'un de ses ouvrages que l'histoire des restitutions des biens juifs est une histoire qui reste à faire. La France en écrit aujourd'hui un nouveau chapitre. C'est un très bon signal que notre assemblée se prononce, de manière unanime sur ce sujet qui nous tient tant à coeur. Ce débat est essentiel au regard de l'immensité et de la complexité du défi de la restitution d'Oeuvres. Il doit se poursuivre dans les mois à venir. Le groupe les indépendants votera ce texte et s'en félicite. Je vous en remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein madame Monique de Marco du groupe écologiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure mais sa collègue. Comme l'écrivait la sénatrice écologiste Corinne Bouchoux en 2013 je cite. Le passé non assumé, ne se digère pas tout ce refoulement cet oubli, il faut en sortir. Certains actes continue à nous glacer le sang des décennies après qu'il a été perpété. On ne voudrait plus d'avoir à découvrir leur nom mentionné dans les documents législatifs. Et hélas les démocraties mettent des décennies à reconstruire ce que les régimes autoritaires détruisent en quelques mois. Pour toutes les victimes de la Shoah, leurs enfants, leurs petits-enfants. Un devoir de réparation nous incombe pourtant de manière imprescriptibles comme le sont les crimes contre une humanité qui auraient été perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourquoi tant que cela sera nécessaire, le Parlement devra prendre les actes nécessaires pour réparer, comme ici pour restituer les biens spoliés pas des actes antisémites en 1933 et 1945. Au-delà de l'aspect patrimonial d'avoir privé une personne de son héritage familial et culturel, c'est aussi le priver d'émotion artistique c'est le privé d'humanité. Nous ne devons pas sous-estimer les circonstances internationales de ses actes. En France les spoliations non pas seulement été le fait de nazis mais aussi 2 Français politique administratif anonymes qui ont écrit des qui, qui ont acquis des Oeuvres avaient des procédures dites de vol légal. Je voudrais saluer ici le travail de ceux qui se sont opposés dans les premières heures guidé par l'intuition de justice. Parmi eux des femmes je pense aussi à Rose Valland bien sûr qui élabore d'abord un 1er registre en 1940 au péril de sa vie. À partir de 19.145, promu Capitaine. Elles seront envoyés en Allemagne sur le front de l'art. Sur plus de 100.000 Oeuvres identifié 60.000 ont été rapportés en France et 45.000 restitués à leurs propriétaires ou leurs ayants droit dans l'immédiat d'après-guerre. Puis rien. Ou presque rien. 104 484 tableaux sur les 2000 tableau 10 musées nationaux de récupération seulement ont été restitués à leurs propriétaires en grande pompe médiatique. Après la conférence de Washington. Des travaux de Corinne Bouchoux que j'ai déjà cité ont enfin permis de relancer la question au Sénat. Nous écologistes, savons que le droit international est impuissant aussi de communication gouvernementale, mais un faible instrument juridique en droit interne. L'étude d'impact adossé au projet de loi confirme le constat de négligence des pouvoirs publics établi par Corinne Bouchoux. Après les années 50, le statu quo s'est imposé tant et si bien qu'il est impossible de dire aujourd'hui combien de biens culturels de nos collections publiques auraient été acquise dans des circonstances douteuses. Dans les collections publiques un énorme travail de recherche s'impose au delà des musées nationaux de récupération pour comprendre le parcours juridique d'appropriation des Oeuvres d'individus frappés par les lois série Cela nécessite également de levée des entraves comme l'accès aux archives nationales et de doter chaque font de moyens suffisants pour conduire ces recherches. Mais aussi pour identifier des ayants droit. Ce y compris pour les collections des collectivités territoriales ou l'initiative repose souvent sur la bonne volonté du du. Enfin notre intransigeance doit être la même avec le collectionneurs privés a fortiori là ceux qui bénéficient de largesses fiscales. L'article 2 pourraient être renforcées dans ce sens. Au-delà de ses limites. Je voulais saluer cette initiative gouvernementale. La procédure de sortie de biens spoliés des collections publiques Nestor lève le frein législatives aux restitutions avec un élargissement de la période historique de recherche. Mais quelle leçon pour l'avenir. Dans sa célèbre lettre au Capitaine Buetler. Victor Hugo écrivait. Les crimes de ceux qui mènent. Ne sont pas la faute de ceux qui sont menées. Les gouvernements sont quelquefois des bandits. Les peuples jamais. L'empire français étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du Palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France délivrée et nettoyée renverra ce butin à la Chine spoliée. Nous savons que seront exposés dans nos musées, les résultats d'autres massacres et pillages à nous à présent nous nous doter des moyens juridiques pour prévenir l'acquisition publique c'est bien d'origine douteuse. Sans eux, nous condamnons générations futures en de nombreuses lois de réparation. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Julien Bargeton pour le groupe RDPI. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, madame la rapporteure. Pour le 1er projet de loi que vous nous présentez la ministre vous. Abordez un sujet extrêmement douloureux solennel et grave je pense que c'est important que nous puissions nous pencher sur ce sujet aussi longtemps après. Dans la tête d'Obsidienne. Malraux dit que l'art et la présence dans la vie de ce qui devrait appartenir à la mort. Il fait référence à Picasso et aux traces qu'il laisse mais ce texte symboliquement je crois nous parle de ça de la façon dont l'art aussi. Transcende transmue le réel et que ce texte c'est précisément cela, la façon dont l'art et la présence dans la vie de ce qui devait, et devrait appartenir à la mort. Alors le moment est venu d'aborder ce texte. Le moment d'abord pourquoi parce que les archives n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi ouverte bien sûr depuis la chute. De l'Union soviétique, et puis aussi avec l'ouverture de toutes les archives et leur numérisation. Et puis les travaux scientifiques se sont également accélérer les États coopèrent de plus en plus sur le sujet de la restitution des biens juifs spoliés pendant les persécutions antisémites de 1933 1945, vous l'avez cité, évidemment le tableau de Klimt. Le rosier. Qui a pu être restitués après un travail en commun entre le musée d'Orsay et le Belvédère de Vienne avec une des intenses recherches et une couleur, une coopération entre ces 2 états qui a permis la restitution et puis les familles sont également peut être que l'éloignement de la Shoah finalement permet aussi et et que ce soit évidemment moins douloureux directement permet aussi d'insister sur la dimension de transmission de mémoire que joue aussi la restitution de ses. Collections, parce que c'est aussi la mémoire de la Shoah. Bien sûr elle même qui est, qui Le gouvernement avait présenté il y a 2 ans un projet de loi et c'était déjà la même rapporteur Madame Gosselin. Et vous aviez dit à l'époque que en effet à chaque fois. C'était long, s'il fallait des textes spécifiques parce que ça prenait un cheminement administratif et législatif assez laborieux et que donc il était temps d'élaborer une loi cadre que vous appeliez de vos voeux et qui. Arrive et puis il y a eu la création en 2019 de cette mission, cette mission de recherche et de restitution des biens juifs spoliés au sein du ministère de la culture et puis également évidemment le fait que le temps passe et que maintenant avec les la disparition des témoins Directs de la Shoah parfois le souvenir, la mémoire de telle ou telle oeuvre disparaît et que donc il est temps vraiment de pouvoir accélérer et de pouvoir restituer les Oeuvres dans de bonnes conditions et c'est pourquoi nous arrivons aujourd'hui à un consensus sur ce texte, ce n'est pas simplement une question symbolique, ce n'est pas simplement une question de justice, c'est aussi une question de réparation intime, en référence à ce que je disais sur le rôle de l'art. Je pense aussi au peintre Marc Roscoe. Peintre américain d'origine juive russe qui était partie bien avant la choix puisqu'il a quitté son père était parti avant. Il a rapatrié sa sa famille au stade unis en 1913. Mai marque Roscoe avait été dans son enfance traumatisée et profondément marqué par les pogroms et les massacres de juifs dans ce qui était à l'époque l'Empire russe. Aujourd'hui ce sont les pays baltes mais à l'époque c'était l'Empire russe et. Il le montre à quel point. Finalement c'est ce traumatisme a nourri son oeuvre et ses rectangles très vibrant de couleurs que nous lui connaissons. C'est une façon pour lui. De. Donner une énergie nouvelle à des tombes en fait on s'en rend pas forcément compte mais on peut chacun interprète les les Oeuvres comme il l'entend mais les oeufs l'oeuf de Marc Roscoe peut être interprétée aussi comme les tombes. Les tombes jamais fait pour ces victimes de pogroms dans l'Empire russe et qui la transmués en tableaux vibrant de couleur et donc d'énergie. Aujourd'hui c'est cela aussi à quoi nous devons penser parce que c'est d'abord des personnes qui avaient fait le choix de faire vivre l'art de faire de de de de se et nous leur restitution. Nous leur restitution leur mémoire de leur restituer leurs bien nous leur restitution aussi en échange le bien qu'ils avaient fait à l'art et aux artistes. Merci beaucoup. Merci cher collègue. La parole est à présent à monsieur Lucien stands Thione du groupe socialiste et vous avez 9 minutes, chers collègues. Dans la présidente. Madame la Ministre. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Je prends la parole aujourd'hui avec une émotion certaine pour aborder une question qui nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire, la spoliation des biens juifs durant l'Occupation, mais également depuis 1933. Vous l'avez cité tout à l'heure. Nous nous apprêtons à discuter d'un projet de loi historique héritage volé des biens ont été arrachés dispersés dans le monde entier. Leur inestimable valeur a été occulté par l'injustice. Plus de 80 après il est tente d'apaiser, de réparer, de rétablir l'équilibre et de redonner voix à cette histoire volé. Ses biens culturels qu'il s'agisse d'Oeuvres d'art de livres ou d'instruments ou d'instruments de musique qui était autrefois en harmonie avec l'âme de leur propriétaire. Mais voilà, les nazis, avec le soutien de l'État français de l'époque complices et acteurs ce soir à donner à des vols des pillages des confiscations abject des saisies sous couvert de l'aryanisation bercer d'antisémitisme le plus radical, ils ont fait des lois du Reich et des rafles une opportunité pour des plus dépouiller les juifs de ses trésors qui leur reviennent aujourd'hui de droit des familles entières ont été dépossédés des communautés ont été réduites au silence des vies ont été brisées. Tout cela au nom de la discrimination et de la haine. Nous nous souvenons tous des débats précédant l'adoption de la loi relative à la restitution des biens aux ayants droit. Les parlementaires de tous bords avaient alors exprimé leur volonté de trouver une solution législative durable. Il est donc temps mes chers collègues, de mettre fin à cette injustice persistante. Nous devons simplifier la restitution lever les barrières qui entravent leur retour légitime. Les procédures complexes ont compliqué les restitutions simplicité des démarches établissement de critères clairs engagement de délais raisonnables. Toutes ces mesures enverront un message clair. Nous reconnaissons votre souffrance nous honorons votre histoire nous rétablirons l'équité. Le contexte juridique entourant les biens spoliés et actuellement un labyrinthe complexe des 19.143 plusieurs ordonnances ont été prises par le gouvernement de Londres. Pour enfin prévoir la nullité de tels actes de spoliation. Un inventaire des biens spoliés a été dressé 1949 1000 était incomplet. De nombreuses institutions ont eu lieu à la suite de procédures de recherche cependant ces heures va spolier sont juridiquement enchaîné n'aliène imprescriptibles. Actuellement il existe 2 moyens de restitution. Une procédure de nullité de l'acte de spoliation devant les tribunaux judiciaires et une ou une décision du juge administratif ou judiciaire de restitution des biens classés Nm Le présent projet de loi propose d'introduire 3 nouveaux articles dans le code du patrimoine pour faciliter la restitution, le premier article crée une dérogation de précise des naines habilité des biens publics. Le 2ème prévoit la nullité de plein droit des actes de spoliation en fin de 3ème article crée une procédure spécifique de restitution qui garantit les délais raccourcis des critères clairs pour les demandes en simplifiant les procédures nous guideront c'est bien vers leurs propriétaires légitimes la restitution n'est pas un simple acte de justice mais une réparation. Une réconciliation. C'est la reconnaissance de la valeur inestimable de c'est bien pour la mémoire collective et pour les générations futures. Nous ne pouvons changer le passé mais nous pouvons agir corriger les torts commis et tisser un avenir de justice et de solidarité. C'est notre devoir envers ceux. Qui ont été dépouillés envers notre histoire et envers nous-mêmes la restitution des biens spoliés aux juifs est une étape cruciale vers la réconciliation. C'est un pas en avant vers la construction d'un avenir. Où le passé n'est pas oublié ou les erreurs sont rectifier. C'est notre devoir de mémoire. Avant de conclure mon propos je souhaite saluer le travail de plusieurs personnes. Tout d'abord celui de la sénatrice Corinne Bouchoux c'est qui a été cité tout à l'heure et qui avait rédigé un important rapport sur ces questions de restitution pluie le travail acharné de notre collègue Catherine Morin- Desailly qui depuis des années, fait avancer cette question des biens spoliés. Notre collègue Béatrice Gosselin rapporteur avec qui j'ai participé à de très nombreuses intéressante audition. Et ce qui est secondé par Aurore. Qui a apporté sa précieuse aide administrative et technique enfin Madame la Ministre merci de vous être saisi de cet. Important sujet des restitutions dans ce projet de loi concerne aujourd'hui les biens spoliés demain seront concernés les restes humains. Et dans un avenir que j'espère proche la restitution des biens mal acquis, projet qui que j'aurais plaisir à pouvoir y travailler sur le fond. Mes chers collègues. Le groupe socialiste, écologiste et républicain soutiendra ce projet de loi visant à simplifier la restitution des biens spoliés ensemble oeuvrons pour réparer des injustices. Pour que les trésors volés retrouvent leur place légitime et pour que la mémoire des victimes soient honorées. Le temps est venu d'agir de rendre justice à ceux qui ont été privés de tout. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent au sénateur Pierre Ouzoulias du groupe communiste pour cinq minutes, chers collègues.

Le texte que nous examinons ce jour est le 1er d'une série de 3 lois destiné à donner un cadre à des restitutions qui n'exigeront plus le vote par le parlement de dispositifs législatifs ad hoc. Un débat préalable aurait peut-être été utile pour dégager les principes du dessaisissement du Parlement par lui même. Car il faut le rappeler, le domaine public mobilier et doublement protégés au titre du code général de la propriété des personnes publiques et du code du patrimoine. C'est pour cette raison que le gouvernement lors du dépôt de la loi de restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal, en juillet 2020. N'avait pas souhaité mettre en oeuvre une loi de principe, selon lui, elle aurait pu être censuré pour l'incompétence négative du législateur et ont été, je cite, un obstacle pour effectuer des restitutions pourtant souhaitable. Le gouvernement a finalement considéré que ce risque juridique dirimant pouvait être contourné par le dépôt de trois lois. Il serait de bonne politique qu'elles obéissent à des objectifs similaires. Le 1er serait celui de la collégialité et de la publicité de l'instruction des restitutions. En l'occurrence, elles sont assurées par la collaboration d'une mission de recherche chargée du récolement des Oeuvres et de la constitution des dossiers, scientifiques et d'une commission administrative En second lieu, il resterait à définir les modalités de l'information du Parlement qui ne peut être totalement exclu de procédure qui touche à la à la domanialité publique le décret d'organisation de la commission placée auprès du Premier ministre répondra sans doute à cette attente. Sur ces 2 points. Je vous le dis sans détour Madame la Ministre le rapport rendu par Monsieur Martinez c'est décevant. La constitution au cas par cas de groupes de travail formé d'experts bilatéraux nommés par leur gouvernement ne peut apporter les mêmes garanties d'impartialité qu'une commission indépendante et pérenne. Par ailleurs, je doute que le Parlement se satisfasse de l'information annuelle donnée par le gouvernement à la seule commission de la culture, lors des débats à venir. Il conviendra donc de nous demander si les attributions de la commission, instituée par le présent projet ne pourrait être pas étendu à d'autres objets. Les conditions de restitution doivent être d'autant plus irréprochables qu'elle concerne des biens qui ont été collectées durant les périodes les plus sombres de notre histoire nationale et qui constitue largement au-delà de leur qualité artistique des témoignages bouleversants du destin dramatique de personnes auxquelles elles ont été arrachés par la violence par la spoliation institutionnelles et par le Dol. Ainsi le texte dont nous débattons n'est pas seulement technique. Il porte pour la première fois depuis 1945 une reconnaissance législative des spoliations antisémites perpétrés par l'Allemagne nazie et aussi l'État français. La voie a été ouverte par le président Jacques Chirac le 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv. J'en rappelle les termes. Je le cite la France patrie des lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole. Elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Prétend entrant après cette déclaration, nous allons chers collègues poursuivent cet effort en identifiant clairement dans la loi la responsabilité spécifique de l'État français. Sauf à engager une coupable opération négationniste. Il est en effet acquis que l'État français a mis en oeuvre de son propre chef, et avec l'aide de l'occupant nazi. Une entreprise de persécution de spoliation des juifs de France citoyens français. Ou des juifs immigrés dans notre pays dont le but ultime fut leur déportation et leur extermination. Cette politique antisémite est au coeur de la révolution nationale voulue par Pétain. Elle fonde le programme de l'extrême droite française depuis Morasse et depuis l'Action française, dont 2000 de ces nostalgiques ont défilé avec les mêmes cris de haine que les ligue factieuse de 1934. Le week-end dernier. Ces crimes antisémites sont des crimes contre l'humanité. Ils sont imprescriptibles. En votant cette loi nous affirmons solennellement la volonté de la nation devrait perpétuellement pour les identifier les dénoncer et aussi en tenter une compensation matérielle. Par la restitution. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure et monsieur le président de la commission et chers collègues. À mon tour je ne peux que saluer le présent texte au nom du groupe l'Union centriste et féliciter notre rapporteur Béatrice Gosselin, qui a effectué dessus un travail remarquable. Comme cela a été signalé à plusieurs reprises en commission le Sénat peut s'enorgueillir d'avoir été moteur en la matière. Le Sénat il vous me permettrez, mes chers collègues, ce petit mot d'autosatisfaction en particulier le groupe d'union centriste puisqu'on ne voit Nicolas bout le 1er texte de loi de restitution de restes humains. À savoir la loi du 6 mars 2002. Restituant la fameuse Vénus hottentote, à l'Afrique du Sud. S'inscrivant dans la lignée Catherine Morin-de la saillie a été à l'origine de la loi du 18 mai 2010, visant à autoriser de la restitution par la France des têtes maories, à la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne plus précisément les restitutions de biens culturels ayant fait l'objet de spoliation de nature antisémite dans le contexte du nazisme Corinne Bouchoux, cela a été dit avait initié le débat en 2013. Nous sommes en 2023. Il aura fallu 10 ans pour qu'un gouvernement se saisisse pleinement du sujet. Pourquoi avoir tant attendu s'interrogeront les esprits les plus critiques. Mieux vaut tard diront les autres. Certes il y a bien eu la loi du 21 février 2022 par laquelle la France a restitué 14 Oeuvres de collections nationales et une oeuvre de collections municipales spoliés ou acquise dans des conditions troubles. Grâce à cette loi. Les Oeuvres en question ne s'était rendu au disait en droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites. Mais pour vraiment procéder à un inventaire global et menée en fait une véritable politique de restitution et de réparation, les lois d'espèces ne suffisent plus. On le sait depuis longtemps un cadre global s'impose. C'est justement ce que propose le présent texte nous ne pouvons que nous en féliciter d'autant plus que le dispositif qu'il met en oeuvre et pertinent. Je ne reviendrai pas longtemps longuement dessus. Il permet aux détenteurs des biens restitués d'avoir l'initiative de la restitution alors que jusque-là une telle restitution ne pouvait avoir lieu que sur l'initiative des ayants droit. Il soumis à la sortie des collections à l'avis préalable de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations si vs. Nous souscrivons l'analyse de notre rapporteur selon laquelle le caractère simples de la vie ne vide pas ipso facto le dispositif de sa substance. On peut imaginer que la plupart du temps la vie d'assez IVS sera suivie. Mais dans la suite de nos travaux, il nous faudra tout de même trancher la question de savoir ce qui se passera. Lorsqu'il ne le sera pas. En fait nous sommes satisfaits de la flexibilité du texte. Il permet en effet que les différentes options pour compenser la spoliation. Autre que la restitution pure et simple puisse être discuté entre la collectivité et la personne qui a été spolié ou ses héritiers. Si par rapport aux lois d'espèces cadre général, il n'en demeure pas moins spécifiquement établi pour les spoliations antisémites. Fallait-il un cadre plus global qui englobe toutes les restitutions. Notre 1er mouvement allait plutôt dans ce sens. La proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques que le Sénat a adopté le 10 janvier 2022 ne portait pas sur les spoliations antisémites mais regrouper les Christine Futian coloniale et restitution de restes humains. C'est un autre choix, qui avait finalement été fait par le gouvernement. Le président, projet de loi et le 1er d'un train de 3 textes qui nous seront successivement présenté celui-ci donc pour les spoliations antisémites. Une nouvelle proposition de loi de Catherine Morin-Desailly sur la restitution des restes d'humains et un projet de loi consacré aux restitutions coloniale. Pourquoi pas. Nous comprenons l'intérêt mémoriel et politique de ce choix. Il s'agit d'éviter tout amalgame et de rendre son importance et sa singularité à chacune des situations. Néanmoins, il serait bon que les excellents principes qui irriguent le texte qui nous est aujourd'hui soumis imprègne aussi les 2 autres, ce à quoi le groupe de l'Union centriste sera vigilant. Pour autant, vous l'aurez bien compris mes chers collègues, que nous voterons favorablement ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole. À présent à notre collègue monsieur le sénateur. Bernard Fiolet du groupe RDSE. Et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure et monsieur le président de la commission et chers collègues. C'est toujours avec une émotion certaine que nous nous retournons vers cette sombre période de notre histoire qui a vu l'idéologie nazi organisé l'extermination du peuple juif et la spoliation, c'est bien. La complicité de l'État français de l'époque nous oblige encore davantage envers les victimes et leurs descendants. Le projet de loi sur la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés entre 1933 et 1945. Est attendu et mérite notre soutien. il permet de revenir sur l'inaliénabilité de biens culturels du domaine public afin de les restituer au même titre que les biens MNR. Profitons Madame la Ministre de cette occasion pour nous interroger sur une évolution possible des principes d'imprescriptibilité et Dean Eliane débilité des biens culturels. Cette inaliénabilité pourrait reposer sur la seule dimension culturelle plutôt que sur la patrimonialité. L'inscription des biens culturels dans un Patrimoine mondial de l'humanité serait en remarquable message de Concorde universelle. Elle permettrait à l'art à la culture de jouer pleinement son rôle d'éveil de conscience. Le débat reposera alors sur l'usufruit la nue-propriété ainsi que sur la localisation des Oeuvres, des Oeuvres d'art dans les musées pour un dialogue interculturel et intergénérationnel. Ou sur leur lieu d'origine. Si elles sont nécessaires à l'identité d'un territoire ou d'un peuple. Si notre émotion est forte en revenant sur les spoliations antisémites. Cette reconnaissance et six réparations. Doivent s'intégrer dans un plus vaste de voir de reconnaissance et de réparation des autres spoliation réalisées à d'autres époques dans d'autres lieux, je pense aux spoliations de l'époque coloniale. Au cours des auditions. Nous avons été alertés sur le risque de ressentiment qu'une loi spécifique aux spoliations antisémites pourrait alimenter si nous négligeons concomitamment d'autres spoliation, celle de la période coloniale, comme je l'ai dit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et nous devons aux victimes des persécutions antisémites et à leurs descendants de ne pas risquer de voir la porte de cet enfer. Une loi cadre qui rassemblerait toutes les spoliations ne stigmatiserait personne et élèverait la France au dessus de contraintes administratives qui serait suspecte. Au regard de notre devoir de reconnaissance et de réparation des préjudices subis. Alors nous accueillons positivement les évolutions de ce que, de ce projet de loi. Ce qu'il apporte aux démarches légales de reconnaissance et de restitution. Si l'obtention automatique du certificat d'exportation pour les Oeuvres spoliées importer sur notre territoire est une juste réparation. Nous pouvons nous interroger sur cette automaticité. Pour les Oeuvres qui ont toujours été sur notre territoire. Sachant qu'elles en sortirait si les négociations n'aboutissaient pas puisque l'autorisation sortie s'imposerait à l'heure. Et plutôt qu'une présence symbolique de parlementaires. Dans une c'est IBS reconfiguré un véritables rapport annuel d'information des commissions culture du Parlement nous apparaît indispensable dès que le Parlement sera dessaisi de la vie dont le privera l'adoption de cette loi. Nous souhaitons enfin Madame la Ministre que les moyens de recherche de provenance soit réellement assurés. Le devoir de réparation. Nous y oblige. Merci, cher collègue, la parole est à présent au président Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains. Et vous avez minutes chers collègues. Madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure. Qui sommes-nous. Juste des parlementaires. Juste des parlementaires. Pas plus pas moins. Alors j'entends beaucoup de choses et je voterai le texte Madame la Ministre. Pas d'inquiétude. Mais. Je dois dire que dans cet hémicycle. Je préférerais ne pas entendre dire qu'un texte. Peut être une réparation. Une réconciliation. Comme je l'ai entendu tout à l'heure. La Shoah ne se répare pas. Ne se réconcilient pas. Ne. N'est pas du même domaine que le reste. Ce texte va permettre. De faire en sorte qu'il n'y ait plus de loi spécifique. Chaque fois qu'on veut restituer. Mais restituer. On dit en France sans parler du reste de l'Europe entre 100.000 et 150.000 biens spoliés. Spoliés. Bien sûr il y avait les trains Goering. Bien sûr il y avait le monument de Linz d'Hitler. Bien sûr il y avait ces Oeuvres d'art magnifiques. Qui était saisis chez les collectionneurs ou chez des galeristes. Mais c'était pour beaucoup des Oeuvres d'art qui n'était pas forcément d'un niveau mondial. C'est là où sont-elles. Dans un certain nombre de nos musées. Mais pour beaucoup, elles ont atterri. Chez les collaborateurs chez les profiteurs de guerre chez des gens qui sans scrupules. Ont utilisé le régime nazi. La collaboration. Le régime de Vichy. Pour s'emparer des biens. Et là-dessus. Où en sommes-nous. Bof c'est tellement difficile. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de restitution juste après la guerre. la le retour si je puis dire. Après la Libération. L'occupation de l'Allemagne et le fait que naturellement on est restitué un certains nombres de bien connu, reconnu. Pour beaucoup. C'est l'administration allemande très clairement enregistré

Alors il faut naturellement Madame la Ministre trouver un texte qui permettent pour ceux au moins qui sont dans les musées. Pour ceux au moins qui sont apparemment dans les collections publiques un retour. Mais regardez je je regardais l'autre jour ce collectionneur viennois. Qui sans rien dire. Sans vous informer une quelconque autorité avait chez lui, chez lui des centaines de tableaux spoliés volés et qu'on a retrouvés pas par hasard mais certainement pas parce que lui-même l'a dit Moi je je pense qu'il faut avancer. En vous remerciant Madame la Ministre comme je remercie d'ailleurs le rapport de Madame Bouchoux comme les travaux de nos collègues centristes. Mais en étant extraordinairement modestes. Parce qu'en vrai. Au-delà de ce que je disais on ne répare pas à la Shoah. On ne. Réconcilie pas moi je considère que la restitution des biens. Franchement, ça n'est en rien il leur réconciliation des Français parce qu'il y a pas de réconciliation à avoir par rapport à ces événements. Et je n'accepterai pas l'idée même qu'il puisse y avoir une réconciliation, ce serait la négation de la République la négation de la République rendre un tableau. Ça n'est pas de la réparation, c'est la justice. C'est la justice et seulement de la justice parce qu'un tableau qui appartient à une famille qui a été spolié appartient à cette famille. Donc la justice nécessite qu'on lui restitue le tableau, on ne répare pas en revanche malheureusement on ne peut pas on ne répare pas le fait que les parents de cette famille a été déporté massacré. Comment voulez-vous réparer ça ça ne se répare pas. Donc moi je. Je considère que la restitution était un acte de justice, ça n'est pas un acte de réparation. Ni de réconciliation et il faut être très clair de là-dessus. Madame la Ministre le vrai sujet. Je rentre pas dans, dans les débats et je remercie la commission des travaux qui ont été faits sur. L'analyse le le le suivi la possibilité de de d'accélérer un peu. Le système de restitution. Mais le vrai. Travail est-il faisable humainement faisable. Le vrai travail serait déjà de dire comment encourager j'utilise un terme Poli. Les musées privés ou publics. Les collectionneurs privés ou publics. Qui ont un doute. Sur l'origine du bien. De faire en sorte de se tourner vers les commissions pour analyser réellement l'origine du bien. Je reconnais les choses. Vous êtes. Le conservateur d'un musée privé. Vous avez un bien. N'avait pas tellement envie d'avoir à le restituer. Donc on sent bien que c'est une activité publique de d'enquête pour savoir où est-ce bien. Et c'est ça la difficulté c'est que. Par définition, c'est long. Il y a beaucoup de bien, qui pour le moment ne sont jamais revenus dans les familles il y a beaucoup de familles qui n'ont plus d'héritiers. Parce qu'ils sont tous morts. Et ces familles-là. Qu'est-ce que vous voulez faire les biens ne seront jamais par définition restituer et je le dis très tranquillement. Madame la ministre. Oui, il faut des textes, il en faudra d'autres sûrement et on peut avancer. Mais ne parlons pas de réparation. Ne parlons pas de réconciliation. La Shoah et ce qu'elle a été elle est irréductible à une réparation avançons restituant rendons la justice mais n'oublions pas. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein. Nathalie Goulet, sénatrice du groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure, monsieur le président de. De la commission des affaires culturelles, pas très facile de prendre la parole après Roger Karoutchi. Tout a été dit ou presque sur ce projet de loi qui comporte à mes yeux, madame la ministre, une erreur historique majeure.

Madame la Ministre, ce n'est pas le se disant ans gouvernement. Qui a expulsé mon père du lycée Charlemagne. Ce n'est pas se, se disant gendarmes qui ont raflé mon père et ses parents le 16 juillet 42. Ce n'est pas le se disant commissaire priseur sur ordre du préfet du Nord, Monsieur le Sénateur. Qui a spolié ma grand-mère et son mari de quelques bien qu'il possédait dans un petit magasin de chapeaux à Douai. D'ailleurs Madame la Ministre voilà la liste des spoliations. Il y a pas que des Oeuvres d'art, il y a le 24 août 42 dans un tout petit magasin de Douai des pieds des rayonnages pour 350 francs. Une caisse et quelques éléments pour 11.160 francs de l'époque. Mon grand-père maternel dit ne s'est pas laissé faire. L'histoire est un peu long pour aujourd'hui mais. C'est bien au préfet du Nord qui l'a écrit parce qu'il avait un problème sur les biens. toujours aussi modeste indiquant vous voudrez bien me faire parvenir toute communication ou instruction une nouvelle adressé par le Commissariat général à Paris relatives à cette affaire, c'est une la lettre du 25 juin 42 que ma mère a gardé précieusement. C'est l'État français comme l'a reconnu, le président Chirac dans un discours historique irresponsable, j'ai déposé des amendements. Dans ce sens dans cette période troublée. Madame la ministre, il faut appeler les choses par leur nom de façon à éviter les amalgames et le négationnisme. Il faut aussi éviter que certains candidats aux élections présidentielles puisse affirmer que Vichy a protégé les juifs les spoliations c'est un vol une injustice commise par l'État français, saisi l'autre les spoliations. C'est une blessure due à cette injustice que le temps n'efface pas. Et qui se transmet de génération en génération. Je veux rappeler ici la mémoire des milliers de familles spoliées de quelques biens meubles, linge de maison, quelques instruments de cuisine. Aussi de toute leur vie, évidemment. Hier il y avait sur France 5. Hasard de la programmation, un documentaire remarquable sur l'opération meubles 44.000 foyers juif. de la, du, du sol au plafond avec de la lingerie, des jouets, des des petites cuillères, madame la Ministre, il faudrait lancer un appel à tous ceux et toutes celles qui pourraient être en possession de documents tels que ceux que j'ai entre les mains pour poursuivre le travail déjà accompli. Le texte que nous allons voter aujourd'hui est un texte mémoriels, qu'il s'appelle ainsi qui ne se l'appelle pas. C'est un texte pour la mémoire et Roger Karoutchi l'a très bien dit, comme je l'ai dit à votre prédécesseur. Madame la ministre vous n'êtes pas aujourd'hui seulement le ministre de la culture, vous êtes aussi celui de la justice. Merci cher collègue. La parole. État présent à Madame Else Joseph du groupe Les Républicains. Pour cette Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Ce texte n'est pas seulement un dispositif qui vise à faciliter la restitution de biens à leurs propriétaires à ne plus pourrait-on dire. Dans un long débat qui touche l'origine de certaines collections des musées européens. Eh bien non, il s'agit de bien plus que de restitution patrimonial. C'est une démarche qui s'inscrit dans la condamnation constante des persécutions antisémites de la 2ème guerre mondiale depuis le général de Gaulle dès 1940 d'un refus de cette injustice profonde. Qui a déshonoré la France et la République au plus profond d'elles-mêmes d'une condamnation enfin de cette barbarie son nom qui a commis des crimes sur des individus dont le seul tort était celui détenait comme le disait si justement André Frossard quand il parlait du Crime contre l'humanité. Ce projet de loi à l'initiative du gouvernement vise à restituer les biens culturels qui ont fait l'objet de spoliation. Dans ce contexte de persécutions antisémites entre 1933 et 1945 sur le sol français. Des biens qui appartiennent à des collections publiques des biens qui n'aurait jamais dû s'y trouver. On peut même s'étonner qu'au regard de cette injustice si profonde, cette restitution n'ait pas été facilitée dès l'origine et que la demande de restitution était été laissée à l'initiative des propriétaires spoliés ou de leurs ayants droit. Comme toute démarche une telle demande peut s'enliser dans les méandres de procédure longue que les familles n'ont pas la force de supporter. Pourtant la spoliation est une négation honteuse du droit de propriété qui profondément ancré dans notre droit ne peut être mis en cause que pour des raisons d'intérêt général. Là elle n'en est pas une. Cette spoliation et pour les familles, la négation de leur humanité, de leur mémoire et de leurs souvenirs et ce texte doit être donc salué pour ses apports, ce texte est attendue par ces familles. Tout d'abord il l'institut une procédure de restitution simplifiée des biens culturels spoliés à l'initiative des personnes publiques cela facilitera les restitutions en rappelant que l'État, les administrations ont aussi des devoirs. C'est donc du côté de la puissance publique que la démarche de restitution doit d'abord être engagée alors même que les autorités françaises ont reconnu leur responsabilité dans les persécutions, comme l'avait fait Jacques Chirac en 1995. Dans son discours du Vel d'Hiv'et il a été cité tout à l'heure par notre collègue Pierre Ouzoulias. La période est défini. Plus largement, ce qui permettra de viser toutes les spoliations de caractère antisémite et évitera de buter sur des problèmes de chronologies. Les persécutions antisémites, n'ont pas commencé avec Vichy mais Vichy il y a bien participé et cela bien au-delà du territoire français. Cela permettra évidemment de restituer les biens confisqués par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, comme le prévoit le nouvel article L 115 2 du code du patrimoine. C'est bien, qui sont considérables et ça a été évoqué. Par tous les intervenants à plusieurs reprises avec des chiffres qui donnent le tournis. Plus de 5 millions £ 100.000 Oeuvres spoliées en France pendant l'occupation, dont seulement 45.000 ont été restitués après guerre et de 1200 d'entre elles font partie des collections des musées nationaux des chiffres. Vraisemblablement sous-estimées. Certes le temps peut faire son oeuvre et les propriétaires spoliés ou le rayon droit peuvent demander autre chose qu'une restitution. Le texte prévoit ainsi une alternative à cette restitution par un commun accord entre la personne publique selon des modalités de réparation de la restitution autre que la restitution du bien mais. La souplesse ne doit pas être entendu comme un abandon de restitution, même s'il faut saluer la possibilité de transactions. Il faudra aider au maximum les propriétaires ou leurs ayants droit. Ce sujet sera suivi cette restitution peut aussi être engagé par les personnes morales de droit privé qui détiennent des biens spoliés. Le texte précise ainsi qu'il s'agit des collections des musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé. C'est également une avancée car elle soulève la problématique des musées privés. Le mouvement des réparations de ces dernières années est en route, marque une avancée et un encouragement à poursuivre avec le avec le sort des autres M, N et R toujours en attente de restitution. Enfin un texte si important ne saurait éluder la question de son application et les démarches qui vont être entreprises. Madame la Ministre quelles initiatives seront prises dans les mois à venir. Certaines personnes publiques sont sous la tutelle de votre ministère. Quels établissements au musée par exemple pourraient être concernés. Comment seront-ils aider financièrement car si les indemnisations était envisagé cela soulèverait des problèmes de financement. Il faudra être vigilant sur le décret qui fixera les modalités d'application de la nouvelle section introduit dans le code du patrimoine pour cette procédure de restitution simplifié. Ce texte va déterminer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission administrative qui donnera un avis à la personne publique effectuera la restitution. Il concernera également des modalités d'application relative aux restitutions qui seront effectués par des musées privés. Salue cette précision apportée en commission par un amendement donc de ma collègue rapporteure Béatrice Gosselin. Sans préjuger de la rédaction de ce décret il convient d'avoir des garanties et un suivi de sur son n'élaboration sera-t-il possible d'être informé. La commission de la culture. Il sera vigilante. Enfin il faudra préciser l'ampleur des restitutions pour avoir une vue globale de plus une vue globale pardon de ce qui nous attend. Madame la Ministre Madame la rapporteure, chers collègues, je voterai avec mon groupe ce texte parce qu'il constitue une démarche dans une France que nous voulons plus juste, qui ne s'abrite pas derrière la complexité du passé pour mieux fouler les droits les plus fondamentaux de l'homme. Ce texte traduit une volonté politique à travers l'émotion suicidé et formule un voeu que ce texte puisse inspirer d'autres pays, d'autres États confrontés au problème des spoliations. Un pays qui reconnaît ses fautes peux toujours rester un modèle dans le monde au maire.

L'amendement numéro 18 présentée par notre collègue Madame Nathalie Goulet. Madame la présidente, madame la ministre, en réalité sur. Les crimes. Commis par l'État français dans la période concernée. il n'existe absolument aucun texte reconnaissant et je pensais que ce texte c'était peut-être l'occasion de pouvoir être complétée. De façon à ce que la nation reconnaisse sa responsabilité à l'égard des des populations juives dans les agissements de l'État français de 1940 à 1944 c'était un amendement. Peut être mémoriel mais c'est un c'est un sujet extrêmement important et ce texte pourrait peut-être. Permettre de le porter. Merci madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. Si la responsabilité propres du régime de Vichy dans les persécutions antisémites est indéniable. L'objet du projet de loi n'est pas. Il vise à créer une procédure de restitution de justice des biens culturels spoliés par ailleurs le Champ de l'amendement et du projet de loi ne coïncide pas le projet de loi couvre un Champ plus étroit que l'amendement proposé puisqu'ils ne portent que sur les spoliations des biens culturels et en même temps son périmètre spatio-temporel et plus étendu puisqu'il couvre toutes les spoliations de biens culturels intervenu entre 33 et 45, quel qu'en soit l'auteur ou le lieu de perpétration.

Oui j'allais proposer un retrait puisque effectivement on ne serait pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu le discours du Vel d'Hiv'de Jacques Chirac, c'est évident, c'est très important de le rappeler. Ce projet de loi n'aurait pas été possible sans ce discours, mais son objectif est différent puisque là en fait c'est à la fois plus restreint et plus vaste, comme vient de l'expliquer la rapporteure le la loi porte sur la sortie du domaine public de biens culturels spoliés, c'est-à-dire donc sur un champ nettement plus étroit que celui de toutes les persécutions commises par le régime de Vichy et à l'inverse, le projet de loi porte sur un Champ géographique et temporelle finalement plus vaste que celui couvert par le régime de Vichy, puisqu'il s'agit de pouvoir faire sortir du domaine public des biens spoliés en Allemagne et ailleurs en Europe par l'Allemagne nazie et divers spoliateur et dès 1933 pour ce qui concerne l'Allemagne. Donc voilà on n'est pas complètement raccord mais ça n'enlève rien au fond de ce que vous avez dit et, à savoir l'importance de ce discours fondateur. Je vous remercie. Monsieur le Président, carottes, explications de vote. Le président ma liste moi je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'amendement correspond à l'ampleur du texte. Je demande à ma collègue de retirer l'amendement. Ça n'est pas la nation qui est en cause. C'est le régime de l'état français de Vichy dans la nation. Il y avait des résistants. Il y avait des juste il y avait des gens qui en aucun cas n'aurait accepté ce qui s'est passé et la nation d'aujourd'hui n'a pas à. Assumer la responsabilité de la Nation d'hier qui en elle même était diverse que la République. Confondent le régime de l'état français. Oui parce que le régime de l'état français était collaborationniste. Mais c'est la République qui dit l'État français était collaborationniste et a permis les les spoliations et la déportation. Mais c'est pas la nation, la nation, c'est un ensemble tellement plus vaste tellement différent du régime politique et moi je, je ne veux pas qu'on dise la nation parce que je n'accepte pas et c'est pas du tout le sens évidemment de l'amendement de Nathalie Goulet, mais ça pourrait prêter à confusion des résistants

Merci. Nous passons aux amendements de l'article 1er, la parole est à monsieur Le Marc Laménie. Portée par votre ministère, madame la Ministre et puis aussi celui le travail. Sous couvert de monsieur le président de la commission. Culture, éducation, communication le. Le travail de Madame le rapporteur et tous les collègues qui sont intervenus sur un sujet. Historique est particulièrement sensible. Alors concernant cet article 1 qui vise la création d'une procédure administrative pour la restitution des biens culturels spoliés intégré aux collections publiques et vous avez cité aussi le rôle important de la C. Ivest. Alors je ferai référence puisque les commissions travaillent aussi ensemble. On avait présenté le 6 juin 2018 en commission des finances dans le cadre de la mission. Anciens combattants. Il y a avec la nation et et mémoire, un travail important, bon puis sur le rapport d'information il fait pas loin de 200 pages. Concernant la CIV commission d'indemnisation des victimes de la spoliation antisémite. Le titre 20 ans après. Redonner un élan à la politique de réparation et Constat mais aussi de recommandations en rappelant aussi le le rôle important, vous avez fait référence aussi. Au au président Jacques Chirac et puis aussi toutes les personnes qui se sont investis. Et engagés Et puis dans les recommandations de la commission des finances. On avait aussi pour une CV c'est Ivest augmenter. Je crois que c'est aussi permettre de donner des moyens de réparation dans le cas de la notion de de respect et, de mémoire, surtout pour les descendants les ayants droit donc voilà donc je je soutiendrais naturellement cet article et vous en remercie. L'amendement numéro 4 présenté par Monsieur Ouzoulias. Merci madame la présidente madame la miss mais mes chers collègues. Mon amendement porte sur. L'article 1 et la phrase que je je vous répète parce qu'elle a son importance dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés par l'Allemagne nazie et par les autorités Touaregs Edouard qu'elle a occupées contrôler ou influencer notamment l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français. Je je pense que l'adverbe notamment peut être ambigu et pourrait laisser entendre que l'État français a organisé la spoliation des juifs sous la pression de l'occupant nazi, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. L'analyse historique a a bien montré que. Le le le gouvernement de Vichy avait organisé lui-même sans contrainte. Une partie de la persécution. Je vais, je vais vous citer juste un témoignage historique c'est celui du du directeur de cabinet de de Pétain Henri du Moulin de la barre tête dans ses mémoires en 1946 qui dit, je le cite. L'Allemagne ne fut pas à l'origine de la législation anti-juives de Vichy cette législation fut si l'on peut dire spontanée et et autochtones. Je propose de remplacer le notamment par et pour bien identifier la spécificité des lois votées par l'État français. Je vous remercie madame la présidente. Je vous en prie madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. Oui, cette question avait déjà été très débattu lors de l'examen du projet de loi en commission et monsieur Julia. Mon collègue il nous avait promis de revenir sur sa rédaction qui n'aurait pas d'incidence sur le périmètre des spoliations couverte par le texte, même si on peut s'interroger sur le bien-fondé du distinguer le régime de Vichy. D'autres territoires occupés contrôlées ou influencées

propose un avis favorable. évidemment notre intention était absolument pas de minorer l'action du régime de Vichy. Donc, avis favorable du gouvernement. je voudrais remercier Pierre Ouzoulias. Pour cet amendement. J'aurais peut-être des amendements à faire mais on en discute renter la tête sur son nette avance au tout à l'heure. Quand la responsabilité des antisémitisme dans notre pays. Peut-être était plus large qu'il a pu la présenter tout à l'heure mais nous parlerons de cela en dehors de l'hémicycle. En revanche je voudrais. Le remercier Pierre Ouzoulias. Et Patrice Gosselin du travail qui a eu lieu entre notre commission et cette séance pour arriver à une écriture qui me semble en effet tout à fait dans le droit fil du discours du Vel d'Hiv'de Jacques Chirac mais je suis bien d'accord avec vous Madame la Ministre, le gouvernement n'avait certainement pas l'intention. De, de revenir sur cette ligne qui êtes totalement fixé et qui précise clairement. Que la politique antisémite de Vichy.

les désirs de l'occupant. Ce qui est précisé clairement par ce épars qu'porte aujourd'hui Pierre Ouzoulias à la réception de votre texte Madame la Ministre donc je suis très heureux que nous arrivions, assez d'accord après cet échange entre la Commission et Pierre Ouzoulias.

Mais je voudrais pas qu'on ait une vision réductrice du discours de Jacques Chirac qui disait ça. Mais qui venait interrompre. Une grande période. C'est pour répondre à monsieur Karoutchi. Parce que je partage que moyennement. Ce qu'il a dit qu'il venait interrompre une grande période où justement. La France. Disait qu'elle ne voulait pas s'excuser pour les crimes d'un État qui n'était pas en représentant de la nation, ni de l'État feront de de la République. Et on disait pourquoi la république va c'est excusez-pour ce qu'elle n'a pas fait, souvenez-vous, ça a été ça

amendement de monsieur Ouzoulias. Mais je voulais quand même expliquer que ce n'est pas que cela. Qu'a fait Jacques Chirac de dire clairement, le gouvernement de Vichy. Il a aussi dit que on ne peut pas s'exonérer des moments sombres de notre histoire et donc je veux par là même. Saluer encore plus ceux qui se réclament du chiraquisme de ce qu'a fait Jacques Chirac. Alors si je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis favorable qui vote pour.

Il s'agit de remplacer le gouvernement se disant gouvernement de l'État français par l'État français, c'est exactement ce que vient de dire notre collègue et qui correspond au discours de Jacques Chirac, il reconnaît la responsabilité de la France. Dans dans la déportation des juifs de France. Madame la rapporteure votre avis. Alors notre souci n'est pas de minimiser la responsabilité de l'État français, on en a déjà parlé tout à l'heure dans les dans son travail dans son

portant 2ème, application de l'ordonnance du 12 novembre 43 sur la nullité des actes de spoliation accompli par par l'ennemi, c'est la raison pour laquelle le gouvernement là sans doute retenu dans la mesure où il s'agissait d'un du seul texte déjà en vigueur applicable aux spoliations antisémites. Il y a intérêt à créer une continuité entre le présent projet de loi et cette ordonnance dans la mesure où c'est sur son fondement qu'un juge peut aujourd'hui annuler l'entrée dans les collections publiques d'un bien culturel et ordonné sa restitution,

Merci madame la présidente. Les explications de la rapporteure sont limpides, ce que nous avons eu beaucoup d'échanges avec le Conseil d'État avant de vous proposer le texte et c'est exactement pour ces raisons que nous avons retenu cette formulation. Donc je me joins à la demande de retrait. Merci. Monsieur Ouzoulias pour. Explications de vote. Merci madame présidente Madame la Ministre j'ai un doute, j'ai un doute sur cet amendement parce que lorsque. Le. Le général de Gaulle signe l'ordonnance de 1945. Il veut montrer par cette formule, se disant gouvernement de de l'État français. Que. La République était à Londres. Et que l'État français était à Vichy. Et que la République avait continué de vivre à l'extérieur sous la forme. Prise ensuite par un gouvernement provisoire et qu'en aucun cas elle pouvait être confondu avec l'État français qui étaient. qu'il avait sombré dans dans la collaboration. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Je pense que cette formule, se disant gouvernementale. De gouvernement de l'État français pour avoir un sens en 1945, je suis pas sûr qu'elle ait le même sens aujourd'hui en 2023 et peut être qu'une formule plus courte en effet où on parlerait simplement du gouvernement de l'État français pourrait être justifiée. Mais encore une fois j'ai j'ai un doute et j'exprime publiquement mon doute sur sur cet amendement merci président. Merci. Le président Karoutchi pour explication de vote. Moi je trouve que les 2 rédactions sont pas terribles. Parce que. Se disant gouvernement de l'État français. Ça ne veut pas dire grand chose. Soyons franc. Dans l'ordonnance bien sûr juste après la guerre on dit bah comme l'a dit excellemment Ouzoulias. La République la légitimité elle était à Londres la légalité. Je sais pas mais la légitimité elle était à Londres. Moi je préférerais quelque chose à leur dire que l'État français. Ça peut prêter à confusion parce qu'aujourd'hui quand vous dites l'État français. On, on imagine que vous parlez bat de l'État tout court de l'état actuel, pas plus de l'État français que de Vichy que ou alors il faudra mettre l'État français du site qui ne signifie ni rien. La rédaction possible serait de dire, le régime de l'état français parce que là, par définition, on sait très bien ce que c'est, c'est pas l'état français d'aujourd'hui, c'est le régime de l'état français des années 40 44, le soi-disant ça a un côté un peu. En vrai il n'avait pas le pouvoir. Ben si il avait le pouvoir. Il y avait un gouvernement. Légal, même s'il était illégitime, mais légal. Malheureusement dans des conditions que l'on sait, le Parlement l'avait. Mis en place donc je pense que le régime de l'état français permettrait de sortir de l'ordonnance et permettrait d'éviter de dire que l'État français si Nathalie Goulet, on était d'accord parce que quand on dit seulement l'État français et l'opinion publique aujourd'hui, elle pense à l'État quoi ils pensent pas au régime de Vichy. Monsieur le président. Oui merci d'abord à notre collègue d'avoir soulevé la question elle est complexe et nous aux iront bien à travers vos interventions. Je suis pas totalement à l'aise avec les les les les 2 appellations. Je ne suis pas non plus à l'aise avec celle que vient de. De de d'indiquer le président Karoutchi parce que le régime de l'état français pour moi ne veut pas dire grand chose, c'est le régime de Vichy ou l'État français. Néanmoins je je moi je préconise quand même de rester à la version initiale. Tout simplement parce que nous sommes en train de faire un texte de loi et et ce qui nous préoccupe avant tout même si bien sûr, nous avons cette dimension historique et la précision des des termes qui est extrêmement importante, mais ceux de consolider et d'assurer. La sécurité juridique de notre texte. Et et et le Conseil d'État, c'est bien dans cette optique là. Qu'il a demandé qu'on fasse référence. À l'ordonnance de de de 45 ou ces mots était. Stipulé pour bien faire le lien juridique. Je pense que la prudence reste de de rester plutôt sur cette version même si nous n'en sommes pas totalement satisfait. Merci Madame Goulet pour explication de vote. Oui moi je, je rejoins ce qu'a dit. Pierre Ouzoulias c'est je remercie le président Karoutchi parce que, en réalité, cette expression est totalement connoté. Alors évidemment elle est reprise par le conseil d'état parce que c'est ce qui existe, mais si on rédige un peu mieux alors. Le régime de Vichy par exemple j'avais un amendement que j'ai retiré entre deux parce que j'ai choisi l'État français. Je voulais pas avoir, je trouvais que ça affaiblissait le raisonnement d'avoir un espèce de subsidiaire sur le sujet qui, comme vous l'avez compris me touche personnellement. Comme nous tous d'ailleurs. Ou peut-être un peu plus donc. J'ai pas voulu décliner. Avec les, le, le régime de l'les de de Vichy qui était un amendement que j'avais aussi rédigé qui était un espèce d'amendements de repli. Donc moi je pense que si on rédige quelque chose maintenant, je pense que évidemment ce que propose Roger Karoutchi. Me convient parfaitement. Mais ça peut être le régime de Vichy. Ça, ça correspond aussi en tous les cas ce qui est sûr c'est que le se disant est complètement connoté dans une période qui est extrêmement troublée ou un texte qui va concerner uniquement les spoliations d'Oeuvres d'art de juifs peut poser des d'autres types de problématiques vous connaissait très bien monsieur le Président Madame la Ministre le président que le climat. Extrêmement compliquée dans laquelle. Évolue notre notre société en ce moment moi je, je trouve que le le ce 10 ans n'est absolument pas conforme à l'idée que je me fais d'un texte. Alors il faudra moi je suis tout à fait prête à sous-amendé. C'est pas un très gros sous-amendement et à mon avis, on pourrait travailler sur ce sous-amendement. Alors, de ce que je comprends la commission ne souhaite pas proposer en sous-amendements. Madame la Ministre. Non plus. Donc je, mais je vois cet amendement, vous le conserver en l'état, où vous le retirer.

Le régime de l'état français conformément à ce qu'a proposé très subtilement. C'est le régime le régime de Vichy un avis défavorable de la commission sur cet amendement rectifier défavorable de. La part du gouvernement. Je mets donc aux voix. Cet amendement modifié. Qui remplacent les mots se disant gouvernement de l'État français par les mots le régime de Vichy avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre.

Oui, cet amendement donc revient sur l'automaticité. Des certificats d'exportation des des biens qui sont rendus aux familles. Je voudrais simplement le le il est pas question du tout de, de revenir sur la liberté. Des des familles des ayants droit qui qui peuvent récupérer un bien et qui qui avaient été. Importés de l'étranger ça me paraît en revanche. Je souhaite que les biens qui ont toujours été sur notre territoire, puissent suivre. La même démarche d'interrogation et de sensibilisation pour savoir s'il n'y a pas. Une possibilité de compensations ou de négociations pour que ces biens reste sur. Notre territoire. C'est. Je pense qu'il y a une différence de traitement à avoir sur sur. C'est bien. Les familles spoliées. N'ont pas eu leurs dans leurs possession sur dans un pays étranger c'est bien puisqu'ils n'ont jamais quitté notre territoire et je pense que on doit s'interroger sur. Plus profondément, que de rendre automatiquement cette cette possibilité. Voilà le sens de de cet amendement. Merci cher collègue. Madame la rapporteure votre avis. Oui hier. En adoptant ce terme cet amendement chers collègue. Nous n'apporterions plus qu'une réparation partielle de la spoliation. À la différence des familles spoliées à l'étranger, les ayants droit des familles spoliées en France qui vivrait aujourd'hui à l'étranger pourraient au final se voir refuser les droits de faire revenir chez eux qu'on aura, confie ce qu'on leur avait qu'on leur a restitué donc les modalités doivent être les mêmes pour l'ensemble des personnes, quelle que soit l'endroit où elle habite et que et que soit l'endroit où se trouve l'oeuvre à partir du moment où le projet de loi offrent déjà la possibilité de négocier à l'amiable rachat du bien culturel. Il me semble que nous disposons déjà d'une mesure permettant d'éviter sous réserve de l'accord des propriétaires évidemment la sortie du territoire de biens constituant des trésors nationaux. C'est pourquoi la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Madame la Ministre. Merci madame la présidente. Je suis d'accord avec la rapporteure même avis défavorable. Monsieur le sénateur pour explication de vote. je ne pense pas qu'il y ait de de préjudice. Ici. Pour que ce bien puisse sortir s'il était resté dans la possession des familles. Il faudrait un certificat d'exportation. C'est donc pour justement. Rendent le les pleins droits mais et les mêmes devoirs à à tout. Possédant d'un bien culturel. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention il n'est pas vous adoptez l'amendement numéro 3 Monsieur sanctionne. Madame la Ministre, cet amendement vise à prévoir la possibilité de passation d'un accord entre la personne publique détentrice de l'oeuvre ou du bien est classé et le propriétaire ou ses ayants droit qui la récupère si Le Havre n'est pas tombé dans le domaine public bien entendu aussi celui de son auteur ou de ses ayants droit, je tiens à rassurer madame la rapporteure sur ce point notre amendement renvoie expressément à l'article L 100 mène 2 IV du code de la propriété intellectuelle qui dispose. Toute représentation reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause était licite. Ainsi, le cas échéant, c'est-à-dire lorsque le vent sera encore sous droits la Corse sera tripartite et associera le 1er concerné de toutes les parties de l'auteur du bien restituer ou son ayant droit. Cet accord a pour objet de permettre la reproduction de cette oeuvre selon les modalités qui pourront être déterminées entre les parties au terme d'un accord soit une photographie soit un hologramme une représentation en 3D. Le but, le but étant de garder une trace de l'oeuvre qui constituait préalablement une part de l'identité de la collection publique. Ainsi la reproduction. Pourrait figurer en lieu et place de l'Oeuvre restituer cet amendement répondent donc à une double préoccupation, celle de pas du partage universel du bien culturel mais aussi celles pédagogique permettant au musée ou à l'institution concernée de garder une trace de cette oeuvre et de communiquer sur la restitution. Voilà l'article L 122 4 et très précis sur cette question et il ne prête pas à confusion. On a pu en discuter en commission mais on a retravaillé cette question depuis et il y a pas de, de problèmes majeurs sur cette question. Merci, merci madame la rapporteure votre avis. Si on peut comprendre l'intérêt de préserver l'accessibilité au public des biens culturels et de mieux rendre compte des spoliations et de la restitution des biens spoliés. L'adoption de cet amendement n'est pas souhaitable d'une part les établissements culturels ont la possibilité de conclure des accords avec d'autres personnes publiques ou privées sans avoir besoin de passer par une base légale à cet effet. D'autre part, ce n'est pas le propriétaire du bien culturel

de retirer ou de donner un avis, enfin ta défavorable. Madame la ministre. Merci madame la présidente. Monsieur le sénateur effectivement en fait l'objectif de votre amendement. On peut déjà y répondre avec le code de la propriété intellectuelle aujourd'hui mais il y a quelque chose qui me gêne derrière. L'idée que cette restitution. Ce que j'entends moi au fond c'est qu'elle serait un appauvrissement des collections et qu'il faudrait compenser. Cet appauvrissement alors qu'en fait ces Oeuvres si on les restitue parce qu'elles auraient jamais dû entrer dans les collections publiques donc elles doivent retrouver leur propriétaire avec 80 ans de retard, voire plus. Le temps qu'on les retrouve donc je, je ne vois pas là la question n'est pas le partage universel dans biens culturels comme vous le dites, c'est celle du retour d'un bien privé à ses propriétaires, qui ont été spoliés. Donc je je trouve. je je suis pas à l'aise avec votre amendement je je suis défavorable. Monsieur le sénateur, pour. Explications de vote. Oui je crois que le le le le texte que j'ai cité est claire là-dessus, on parle bien de de de de l'oeuvre d'art et de son auteur. C'est clair, l'article est très clair dessus. Quant à votre remarque Madame la Ministre. Bien entendu que on ne fait que réparer ce qui ce qui n'aurait jamais dû être c'est-à-dire le le vol ou. mais en même temps une oeuvre de dimension culturelle, elle est universelle et elle doit être partagée par tous et donc il est pas question de retirer Alain. Pour que les autres ne ne puisse plus en profiter. C'est ça la question. Il faut restituer. Mais en même temps continuer à faire profiter. Nous même nos enfants les, et d'ailleurs ça permettra de, d'expliquer pédagogiquement ce qui s'est passé parce que c'est ça qui est intéressant c'est l'oeuvre d'art et en même temps, la démarche que nous entreprenons nous tous ici, de restitution et on pourra expliquer à nos enfants mais que ce qui s'est passé dans cette affaire-là et je crois que ça en vaut la peine de continuer à perpétuer. Le souvenir de cette histoire là et ça rejoint le débat que qui a été anémie Monsieur Brisson pour explication de vote. Sans prolonger nos débats je moi je voudrais dire que je partage le malaise qui vient d'être exprimé de pas par Madame. La ministre sur l'amendement de notre collègue et je ne voterai pas. Je vais donc on voit cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention il n'est pas z'. Nous passons à l'amendement numéro 12 Madame de Marco. Merci. Mais dans la présidente Madame le Ministre, mes chers collègues. À la suite des travaux engagés au Sénat l'initiative notre ancienne collègue Corinne Bouchoux. Ce projet de loi instaure une procédure permanent déclassement d'Oeuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous soutenons cette volonté d'accélérer la restitution. Cette procédure lève une importante rigidité qui obligerait le recours à une loi classement par des classements comme elle a été fait avec la loi du 21 février 2022. Afin également de renforcer le droit des propriétaires spoliés et de leurs ayants droit. Nous proposons de renforcer l'opposabilité de la décision de la Commission. D'indemnisation des victimes de spoliations en prévoyant que les avis soient rendus publics. Merci madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. qui sont intervenues du fait des des législations antisémites pendant l'occupation. C'est la raison pour laquelle ces avis ne sont pas jusqu'alors sur le cas lors rendu public, même s'ils sont évidemment transmis aux demandeurs. Le projet de loi confie à la CIV le soin non de formule formuler des recommandations, mais de donner son avis sur l'origine spoliés des biens appartenant aux collections afin d'assurer la plus grande transparence de la procédure il paraît souhaitable que ces avis puissent être rendus publics. Cela permettra sans doute de faciliter l'établissement progressif d'une doctrine et plusieurs commissions équivalente à la CIV. À l'étranger publie d'ailleurs le contenu de leurs avis. C'est pourquoi la Commission a donné un avis favorable. remercie, madame la Ministre votre avis. Merci madame la présidente, avis favorable également toujours d'accord pour plus de transparence. Merci. Si je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avides. 2. Avis favorable pardon qui vote pour. Contre, abstention il était adopté, je mets aux voix l'article premier ainsi modifié qui votent pour, contre, abstention il était adopté des amendements à l'article de l'amendement numéro 5 Monsieur Ouzoulias. Merci la la présidente madame il c'est éteint un amendement de coordination qui reprend la. La formulation que nous avons voté précédemment. Merci. Merci madame la rapporteure. Je n'aurais pas dis mieux. Donc la vie favori. Bien Madame la Ministre même avis je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis favorable. Monsieur Brisson. Vous vouliez prendre la parole, c'était pour le vote. Très bien. Donc qui votent pour qu'ils votent contre, abstention il était adopté l'amendement numéro 8 Madame Goulet. Demande de de coordination avec la l'amendement rectifié. Qui a été votée à l'article précédent, c'est-à-dire que, à la place de l'État français c'est régime de Vichy. C'est un amendement de cohérence. Quel est votre avis sur ce 8 rectifié madame la rapporteure. On ne vous avez un avis défavorable sur l'article 7 donc je aussi un avis défavorable sur cet article 7, la commission était parti sur un avis défavorable également. Madame la Ministre même avis défavorable. pardon madame la présidente, je relisais le fameux article. Que vous avez à amender et je me dis qu'il y a quand même encore des mots sur lesquels il faut revenir parce que le texte se disaient notamment l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français. Donc là vous avez remplacé se disant gouvernement de l'État français par le régime de Vichy mais il reste l'autorité de fait avant, donc il faut il faut être réajustés tout ça là je je ne suis pas juriste mais je, je vous le signale et je reste sur le même avis. De gare de revenir au texte initial, pour ma part puisque ça avait fait l'objet de plusieurs échanges avec le conseil d'état, donc je reste sur l'avis défavorable.

Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. J'ai mes aux voix l'amendement numéro 13 je sais pas je ne aimais pas aux voix mais. Je vous demande de le présenter, chers collègues. Madame de Marco. L'amendement numéro 13. Oui merci. En miroir avec article un premier qui concerne les collections publiques. L'article 2 établit des règles de de restitution applicable aux personnes privées labellisé Musée de France. Parmi les plus de 1200 musées de France 13% relève de personne morale de droit privé associations fondations. Pour les personnes privées ce Label donne accès à des subventions publiques à des dispositions fiscales avantageuses à des transferts de propriété de notre musée de France et de bénéficier de dépôt de musées nationaux. Pendant l'occupation des collectionneurs privés ont pu acquérir des biens culturels spoliés à des familles juives au même titre que des collectionneurs privés. Or pour ses fondations et associations privées. L'article de ne prévoit qu'une possibilité de restitution et dont une restitution systématique ce qui existait déjà. À terme, cela risque de fragiliser les collections publiques face aux collections privées dérogeant à toute obligation de restitution. Les principes de Washington et l'obligation de réparation sont supérieures ne semble-t-il à la protection de la propriété privée qui plus est lorsqu'elle est mal acquises. Les États-Unis par exemple, sont par exemple beaucoup plus intransigeante dans l'application du principe bien mal acquis ne profite jamais. Dans ce cas précis, c'est pourquoi nous proposons cet amendement de remplacer les mots pas peuvent être pas les mots sont. Merci madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît sur cet amendement. Il n'est malheureusement pas possible de contraindre un musée privé à restituer un bien spolié dans la mesure où il le propriétaire de ces collections, et que la décision de restitution ne relèvent que de lui. Je veux croire que les dispositions de l'article 2 auront ah un rôle incitatif sur les musées privés quand bien même s'il ne s'agit que d'une simple faculté d'autre part parce que la CI vs sera préalablement saisi pour avis, pour caractériser la spoliation d'autre part parce que la procédure ménage la possibilité d'une supervision par le Haut Conseil des musées de France. Il est évident que le Haut Conseil des musées de France qui assure le secrétariat de ce Haut conseil engagera un dialogue avec les propriétaires de l'établissement si celui-ci refusait de restituer

Merci madame la présidente, madame la sénatrice de Marco en fait effectivement le juge judiciaire et le gardien de la propriété privée et à même d'ordonner des mesures de réception à une personne morale de droit privé, en application des dispositions de l'ordonnance du 21 avril 45 en cas de litige cette loi, elle peut inviter les personnes morales de droit privé à suivre l'avis de la si vs mais en cas de non-restitution en méconnaissance de la vie de la Civette les ayants droit disposeront de cet avis pour étayer en fait et en droit leur requête devant le juge judiciaire. je comprends vraiment l'intention de votre amendement mais malheureusement on ne peut pas. Légalement. Iliad favorable avis défavorable. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention il n'est pas adopté, j'ai mais voix l'article 2 qui votent pour. Contre, abstention il était adopté des amendements. Après l'article 2 amendements additionnels l'amendement numéro 14 Madame de Marco. Madame la rapporteur vous citez dans votre rapport, le rapport d'information publiée en 2013 par le Sénat après les travaux conduits par notre cause anciennes collègues, historienne. Corinne Bouchoux que j'ai déjà cité plusieurs fois. À la page IV de la note de synthèse de ce rapport, la mission d'information souligné le frein résultant d'une inaccessibilité des archives pour établir la trajectoire des acquisitions d'Oeuvres. Je cite l'accessibilité des archives illimité, ce qui est contraire au principe numéro de de Washington non seulement certains accès sont limités ou inexistants. Comme certaines archives du Louvre par exemple mais parfois les conditions matérielles de stockage et de l'indexation constitue un obstacle à la recherche de provenance. L'action entreprise par le ministère des Affaires étrangères pour moderniser ses archives de la Courneuve met en évidence le retard de la France par rapport à d'autres pays. Les archives nécessaires à la mission de restitution ne sont pas seulement celle du ministère de la culture mais celle de tous les ministères et il aurait été concerné par les lois d'arguer d'aryanisation par les spéculations et par les déportations. C'est pourquoi il importe de lever toutes les entraves juridiques d'accès aux archives nationales et de prévoir une règle dérogation exceptionnelle aux règles d'accès aux documents administratifs sensibles habituellement protégés par le secret. Telle est l'objectif de cet amendement. Madame la rapporteure votre avis. Oui, l'accès aux documents d'archives évidemment une condition essentielle pour parvenir à la recherche des documents de commenter de correctement le parcours des biens culturels la ne semble pas pour autant rencontrer de difficultés particulières pour accéder au fonds d'archives. Elle a conclu plusieurs partenariats avec des institutions en France comme à l'étranger afin de faciliter sa consultation pour exemple le et le décret de 2015 a notamment permis d'ouvrir des archives des juridictions d'exception de Vichy, celle des juridictions d'exception du gouvernement provisoire de la République. Les archives de la police judiciaire de 39 45 et de 45 à 60 pour les affaires relatives à des faits de guerre survenue entre 39 et 45 et plus il y a quand même des décrets qui ont permis d'ouvrir les deux des archives de la seconde guerre mondiale qui a été soumis à des des de communication et qui sont ouverts maintenant et ou qui étaient couvert par le secret défense, mais qui sont ouverts, maintenant il y a donc pas de près. Lieu de prévoir une dérogation particulière à ces règles de communicabilité au profit de la CEI vs d'autant que l'article L point de 113 très très tiré 3 du code du patrimoine rang de toute façon possible la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais de communicabilité fixé dès lors que l'intérêt qui s'attache à la consultation consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger donc la consultation des documents peut se faire et je vous propose donc. Je vous donne donc plutôt un avis défavorable sur ce. Ou un retrait de votre amendement. Merci madame la ministre. Merci madame la présidente, effectivement. Madame la sénatrice de Marco. Aujourd'hui, nous nous voyons aucune difficulté dans l'accès aux archives publiques qui concerne la période de la Seconde Guerre mondiale et les spoliations. Il a pu en avoir évidemment dans le passé, mais ce n'est plus le cas. Les archives de l'État sont accessibles, les archives nationales, les archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, accueil de, de très nombreux chercheurs sur ce sujet le délai de consultation des procès-verbaux des commissaires priseur qui doivent être versés par ces derniers, aux archives départementales reste fixée à 75 ans, mais les procès-verbaux des ventes de la période de la guerre sont accessibles puisque nous sommes aujourd'hui 79 ans après la fin de la guerre en France pour des ventes plus récente, il est toujours possible de demander un accès dérogatoire et je voulais aussi vous rappeler que le gouvernement a en deux temps accordé une dérogation concernant l'accès aux archives relatives à la seconde guerre mondiale. Il y a eu l'arrêté du 24 décembre 2015 qui a permis la libre consultation avant l'expiration des délais prévus dans le code du Patrimoine de l'ensemble des archives, notamment celles qui relèvent du ministère de l'Intérieur et de la justice mais aussi du ministère des Affaires étrangères et il y a eu une circulaire le d'octobre 1997 qui. Relatives à l'accès aux archives publiques de la période 1940 1945. Donc tout ça est déjà possible demande de retrait pour ma part. Merci. Pour l'explication de vote Madame de Marco. Mais des explications de Madame la rapporteur mesdames la ont convaincu je retire. Gardez le micro puisque vous présenter l'amendement numéro 17. la restitution ou la réparation pas constituer un effort nécessaire, y compris pour les collectivités territoriales. Afin que la responsabilité ne pèse pas que sur elle, tous les intermédiaires du marché de l'art devrait être responsabilité. Pour mener à bien la mission de restitution. C'est parfois déjà le cas, je pense notamment aux gestes d'une maison d'enchères au moment de la restitution du tableau Carrefour à Sannois du peintre Maurice Utrillo spoliés 1942 à l'initiative du maire de la ville de Sannois. cette cette participation active des maisons d'enchères marchande Apps devraient être systématisés. C'est pourquoi nous proposons de fixer la lutte contre la vente des biens spoliés parmi les missions du Conseil national maison de vente. Si nous voulons accélérer les institutions de nous devons douter de tous les moyens pour le faire. Madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. Je reste sur la position d'avoir un avis de retrait ou défavorables, parce que, parce que je pense que nous avons déjà tout ce qu'il faut et que ça me paraît compliqué de, d'aller au-delà. Madame la Ministre même avis. Madame la sénatrice, je mets aux voix votre amendement, vous le retirer. Pardon si vous affirmez que nous avons tout en notre possession, je retire mon amendement.

Oui ce présent amendement vise à permettre au Parlement de rester informés de l'ensemble des restitutions de biens spoliés réalisés au cours de l'année calendaire. L'adoption de cette loi cadre sur les restitutions des biens spoliés dans le contexte de 1933 à 1945 ne peut faire ni l'économie d'un inventaire précis de nos collections ni d'une information de qualité sur l'évolution de ces restitutions. Il en va du respect des ayants droit spoliés et de la vigilance que nous devons porter sur nos collections. Or le présent projet de loi écartera de la procédure de restitution de Parlement puisqu'on lui substitue les lois d'espèces à un dispositif pérenne dérogeant au principe d'inaliénabilité des biens culturels du domaine public afin de simplifier le dispositif de restitution des biens. Les parlementaires que nous sommes vont se voir donc retirer leur capacité d'examens et d'appréciation du bien-fondé de ces restitutions la remise de ce rapport, permettrait au Parlement de ne pas quitter définitivement la procédure de restitution de ces biens. Par ailleurs, face à l'éparpillement lié aux différentes procédures de restitution de ces biens et par souci de clarté, il paraît nécessaire de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des biens restitués en consultant un unique le document. Là pourquoi présente cet amendement. Merci madame la rapporteure votre avis. a plutôt tendance à, à ne pas accepter ce genre de disposition il peut sembler logique d'assurer une information du du parlement maintenant qu'il n'autorisera plus le cas au cas par cas les restitutions donc la commission donne un avis de sagesse. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, avis de sagesse également. Très bien je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis de sagesse. Qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient il être adopté, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi il y a-t-il des demandes d'explications de vote. Madame Goulet pour explication de vote.

je je voulais. Évidemment à ce moment précis. Remercie le gouvernement. Et et le travail de de la commission. Restant. Convaincu. Que même si l'ordonnance de 44, celle de 45, ont une valeur législative, je pense que. Le terme ce 10 ans demeurant. Il est absolument normal la la Ministre que les décisions du Conseil d'État, se fondant sur un texte existant et de mon point de vue rédigé de façon inappropriée. En 2023, mérite qu'on lui ait retravaille alors je ne sais pas si ce sera possible dans le cas de la commission mixte paritaire. À mon sens il y a quand même un problème d'éclaircissements avec ce, avec qui reste. En suspens par rapport à la réalité. De l'histoire. Ceci étant je je trouve que le texte est est parfait. Sous réserve de cette. qui je crois est utile. D'un point de vue historique. Comparaison des pas raison mais vous avez eu des dizaines de textes qui étaient en francs et qui ont été transformés en euros, vous avez une évolution législative sur un certain nombre de points pour lequel le vocabulaire change en fonction du, du temps je crois qu'il faut retravailler ce, ces, ces ces 2 alinéas de façon à ce qu'il soit plus en conformité avec l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui et non pas celle qu'elle était juste au moment de l'après-guerre mais évidemment notre groupe votera avec enthousiasme. Ce texte telle que proposée par la Commission et néanmoins amendé par notre haute assemblée. Merci monsieur Brisson pour explication de vote. est un triptyque dont on a déjà parlé donc Pierre-Antoine Levi en particulier a parlé tout à l'heure, c'est le premier acte. Un second interviendra en vue

après sur le texte, nous avons travaillé cet après-midi j'ai un petit malaise parce que il y a comme discordance entre l'article 1er et l'article 2 qui mérite aura. Que nous retravaillerons enfin il y aura une navette mais je regrette un petit peu que sur un sujet aussi important et à partir du texte vous avait porté. On ne doit pas arriver à une écriture plus satisfaisante mais nous voterons. Bien entendu, ce projet de loi. Merci monsieur Ouzoulias pour explication de vote. Merci madame présidente madame la miss mais mes chers collègues. Ce texte est d'apparence technique et je crois que c'est justifié parce que le président Roger Karoutchi. L'dit avec beaucoup de force. Je je je dois le répéter. Jamais un texte de loi pourra. Réparer ce qui a été la Shoah. La Shoah est une une plaie ouverte au flanc de notre humanité et il faut que très humblement en faisant la loi nous ayons le le sentiment de, d'apporter une réponse de droit et pas réparer l'irréparable. Ce que nous avons essayé de de poser ensemble avec vous et avec le gouvernement. Dans une relation de confiance que je salue hein et et d'un travail collaboratif qui a a montré que nous aurions pu commencer comme ça sur les lois précédentes. Je je je referme la parenthèse mais ce que nous avons essayé de faire c'est de poser des critères juridiques des critères de droit très forts pour permettre ensuite la pleine transparence des procédures de transposition hein et je le je le redis, je pense que la façon dont vous avez organisé l'instruction des des des dossiers avec une commission scientifique une commission administrative est un très bon modèles parce qu'il permet la recherche scientifique et je j'espère vivement que demain, les universités vont et persil vont y participer pleinement je vois en tant que ancien enseignant l'université des innombrables projets de, de recherche de thèse et je crois qu'on peut faire justement collaborer. La jeune génération à tout ce travail de de mémoire et de récolement des données et à côté il y a une commission administrative qui est composé de de de juriste et qui donne un avis au gouvernement, je pense que c'est la bonne voie et je m'associe aux propos de mon collègue. Max Brisson pour pour souhaiter que le 3ème texte puisse s'inspirer de la méthode que nous avait mis en place ce soir. Merci ma président. Oui Madame la Ministre. Je crois que nous, on est satisfait de, de ce travail que nous avons menés ensemble même si nous aurions aimé quelques améliorations qui ont pas pu arriver à leur terme mais. Il n'empêche que c'est, c'est quand même un moment il ment historique Notamment ces améliorations le le viser à à pouvoir continuer à expliquer ce que ce que ce que nous faisons en, en décidant ce soir de de créer l'automaticité de la restitution. il ne faut pas que la l'automaticité soit synonyme d'oubli. C'est-à-dire qu'on règle ça de façon administrative. Et que. Des gestionnaires de de musée ben restitue sans que en fait on, on puisse en reparler puisque chaque fois que nous venions. Au parlement pour débattre de la restitution d'un objet ça faisait l'objet d'un débat. Large et qui a d'ailleurs qui sortait. donc prenant le soin de de trouver le moyen de continuer à parler de de de de cela et puis comme ça a été dit auparavant dans le triptyque des des textes que nous avons à travailler. Il en reste encore deux. et notamment le troisième sur la restitution des des biens mal acquis. Je pense que là aussi c'est quelque chose d'important il y a il y a une réparation aussi historique. Majeure. Que nous allons conduire et que et que il faudra que nous y travaillons vraiment avec autant de sérieux que ce que nous avons fait présentement voilà merci. Et monsieur Fiole. Pour explication de vote. Oui madame la présidente. Nos collègues Karoutchi Ouzoulias sont ont dit que c'était un texte. Effectivement techniques qui ne prétendait pas. Corrigé réparer. Toutes les atrocités qui ont été commises et et les inactions.

Alors il doit aussi au au-delà avant que se fasse la restitution. Il y a tout le travail de recherche de provenance, qui est un travail extrêmement important pour lequel il faut former. Des Des professionnels, il y a des formations qui débute juste et qui doivent être développées. Donner des moyens aussi pour pour qu'ils soient faits, parce que chaque travail. De recherche est aussi un travail de mémoire et d'entretien de cette mémoire Merci madame la présidente.

et toutes les personnes que nous avons rencontrés et également qui nous ont apporté leur éclairage leur témoignage leur expérience qui nous a permis d'enrayer film d'enrichir le texte, mes collègues avec des amendements qu'on a pu accepter ou d'autres qu'on n'a pas refusé mais qui nous ont fait travailler. Réfléchir sur les propositions et sur les ouvertures et puis enfin Madame. Madame la Ministre pour ce travail et et tout ceux qui ont pu même accompagné et bien sûr Aurore qui n'est pas parmi nous parce qu'avec son petit souci de santé mais qui a largement travaillé et avec son expertise que je remercie très de façon très importante. Merci à vous. Merci, monsieur le Président la font. Si madame la présidente. Ce texte n'a pas vocation à réparer la Shoah comment pourrais.-t-on le le prétendre, il a vocation à. Réparer les spoliations et rendre justice et aux familles et aux personnes qui en ont été. et bien sûr nous devons nous satisfaire de ce consensus et surtout de de ce vote qui va intervenir dans. Dans quelques minutes, qui va permettre d'accélérer, j'allais dire enfin accélérer le processus de de restitution. Moi je voudrais donner de date et un chiffre pour nous appeler aussi à la modestie de dates 1933 2023, 90 années pour parvenir enfin. À. Faire ce travail de de justice 90 années c'est-à-dire ces 3 générations et comment ne pas penser aux générations qui ne sont plus là et qui ont été victimes directement. De ces spoliations nous leur devions aussi ce ce travail. 19.195 2023 19.195. C'est les déclarations du président Chirac et beaucoup parmi vous l'ont rappelé à l'occasion de ce débat et c'était nécessaire de de le rappeler parce qu'on voit bien. Comment ça a pu déclencher un processus auquel nous arrivons aujourd'hui il a quand même fallu 28 ans depuis les déclarations du président de la République Jacques Chirac. Pour parvenir à ce texte. Cadre et puis enfin dernier chiffre c'est le nombre de spoliation qu'on ne connaît pas mais quand on parle de 100.000 ou 150.000, on mesure. L'. L'importance des spoliations commises. Il faut dire en toute modestie que bien sûr nous n'en restitue rond sous une forme ou sous une autre que très peu. Aux. Aux familles qui en ont été. Victimes et qui portent encore dans leur histoire cette période. période. De l'histoire de France. Bien sûr je vais me joindre d'abord remercier là notre rapporteur. Sur le travail fait me me joindre aussi à la demande qu'elle a formulées dans son propos initial. Parce que ce texte à vocation à accélérer le processus et pour accélérer le processus, il faut aussi qu'il y ait des moyens notamment humains qui soit mis pour. Accélérer le travail de d'identification des provenances et et et de restitution. Donc je me joins à la demande. Faite auprès de l'État est à madame la ministre en particulier. Sur la nécessité de de d'adjoindre des moyens à à cette loi-cadre et et remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé remercie aussi Madame la Ministre. Du de la collaboration faite sur ce texte. Et dire que nous attendons avec impatience bien sûr les 2 autres textes. Merci je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés entre 1933 et 1945. Qui vote pour. Contre. Abstention. Merci pour cette unanimité. Madame la ministre, je crois que vous souhaitiez prendre la parole en conclusion. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité de ces débats-là le sérieux de ses analyses et de tous nos échanges ces dernières semaines, Heureuse que le texte comment son cheminement législatif par le Sénat parce qu'il y a aussi eu un travail de longue date du Sénat, nous avons mentionné le travail de la sénatrice Corinne Mondou notamment. Mais aussi, c'est avec les sénateurs que nous avons le plus travailler sur les prochaines lois-cadres, qui seront débattues. Et qui vont arriver très bientôt, je voulais. Également redire. Le président Karoutchi n'est plus là mais que dans mon discours, j'ai veillé à peser chaque mot et que j'ai bien dit que la réception est un acte de justice et non pas un acte de réparation. Et j'ai dit plusieurs fois que rien ne pourrait réparer le drame de la Shoah qui n'est comparable avec aucun autre drame d'ailleurs. Mais c'est une loi de reconnaissance. C'est une loi d'action et je voulais vous assurer de l'engagement total du ministère de la culture de nos musées. Des équipes dans les musées et pas uniquement celle des musées nationaux, mais pour avoir échangé avec celle des musées territoriaux aussi je je connais leur engagement, leur mobilisation. La l'engagement aussi sur les formations je l'ai cité rapidement dont discours liminaire mais il y a aujourd'hui cette prise en compte dans les formations qui est très importante avec un nouveau master aussi à Nanterre. Mais dans les formations de l'École du Louvre de l'Institut national du Patrimoine, c'est avec l'ensemble de ces leviers formation enquête recherche de provenance. Que nous allons rendre cette loi. Effective et je voulais vous assurer de mon engagement pour la rendre effective, merci 1000 fois. Je vous Je vous remercie, madame la Ministre je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. La parole est à Madame Micheline Jacques pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci madame la présidente donc de, je tiens à faire la mise au point suivante sur le scrutin public numéro 291, mes collègues Françoise Dumont Viviane Malet et Dominique Le Lège souhaitaient voter pour. Merci, avec les données de votre mise au point figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une majorité numérique il a lutté contre la haine en ligne. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications.

L'insécurité sur Internet progresse de jour en jour et nos enfants sont les principales victimes des travers. De la société numérique. Surexposition aux écrans. Addiction aux réseaux sociaux. Cyber harcèlement Exposition à des contenus inappropriés autant d'atteintes brutale à leur innocence. Autant de violence psychologique faite à une génération qui menace d'être sacrifiée. Si rien n'est fait. Alors oui, mesdames, et messieurs les sénateurs. Nous devons à nos enfants d'agir et depuis quelques années sous l'impulsion du président de la République sous l'impulsion des parlementaires. La France agit et d'ailleurs s'agissant de la protection de l'enfance en ligne. La France montre la voie. Grâce à une initiative parlementaire. La France sera dans quelques mois le 1er pays du monde à imposer le contrôle parental sur tous les équipements qui sont vendues sur son sol. Grâce à la mobilisation de l'éducation nationale du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Économie et des Finances l'année prochaine dans notre pays. Tous les élèves de 6ème bénéficieront d'un passeport numérique, c'est-à-dire d'un Module de sensibilisation aux risques et aux gestes gestes à adopter en ligne pour se prémunir contre les dérives que j'évoquais tout à l'heure. Grâce à l'engagement de la secrétaire d'État chargé de l'enfance et du ministre de la prévention, Internet je protège mon enfant Point gouv Point FR a été conçu. Pour les parents, pour les accompagner dans la parentalité numérique, c'est-à-dire dans la façon dont ils peuvent accompagner leurs enfants dans l'espace numérique. Nous avons d'ailleurs avec Charlotte Caubel lancé au mois de février une campagne, une campagne nationale de diffusion. De ce site internet je protège mon enfant Point gouv Point FR vers lequel tous les parents de France peuvent se tourner lorsqu'il s'interroge sur la manière d'accompagner au mieux leur enfant dans l'espace numérique. Et c'est enfin grâce au volontarisme de la France que l'année dernière lorsque la France présidait l'Union européenne a été adopté un règlement majeure le règlement sur les services numériques qui fait entrer les grandes plateformes de réseaux sociaux dans l'air de la responsabilité. En leur imposant un certain nombre d'obligations nouvelles d'ordre général. La modération des contenus illicites qui leur sont signalés. Le l'audit par des tierces parties de leurs algorithmes. Le partage avec des chercheurs de leur donner ce qui permettra aux chercheurs d'analyser les les les ressorts des des dérives que que nous dénonçons, mais aussi des mesures très concrètes Crète pour mieux protéger les enfants. En ligne et en particulier l'obligation qui leur sera faite de publier des conditions générales d'utilisation facilement compréhensibles par les enfants. L'obligation de garantir un haut niveau de sécurité. De sûreté et de protection de la vie privée des enfants notamment en mettant en place des interfaces adéquate et puis l'interdiction de faire de la publicité ciblée sur les mineurs. Je le répète, c'est là un règlement majeure, une révolution dans la manière dont nous régulons l'activité de ces éditeurs de réseaux sociaux et ces obligations entrera en vigueur cet été au mois d'août 2023. Et en cas de manquement à ses obligations. Les plateformes concernées s'exposeront à des pénalités allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. La première fois et en cas de récidive. Une pénalité allant jusqu'à l'interdiction d'émettre sur le territoire de l'Union européenne. Nous avons agi, mais il nous faut aller plus loin. C'est l'objet du projet de loi que j'ai présenté il y a quelques semaines et qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique et qui créent de nouvelles protections pour nos concitoyens, nos entreprises et nos collectivités mais singulièrement pour nos enfants. Et au chapitre de la protection des mineurs en ligne figure une mesure qui est issu des travaux de madame la la rapporteure et de ses collègues. Les sénatrices Billon. Cohen et Rossignol et qui vise à donner à l'Arcom, le pouvoir de bloquer. Les sites pornographiques qui ne vérifie pas l'âge de leurs utilisateurs de millions d'enfants chaque mois. Mesdames, et messieurs les sénateurs sont exposés à des contenus pornographiques en ligne. Pourquoi, parce que les sites concernés ne vérifie pas sérieusement l'âge de leurs utilisateurs. Avec cette mesure issue d'un rapport sénatorial nous pourrons en quelques semaines, obtenir le blocage des sites qui ne se conformeront pas à cette obligation. Autre mesure de protection de l'enfance en ligne une peine d'un an d'emprisonnement et 250.000 euros d'amende pour les hébergeurs qui ne retireront pas en moins de 24h les contenus pédopornographiques qui leur seront signalés par les forces de l'ordre. Une sanction qui sera calqué sur le modèle de la sanction s'appliquant au non retrait des contenus terroristes par. Ces mêmes hébergeurs. il nous faut aller plus loin avec cette proposition de loi. Qui a été initié à l'Assemblée nationale par le président Laurent Marcangeli et qui vient imposer aux réseaux sociaux de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, mais aussi lorsque leurs utilisateurs ont moins de 15 ans de recueillir le consentement parental et je veux féliciter la rapporteure et les membres de la commission qui ont permis d'améliorer le texte lors de son examen en commission. Tout en veillant à éviter 2 écueils. Le 1er c'est d'empiéter sur ce qu'accomplit le règlement sur les services numériques. Le DSA, comme je le disais tout à l'heure ce règlement majeurs adoptés l'année dernière, à l'initiative de la France et le 2ème c'est de déposséder l'autorité. Parentale. Je crois que compte l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu, le Parlement s'est trouver les voies du consensus. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Tout cas le gouvernement madame la ministre aura l'occasion de de s'exprimer en en ce sens soutiendra. La proposition de loi amendée par la la la commission. Et et je remercie une nouvelle fois la rapporteure et les membres de la commission pour leur travail. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à présent madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargé de l'enfance. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs. Nous le disons, nous le répétons l'espace numérique apporte au monde des atouts formidables, mais aussi des sources de danger, et tout particulièrement pour les enfants qui naviguent sur Internet dès l'âge de 10 ans, parfois même avant. Dans le monde réel comme dans le monde virtuel, il est de notre devoir de garantir la sécurité. Les droits et le bien-être de nos enfants. C'est pourquoi la protection des enfants dans l'espace numérique et l'un des 5 chantiers prioritaires fixés par la Première ministre à son gouvernement à l'occasion du 1er comité interministériel de l'enfance en novembre 2022. Notre feuille de route est très clair, il nous faut lutter contre l'utilisation excessive des écrans qui génère de nombreuses difficultés et de nombreux troubles du comportement de langage des addictions, des troubles du sommeil, il nous faut aussi interdire aux mineurs l'accès à des contenus inadaptés à leur âge, au 1er rang desquels les contenus pornographiques sur ce point. Jean-Noël Barrot et moi sommes intransigeants. Nous avons pris des mesures plus contraignantes encore qui s'appliqueront aux éditeurs de sites pornographiques. Il nous faut aussi combattre toute forme d'infractions dont les mineurs peuvent être victimes sur Internet au 1er rang desquels le cyber harcèlement et le gros. Enfin, il nous faut garantir les données et le droit à l'image des enfants sur les réseaux Sochaux, je le rappelle, une image sur 2 retrouver dans les ordinateurs portables des pédocriminels est une image d'enfants volés sur les réseaux une image sur deux. Depuis un an, nous sommes tous pleinement mobilisés avec l'ensemble des ministres concernés. Je souhaite saluer l'action de mes collègues Jean-Noël Barrot Pap Ndiaye mais aussi Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti pour lutter contre les excès des réseaux. Nous pouvons également compter sur l'engagement des parlementaires des 2 chambres. Les autorités de régulation et de nombreuses associations. Car, collectivement, nous prenons tous les jours un peu plus la mesure des risques que représentent les écrans Internet et les réseaux sociaux pour nos enfants. Je me réjouis en tant que secrétaire d'État chargé de l'enfance de constater que nous conduisons à tous les niveaux, une véritable stratégie pour prévenir les risques. Mieux accompagner les familles responsabiliser les acteurs du numérique notamment les plateformes. Au Parlement, 3 propositions de loi visant à mieux protéger les enfants en ligne sont ainsi examinés depuis le début de l'année. C'est un message politique très clair et très fort. Caroline janvier Bruno Studer et Laurent Marcangeli, ont en effet porté des textes ambitieux à l'Assemblée nationale a adopté très largement. Au Sénat, des travaux importants nourrissent notre action au quotidien. Je salue bien sûr le rapport porté par Annick Billon Laurence Rossignol, Laurence Cohen, et vous madame la rapporteure sur l'industrie de la pornographie et bien sûr la commission conduite par le président Maluret sur TikTok. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je suis ce convaincu que la protection des enfants ligne peut une nouvelle fois nous réunir nous unir aujourd'hui. Je ne crois pas me tromper en disant comme vous qui nous est insupportable de lire des rapports qui font état de dégâts causés par les algorithmes addictif la désinformation. Les violences commises sur les enfants en ligne. Loin de moi l'idée de diaboliser les réseaux sociaux et les grandes plateformes mais en tant que secrétaire d'État chargé de l'enfant. Je me dois d'alerter sur ces risques et d'Éric grave qui abîment la santé des plus jeunes. Il faut l'admettre. Nous avons été dépassés, nous adultes. Nous avons probablement baisser la garde par imprudence et surtout par méconnaissance, et incompréhension. Jean-Noël Barrot là dit aujourd'hui nous sommes dans l'action pourra après peut-être le temps perdu. Face à ces défis, nous avons choisi plusieurs choses. Nous avons choisi de renforcer l'éducation des enfants, de renforcer l'accompagnement des parents et la formation des professionnels. Nous avons choisi de généraliser les ateliers de parentalité numérique sur l'ensemble du territoire, nous renforçons les dispositions et donc les obligations résultant de l'autorité parentale dans l'environnement numérique. Et nous pouvons aujourd'hui en cette assemblée déterminer l'âge à compter duquel un enfant peut de façon autonome s'inscrire sur un réseau social. Il nous faut à nouveau rappeler une évidence s'inscrire sur un réseau social n'est pas un acte anodin. En particulier lorsqu'on est encore enfant.

là où il y avait harcèlement. Aujourd'hui il y a cyberharcèlement. Qui décuple démultiplie l'impact sur les enfants là où il avait ponctuellement, incitation à la haine et au suicide. Il y a numériquement déploiement de ce type d'influence. Les réseaux sociaux sont sources de danger réel et grave. En cela, contrôler et accompagner l'accès des mineurs à l'entrée des réseaux est une réponse efficace. C'est pour cela que avec Jean-Noël Barrot, je soutiens la proposent, ils soient proposition de loi de Laurent Marcangeli pour qu'aucun enfant de moins de 15 15 ans de s'inscrivent sur un réseau social sans l'accord de ses parents. Ce sera un nouveau moyen d'accompagner les enfants dans leur j'usages numériques et de les préserver des excès d'Internet. Je sais qu'en privilégiant l'intérêt supérieur de l'enfant, il peut nous être reproché de porter atteinte à la liberté des adultes. En l'occurrence, nous leur rappelons de ne pas céder à la facilité et de prendre leurs responsabilité je l'assume, nous ça nous assumons parce que prendre soin de nos enfants et la priorité du président de la République. La priorité du gouvernement est ma priorité entrant que secrétaire chargé de l'enfance. Je vous remercie. Merci la parole est à présent à madame Alexandra Borchio-Fontimp. Rapporteur de la commission de la cuve. De l'éducation et de la communication. Vous avez 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans leur monde idéal, les réseaux sociaux constitue un formidable espace de partage de créations, d'échanges et de débats. Un outil de culture également de connaissance. Un idéal qui est malheureusement restée en partie une projection, c'est-à-dire à l'heure mais qui a réussi son envolée en absorbant de nombreux utilisateurs tomber dans le piège. Avant d'en connaître les dangers. La plupart d'entre nous ici présents mais surtout les plus fragiles, aveuglés par les sirènes manipulatrice, les autres à faire croire que cet espace de divertissement était sans risque. Conçu pour attirer et retenir notre attention. Les plateformes numériques ont sucré, un écosystème qui fait désormais partie de la société. Nommée rapporteur de cette proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et lutter contre la haine en ligne. Je me suis penché depuis plusieurs années avec une grande attention sur les conséquences de la sur utilisation d'Internet par les mineurs. Je suis aussi mère de famille aujourd'hui d'adolescents et donc quelque part témoin éclairé de ce que génère au quotidien l'utilisation de ces plateformes sur leur vie. L'auteur de la proposition de loi initial a choisi un sujet qui ne peut faire que consensus c'est-à-dire légiférer sur l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux est-il vraiment besoin d'expliquer pourquoi un focus a été fait sur les réseaux sociaux, tant ils sont partout. Nos enfants encore plus nos adolescents n'imagine plus vivre sans eux. Il ne s'agit pas ici de faire un procès aux plateformes ou d'adopter une posture moraliste. Ils ne sont évidemment pas à eux seuls responsables de toutes les dérives constatées sur Internet mais il est impossible de nier qu'il présente pour nous, singulièrement pour les plus jeunes des conséquences spécifiques. Commençons avec quelques chiffres près de la moitié des enfants de 6 à 10 ans ont déjà leur smartphone, ans, je vous le rappelle, c'est l'entrée au CP, c'est-à-dire là où on apprend à lire. 65% des 10 14 ans ont un compte au moins sur un réseau social et près de la moitié des ados pensent qu'il serait dévastée s'il devait se passer des réseaux alors non pas définitivement mais juste pendant plusieurs jours. Cela en dit long sur le caractère addictif des réseaux sociaux. C'est toujours d'ailleurs le même geste d'abord un scroll vers le bas. Un coup d'oeil aux commentaires puis l'entrée dans la spirale, celle qui va transformer vos cinq minutes de pause en un long tunnel sans fin. C'est là d'ailleurs tout l'objectif des algorithmes retenir notre attention coûte que coûte, en choisissant des contenus adaptés à nos intérêts avec 2 variables la satisfaction générés par la réception de commentaires positifs ou autres récompenses et le partage d'expérience afin de montrer son appartenance à une communauté, c'est le marché de l'attention, une sollicitation optimisée du cerveau humain, par le biais d'algorithmes qui engendre une recherche constante de nouveaux contenus numériques à des fins de stimulation cérébrale le même mécanisme d'ailleurs serait à l'oeuvre dans les cas des addictions aux drogues et je vous invite à lire le témoignage, récent d'une adolescente dans un grand quotidien national je cite TikTok pour nous c'est un peu comme le tabac. Pour l'ancienne génération, on essaye de décrocher mais on tient une semaine Mes chers collègues, est-ce que vous connaissez le FOMO. Vous savez c'est la chromie l'acronyme de Fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer de quelque chose, cela se traduit par un syndrome d'anxiété qui nous pousse à rester connecté, afin de ne pas risquer de rater quelque chose un phénomène qui est une conséquence directe de l'utilisation des réseaux sociaux un syndrome particulièrement présent là aussi chez nos adolescents et puis il y a la comparaison qui parfois peut être une source de plaisir mais souvent facteur de déprime. Poison pour l'estime de soi, racines de envie et de la jalousie lorsque nous parcourons les différentes plateformes. On peut avoir la sensation de voyager. Trop peu de se sentir moche au finalement que notre vie de famille bien plus triste que celle des autres. Notre cerveau ne compare systématiquement aux autres finalement, c'est un réflexe plutôt naturelle en tant qu'adulte le discernement nous offre une arme pour prendre de la distance mais cet outil n'est qu'en cours d'acquisition chez nos enfants et ne leur permet pas encore d'avoir le recul nécessaire pour digérer certains contenus. Les réseaux sociaux sont la vitrine d'une vie rêvée hé bien mené et leur sur-utilisation a un impact physique, mentale sociale des chercheurs de l'Université de Pittsburgh se sont intéressés au sujet et les informations scientifiques obtenues affirme qu'un lien Direct existe entre l'isolement social éprouvé et une importante utilisation des réseaux sociaux, maux de tête, insomnie, problèmes de vision des primes baisse des résultats scolaires ou des performances professionnelles tout autant d'indices qui doivent nous alerter, là encore, nos enfants et ados sont bien plus sensibles que les adultes et il a été constaté que les plus gros consommateurs de réseaux sociaux sont les plus jeunes et les premiers concernés par ces risques cognitifs et mentaux en raison bien sûr de leur a des de leur usage démesuré et de leur vulnérabilité aujourd'hui près de 50% des adolescentes présentent des symptômes cliniques de dépression pour un équivalent de 5h par jour passé sur les réseaux sociaux. Encore cinq minutes de TikTok et je vais me coucher. Nombreux sont les parents qui se reconnaîtront dans cette phrase prononcée par leur enfant pourtant depuis plusieurs années, les spécialistes ne cesse d'alerter sur les troubles du sommeil, les difficultés de concentration ou encore la dégradation de la mémoire en cas d'utilisation répétée des écrans la nuit et puis autorisé son enfant à utiliser les réseaux sociaux, c'est une chose mais savoir ce qu'il regarde c'est mieux parce qu'aujourd'hui 82% des 10 14 ans, indique consulter sans leurs parents. Cette forme de liberté véhiculé par les réseaux sociaux où chacun finalement peut prendre la parole peut entraîner également des dérives cette problématique identifié depuis des années désormais s'appelle la haine en ligne une haine qui a trouvé un nouveau corps, un terreau privilégié pour se diffuser de manière lâche un plus grand public et plus facilement derrière un écran, l'anonymat la violence de certaines personnes qui peut s'exprimer bien plus librement un réel espace de défoulement. Pour les autres et puis le début d'un cauchemar pour les autres. Selon l'association et enfance 12% dès 8 18 ans ont déjà été confrontés à une situation de cyber harcèlement c'est un fait, un fléau qui touche particulièrement les mineurs. Si les plateformes mettent en place des outils pour lutter contre des contenus indésirables, il s'avère que ces dispositifs ne sont pas suffisants pour protéger les plus fragiles, nos enfants et n'évoque pas ici les mauvaise rencontre notamment des prédateurs sexuels ou les vendeurs de drogue qui savent bien tirer parti des réseaux sociaux pour attirer leur victime. Premier lieu des interactions sociales ou sont incorporés les notions basiques du civisme, l'éducation nationale qui a aussi pour mission d'apprendre aux futurs citoyens de la République. Quelles sont les règles de vie en société. Notre société faisant de plus en plus corps finalement avec le numérique, le cyber harcèlement doit être abordé en classe ce texte que nous examinons aujourd'hui c'est un texte de bon sens en réaction au constat présentés dans mes propos liminaire. Cette proposition de loi prévoit ainsi qu'en dessous de 15 ans, l'inscription d'un jeune sur un réseau social ne pourra se faire qu'avec l'autorisation d'un des 2 parents c'est donc cela la fameuse majorité numérique c'est l'article 2 et c'est le coeur de la proposition de loi. J'ai tenu à rendre ce texte plus opératoire afin de renforcer la protection de nos enfants avec des amendements adoptés à l'Uni unanimité par la commission de la culture. Ils ont pour objectif est bien de rendre le texte. Plus applicable et efficace tout en associant la CNIL. Pour assurer un meilleur respect des données personnelles. Ce texte place ainsi l'autorité parentale au coeur de la relation entre la l'enfant et les réseaux sociaux fixer une majorité numérique permettra demain d'instaurer un dialogue en famille afin chacun puisse en connaissance de cause et en responsabilité, être conscient des dangers que peuvent engendrer une sur utilisation surtout quand on observe la proportion des moins de 13 ans inscrits malgré je le rappelle. L'interdiction fixée actuellement par les plateformes, ce sera donc un outil au service des parents pour mieux superviser la vie numérique de leurs enfants tout montre que la puberté numérique et de plus en plus précoce et que souvent les parents sont dépassées par la rapidité avec laquelle leurs enfants adoptent de nouveaux usages. Sachez que 83% des parents reconnaissent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font sur Internet. Cet arsenal juridique que nous nous efforçons enfin de mettre en place pour réguler l'espace numérique ne pouvait plus attendre. Il complétera d'ailleurs les deux textes que nous venons d'examiner celui visant à encadrer l'influence commerciale et celui visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. 3 textes. Un seul objectif, protéger les mineurs. Le Sénat a de nouveau prouvé son intérêt pour ces grands enjeux de notre siècle et le Sénat sera de nouveau d'ailleurs au rendez-vous dans quelques semaines, Monsieur le Ministre pour examiner votre projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Son article 2 propose d'ailleurs de nouvelles modalités de contrôle pour l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Alors évidemment il m'est impossible car il s'agit du même objectif de ne pas aborder ici les derniers travaux de la délégation des droits des femmes dont j'ai été coauteur du rapport porno l'enfer du décor qui a tant fait parler de lui depuis un an maintenant, là aussi ce travail visait à éveiller les consciences sur les dérives de l'industrie et sur les conséquences sur les plus fragiles avec une trentaine de propositions et je remercie d'ailleurs Madame la Ministre et Monsieur le Ministre de l'avoir rappelé dans vos propos liminaire et d'avoir tenu compte de nos préoccupations visant à protéger les mineurs des sites pornographiques. Aujourd'hui il est temps pour le Sénat de franchir donc une nouvelle étape cette proposition de loi ne prétend pas résoudre en quelques articles l'ensemble des conséquences néfastes de l'utilisation des réseaux sociaux sur les moins de 15 ans mais l'une Pierre de plus à la construction d'un véritable écosystème global de protection de l'enfance aligne moins d'expo précoce à la violence des réseaux sociaux. C'est moins de risque de cyber harcèlement moins d'Exposition au cyber. Violences sexistes et sexuelles et moi d'accès à la désinformation, je vous rappelle que la théorie de la Terre plate. D'ailleurs récemment sur les réseaux sociaux a séduit un jeune sur six et puis c'est aussi une question de santé publique qui ne dit pas son nom. L'adoption non de cette proposition de loi à l'heure où les pays du monde entier et singulièrement l'Europe s'attache enfin imposer un cadre constituerait un signal fort pour conclure, mes chers collègues. Ce texte qui acte la prise de conscience du Sénat du caractère urgent et impérieux de construire un cadre juridique solide permettra de mettre chacun face à ses obligations à ses obligations et à ses responsabilités. Nous ne pouvons plus nous contenter d'observer les potentiels dommages nous devons poser des garde-fous indispensables à leur protection et je suis convaincu que cet enjeu peut nous rassembler. Et je vous remercie d'ores et déjà pour les propositions d'amélioration du texte porté par vos amendements. Merci madame la rapporteur. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Thomas Dossus du groupe écologiste pour cinq minutes. Madame la présidente madame la rapporteure Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons très d'une question essentielle, la place des mineurs dans le monde numérique. Ce n'est pas la première fois que le Sénat se penche sur cette thématique, la proposition de loi vite en visant à lutter contre le cyber-harcèlement. La commission d'enquête sur l'usage de TikTok. La proposition de loi protégeant le droit à l'image des mineurs en ligne notre agenda législatif hé bien occupé par la question. Qu'est-ce qui différencie ce texte proposé par le président du groupe horizons. À l'Assemblée nationale de tous les textes précédemment cité. Il s'agit ici de réguler la présence de mineurs au sein de l'espace numérique dans lesquels ils peuvent être particulièrement vulnérables, les plateformes des réseaux sociaux. Pour ce faire et comme son nom l'indique, cette proposition de loi fixe une majorité numérique à 15 ans en dessous de laquelle l'accord parental est indispensable pour l'inscription à un réseau social. C'est le coeur du dispositif, ce texte propose d'inscrire pour la première fois dans la loi une définition juridique des réseaux sociaux, reprenant celle du DMA européen corriger bientôt, je l'espère avec l'amendement qui en exclut Wikipédia par exemple c'est un pas en avant pour le législateur. Il propose également d'obliger les opérateurs de réseaux sociaux à diffuser des messages de prévention contre le harcèlement, ça ne mange pas de pain ou de fixer un cadre plus contraignant dans lequel les opérateurs de plateforme en ligne doivent répondre aux réquisitions judiciaires dans le cas d'une enquête préliminaire ou de flagrance. Toutes ces propositions ont été affinées enrichies par la navette parlementaire et aboutissent au final un texte qui va évidemment dans le bon sens. J'aurais pu arrêter ici mon intervention remercier notre rapporteur pour son excellent travail et annoncé le vote pour des écologistes sur ce texte, je vous rassure, c'est ce que je compte faire dans quelques minutes mais ce texte pose encore quelques petits problèmes puisqu'il est très floue en réalité sur sa mise en oeuvre. C'est d'autant plus ennuyeux, car cela concerne la mesure phare de cette proposition de loi en effet comment contrôler effectivement l'âge des personnes qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Cette PPL trouve une solution qui en réalité n'en est pas une, ce sera l'Arcom après consultation de la CNIL de définir un référentiel auxquelles devront se plier les plateformes, en un mot on laisse l'Arcom se débrouiller pour mettre en oeuvre une solution dite technique qui à l'heure n'est à l'heure actuelle n'existe pas. Cela fait plusieurs années hé bien avant cette proposition de loi que la CNIL s'est penché sur la question de la vérification de l'âge. Voici ce qu'elle disait. S'agissant de la vérification de l'âge les dispositifs existants ou envisagés sont généralement hein satisfaisant à 2 titres certains repose sur une collecte massive de données personnelles et apparaissent dès lors difficilement conforme aux principes de protection des données, d'autres moins intrusif sont cependant inefficace parce que trop aisément contournées par les mineurs par exemple le système déclaratif. Ainsi, les experts, ceux-là mêmes qui devront élaborer ce fameux référentiel de l'article de de ce texte reconnaissent leur incapacité ou ou le flou. Juridique pour le faire dès lors j'estime que le texte que nous examinons aujourd'hui relève quelque part d'un voeu pieux de la pensée magique une croyance selon laquelle demain peut-être nous serons à même de résoudre un problème quasi aussi vieux qu'Internet mais dans ce cas pourquoi légiférer maintenant pourquoi décharger le législateur de sa responsabilité à trouver une solution car cette solution n'est pas uniquement technique comme l'expose la CNIL entre les lignes, elle est éminemment politique. La solution qui sera peut être trouvée mobilise des sujets aussi importants que l'anonymat sur Internet la protection des données. Le rôle des, des algorithmes dans la vie de la cité, la place des géants du Net dans la mise en oeuvre de la majorité numérique, la protection des enfants. Face Face aux contenus violents et ne ou pornographiques. Toutes ces questions sont trop importantes pour que le législateur sont dessaisissent avec il faut le dire, un peu d'hypocrisie. Je pense que tout le monde sur ces bancs, on est bien conscient de ce problème. C'est à mon avis une des raisons pour laquelle l'article 6 de la proposition de loi repousse la mise en oeuvre des dispositions du texte. Toutefois. Au vu d'autres, des autres avancées du texte parce que celui-ci ne comporte pas de mesures que nous jugeons néfastes parce qu'il faut parce qu'il peut aider et ça a été dit les familles à accompagner leurs enfants à dialoguer avec leurs enfants dans leur découverte du numérique et comme convenu. Précédemment pour reconnaître le travail et la qualité de notre rapporteur les écologistes voteront pour cette proposition de loi. Merci la parole est à présent à monsieur Julien Bargeton du groupe RDPI pour six minutes, chers collègues.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président Madame la rapporteure. Alors en effet, le numérique a ouvert et Nantes possibilité et en même temps a ouvert tous les dangers et notamment pour les jeunes et c'est vrai que les conséquences de l'utilisation du numérique par les jeunes c'est hé bien une Exposition accrue aux risques. Ça a été dit 82%. Des enfants. De 10 14 ans vont sur internet. En l'absence de leurs parents. Et c'est 95% d'ailleurs pour les adolescents sur les réseaux sociaux. Donc il y a un usage massif. Des réseaux sociaux par les jeunes, l'âge de la première inscription en moyenne c'est 8 ans et demi les conséquences. Les conséquences possibles de de ses usages. Évidemment ça va en lien avec certaines pratiques, une progression des jeux vidéo au détriment. Par exemple, de l'échange des des devoirs ou des cours. Cela a été accrue en particulier. Par le confinement et cela n'a pas cessé. Depuis. Et donc en effet, on le voit par exemple. TikTok est massivement utilisé pas que par les jeunes hein d'ailleurs puisque TikTok en trois ans s'est passé de 4 millions à 15 millions et il y a 20 millions et donc. Évidemment, à peu près 60% des jeunes utilisent un réseau social et notamment son son sur TikTok. Donc on le voit. Que cette cette massification. bon usage numérique par les jeunes. A une conséquence, c'est évidemment la maximisation des risques alors. Quels sont ses risques. Ils ont été cités risque de dépendance liée aux algorithmes les risque de tomber sur des mauvaises rencontre des prédateurs ou des vendeurs de drogue risque d'isolement risque de baisse d'estime de soi. et risque bien sûr d'une sédentarité accrue. Voilà. La plupart des dangers qui sont désormais bien bien connu sur sur le numérique. les conditions se sont accrues pour contrôler l'âge récemment mais c'est vrai que ça a été signalé. Il faut encore pouvoir s'assurer de la vérification réel de. De, de l'âge par les opérateurs. On voit qu'il y a quand même eu des avancées, notamment en matière par exemple de jeux en ligne qui aujourd'hui sont beaucoup mieux protégés. En revanche, c'est le cas notamment pour l'accès aux sites pornographiques, où il y a encore un effort à faire dans la réalité de la vérification de la condition de l'âge alors un certain nombre d'études Ses, ses conséquences, je pense à une étude récente de la fondation Jean Jaurès. Qui indique qu'une Exposition plus grande aux réseaux sociaux induit une croyance dans. Des thèses complotistes ou anti-sont scientifique hein. 33% des jeunes seulement estime que la science apporte plus de bien que de mal, c'était 55% en 1972 et c'est le cas pour 82%, la croyance à des De donner nom scientifique notamment par exemple sur. Le climato-scepticisme. Eh bien, de 82% pour des jeunes qui utilise très très fréquemment les réseaux sociaux et c'est plus faible pour ceux qui les utilisent moins cette cette étude de la Fondation Jean-Jaurès le montre bien. D'autres études montrent évidemment que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a en réalité un isolement social perçu plus grand avec l'utilisation des réseaux sociaux. Alors quand même, c'est un peu contre-intuitif. D'autres études montrent également que il y a effectivement un effet proche de ce qui existe par exemple en matière de machines à sous, hein, c'est-à-dire ce mécanisme psychologique bien connu qui fait appel à la dopamine en fait et qui est liée aux algorithmes parce c'est le même fonctionnement psychologique et puis. Enfin je je revenir vient pas parce que ça a été largement. Largement cités mais également les le cas des normes hein le fait que. L'utilisation des réseaux sociaux impose finalement les mêmes normes, et donc ça peut entraîner évidemment des effets de comparaison négatif. cette ce texte s'inscrit dans. Une série de textes que nous avons déjà pris. Sur sur ces sujets, je pense bien sûr à l'encadrement de l'utilisation des téléphones dans les établissements scolaires Je pense également aux textes sur les le travail des enfants influenceurs. Je pense également aux textes en cours sur l'image des enfants la CMP a été. Je crois, s'est tenu le 11 mai. Je pense également bien sûr aux textes sur le cyber harcèlement c'est-à-dire comment le harcèlement harcèlement scolaire peut finalement prendre une dimension de cyberharcèlement, avec la possibilité, notamment de confisquer les appareils qui ont servi au cyber, harcèlement, on voit qu'il y a déjà eu donc donc 4 textes qui précède ce texte sur la majorité numérique, hé bien qu'vont être complété par votre texte monsieur le Ministre, notamment sur la sécurisation de l'espace numérique il y a donc, étape par étape jalon après Jâlons, une consolidation de l'encadrement de l'utilisation du numérique par les jeunes car si cela a suscité un formidable espoir au moment de la création d'Internet et également au moment de la création des réseaux sociaux, on voit toutes les conséquences négatives. Il faut donc qu'on aboutisse à un 3ème temps après le temps de l'espoir et et celui finalement des dangers, des risques doit venir celui du temps d'un Internet régulé apaisé et notamment au bénéfice de nos jeunes. Merci beaucoup. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur David Assouline du groupe socialiste pour 9 minutes,

Les sujets concernant la haine en ligne et les problématiques en particulier autour de la jeunesse et des réseaux sociaux ont toujours été. Au coeur des combats, du groupe socialiste, écologiste et républicain pour lequel je parle. J'avais été rapporteur dès 2008 d'une mission sur ce sujet et j'avais voulu intituler mon rapport. Nouveaux médias, les jeunes libérés ou abandonnés. Je pense que la problématique était déjà mises sur la table puisque c'était l'époque où on voyait tous les bienfaits du Net et on avait tendance à plus parler de libération. Et pas se rendre compte que pour les enfants et pour les jeunes, c'était aussi un moyen. Presque d'abandon des jeunes de la part de tout ce qui les éduquent les parents et l'éducation nationale. visant à instaurer une majorité numérique qui a lutté contre la haine en ligne va dans le bon sens en effet quand nous regardons les chiffres. La situation est toujours plus inquiétante. Il est donc grand temps d'agir encore plus vite et plus fort. Vous le savez, les enfants sont massivement connectés aux réseaux sociaux et s'y inscrivent de plus en plus tôt. Ça a été dit. D'après une enquête de la CNIL de 2021 la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi et plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient présents sur ces plateformes. Ces données sont confirmées par une enquête de l'association Génération numérique selon laquelle en 2021 63 % des moins de 13 ans avait un compte sur au moins un réseau social alors même que ces réseaux leur sont en théorie interdites du fait de leurs conditions générales d'utilisation. Parallèlement. Les parents supervise peu ou pas. Les activités en ligne de leurs enfants. À peine plus de 50% des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 80% déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font en ligne ce qui. N'a presque pas bougé depuis 2008. Quand je faisais mon rapport l'Exposition à internet et aux réseaux sociaux des plus jeunes peut avoir des conséquences telles que l'addiction aux écrans. Problèmes de sommeil, trouble de l'humeur, donc c'était de dépression risque de désinformation ou d'Exposition à des contenus pornographiques. Tout cela a été dit ou haineux ou encore cyber harcèlement véritable fléau pour notre jeunesse. L'anarchie libérale j'ose dire sur le Net qui existe actuellement est une trop faible régulation des plateformes sont un danger car leur seul but est le plus de profit et les enfants sont des proies faciles pour ces entreprises, comme vous le savez, l'exemple le plus criant et qui est sur le devant de la scène depuis plusieurs années et TikTok. Ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'une commission d'enquête a été créé ici même au Sénat pour comprendre en profondeur les risques liés à cet acteur chinois qui inquiète. Il faut davantage de contrôle sur la consommation des médias sociaux par nos plus jeunes. Il était donc grand temps. D'avancer sur ce sujet déjà des choses réalisées réalisés précédemment. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Son article 6, qui vise à imposer aux acteurs. Du secteur à lutter compta diffusion d'apologie des crimes contre l'humanité de l'incitation à la haine raciale, ainsi que de la pornographie enfantine. Il y a eu à travers la loi Avia, puis en 2020 puis. Celle sur le séparatisme des. Tentatives et des avancées mais à côté de choses beaucoup plus contestée et. On peut dire que le texte dont nous parlons aujourd'hui, suit une logique de tendance à plus d'encadrement de la haine en ligne mais aussi. Cette volonté. Que vous avez 2 actualiser la réglementation de la majorité numérique présente. Dans celle de 2004. Ces nouvelles réglementations pourront compléter les dispositifs déjà existants, mais qui sont encore trop insuffisants pour protéger les enfants en ligne comme le contrôle parental par défaut sur les appareils vendus en France en mars 2022. Cette proposition de loi souhaite aussi donner une définition concrète des réseaux sociaux cette définition reprend celle figurant dans la législation européenne sur les marchés numériques au DMA. C'est une bonne chose. Par ailleurs, notre groupe souhaite à travers un amendement excluant les encyclopédie en ligne. Wikipédia à but non lucratif de la définition des réseaux sociaux, à l'instar du choix opéré par la directive européenne. Ce texte souhaite également contraint des réseaux sociaux a refusé l'inscription à leur service des enfants de moins de 15 ans, sauf si les parents ont donné leur accord pour ce faire, ces plateformes devront mettre en place une solution technique permettant de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'autorisation des parents. En toute logique, ce sera l'Arcom qui sera chargée de certifier ses solutions techniques qui devront être conformes à un référentiel qu'elle aura élaboré après consultation de la CNIL en cas de non respect de cette obligation. Le réseau social pourra se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial des solutions de contrôle de l'âge en ligne existe, mais aucune n'est appliquée de façon satisfaisante, il est nécessaire de progresser sur cet enjeu important, notamment concernant l'accessibilité des sites pornographiques pour les mineurs. Des évolutions adopté par l'Assemblée nationale ont amélioré le texte avec notamment la possibilité de permettre aux parents. De demander la suspension sur un réseau social du compte de leur enfant de moins de 15 ans d'obliger les réseaux sociaux à diffuser des messages de prévention contre le harcèlement et a indiqué le numéro. 30 18, numéro Vert pour lutter contre le cyberharcèlement ou encore d'étendre la liste des contenus illicites, que les utilisateurs peuvent signaler aux réseaux sociaux, afin qu'ils soient retirés. Toutefois, ce même texte modifié par l'autre chambre et la commission culture, de l'éducation du Sénat ne va pas assez loin en effet déjà dans le rapport que je faisais en 2008 j'insisté sur la nécessité d'instaurer une ambitieuse éducation aux médias et aux réseaux sociaux afin de les sensibiliser sur les enjeux parce qu'il y a la répression des raisons mais on sait très bien qu'il faut aider les enfants à se protéger eux-mêmes et que ça passe par l'éducation parmi les recommandations il y avait déjà le renforcement des messages de prévention sur les plateformes de blogs et les sites communautaires, le lancement d'une étude de grande ampleur relative à l'impact de la publicité sur la jeunesse et le renforcement du rôle des professeurs documentaliste dans l'éducation. Je proposais également l'utilisation des nouveaux médias. Que cette utilisation soit le support pédagogique prioritaire dans les cours d'éducation civique, ce qui permettait de joindre le fond à la forme. De cette utilisation, la mise en place d'un maudit de 10h annuelles d'éducation aux médias en quatrième et en seconde, ou encore le renforcement des obligations de l'audiovisuel public en matière de programmation d'émissions de décryptage des médias et des nouveaux médias. Je déplore que beaucoup de ces propositions n'aient pas été mises en oeuvre depuis ou ont parfois peu avancé ou alors ont été intégrées au code de l'éducation sans donner les moyens. Ensuite, que ce soit une réalité vécue par l'ensemble de la jeunesse dans l'éducation nationale, il faudra continuer à avancer là-dessus je. Veux souligner en ce qui concerne le cyber harcèlement que l'article 1er Terre est une des recommandations de la mission d'information de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement que ma collègue Sabine vendent elle a présidé, c'est une bonne chose. Rappeler que nous sommes également favorables à l'article 5, il ne faut pas fusionner le 30 18 le 30 20 qui ont été des spécificités des utilités différentes qu'il ne faudrait pas fragiliser pour ce texte, nous avons déposé plusieurs amendements, nous allons les développer en séance, donc je ne vais pas les développer ici, à la tribune mais en général ces amendements visent à faire que le texte prenne en compte les recommandations du rapport de Sylvie Robert au nom de la CNIL, qui est un rapport de la CNIL et nous voulons avancer dans cette direction. Ce texte va donc dans la bonne direction mais il y a encore du chemin à réaliser une prochaine loi numérique va arriver ce sera encore l'occasion plus généralement d'aborder bien entendu ce sujet pour protéger les enfants des dérives sur les réseaux sociaux. Merci la parole est à présent à notre collègue Monsieur Jérémy Bacchi. Au nom du groupe communiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui à débat d'un sujet majeur, celui de l'accès. Ainsi que de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux par les mineurs, nous savons l'accès des plus jeunes à Internet est devenu une tendance lourde, ça a été dit la première inscription à un réseau social intervenait à moyenne vers huit ans et demi et plus d'un quart des 7 10 ans se rendrait régulièrement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font donc partie du quotidien de nos enfants, de nos adolescents. Tandis que le risque d'addiction Guy et à leur consommation et irréfléchie méticuleusement organisée par des multinationales, de ses usages sont nombreux naturellement le 1er qui vient à l'esprit et qui fait d'ailleurs l'objet de cette proposition de loi, c'est le cyber harcèlement, selon une étude datant de novembre 2022 près de 60% des enfants et adolescents déclarent avoir été victimes de cyber harcèlement peut laisser des séquelles conduire à la dépression voire à des conduites suicidaires. Lorsque l'on sait que le suicide représente 16% des décès chez les jeunes et qu'un enfant cyber harcelé sur deux il y a déjà songé. Il est clair que nous sommes face à un enjeu national de santé publique. Plus largement, cet accès précoce à Internet induit également un risque d'une modification de l'image de soi, d'uniformisation, ainsi qu'un risque ça a été dit là aussi d'Exposition à des sites à caractère sexuel ou encore des sites idéologique à caractère raciste, antisémite ou homophobe. L'ampleur de ces phénomènes est attestée par plusieurs études utilisés à bon escient. Il est indéniable que ces plateformes permettent d'acquérir des connaissances en revanche, elles peuvent également mener à l'intériorisation pardon de stéréotypes et exposé à des contenus violents. Aujourd'hui, il existe un gouffre entre les obligations réglementaires des plateformes et la réalité pratique sur le terrain, en effet, alors même qu'il existe un âge minimum requis pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. C'est plus de la moitié des enfants de moins de 13 ans qui sont déjà inscrits sur un réseau social. une précocité croissante dans l'accès aux smartphones exposants également de fait les enfants aux dérives de ces technologies. Le constat est double, d'une part la responsabilité des entreprises propriétaires des réseaux sociaux apparaît clairement et il serait temps de les encadrer plus fermement pour qu'elle respecte les dispositions qui les concernent. Cette situation nous oblige à nous parlementaires à élaborer des lois mettant en sécurité nos jeunes et nos mais ne doivent pas tremblé quand tu la possibilité que celle-ci suffisent. Pardon. 30 quant de la possibilité que celles-ci soient suffisamment exigeante et contraignantes pour que les plateformes mettent un arsenal de mesures pour réduire au maximum les risques de nos mineurs d'autre part, il est nécessaire que nous accompagnons davantage les enfants dans leur usage d'Internet mais aussi les parents dans l'accès. De leurs enfants à Internet par des outils de prévention. C'est pour cette raison que nous sommes favorables à l'instauration d'une majorité numérique à l'âge de 15 ans. Cette disposition étant d'ailleurs conforme à la législation européenne et aux recommandations de la CNIL. L'instauration d'une telle mesure aura le mérite d'inciter aussi le dialogue entre les parents et les enfants sur les usages du numérique. En ce qui concerne la question proprement techniques de la mise en place du contrôle de l'âge faites par les plateformes nous devrons rester vigilants quant à la protection des données requises pour cette vérification. Par ailleurs, il est également prévu de faciliter les demandes d'information auprès des plateformes dans le cadre d'une réquisition judiciaire dans un délai de 8h pour les cas urgents et de 10 jours pour les autres cas afin de livrer toute information utile dans le cadre de l'enquête, même si nous aurions préféré un délai plus long Plus court pardon que les 10 jours. Pourquoi pas 48 heures au regard des possibles conséquences gravissimes que peuvent engendrer la lenteur des procédures, nous considérons que la sanction permettant de s'assurer que les plateformes respectent cette disposition n'est malheureusement pas tout à fait en adéquation avec le poids économique de ces grandes entreprises, il s'agit d'un manque notable de cette proposition de loi alors même qu'à l'origine, il était prévu un maximum d'un pour 100 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. De plus nous souscrivons pleinement à la demande de rapport inscrit à l'article IV de cette proposition de loi puisque celui-ci permettra. De gagner en efficacité par un apport de connaissances sur les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur les jeunes. Toutefois, nous resterons vigilants à ce que la fusion des plateformes d'appel destiné aux victimes de harcèlement scolaire et de harcèlement en ligne mise en place par l'article 5 ne soit pas synonyme d'une baisse de moyens global à ces dispositifs de prévention indispensable. Dans l'aide aux victimes, vous l'aurez compris, mes chers collègues. Malgré quelques points de vigilance dont j'ai eu l'occasion de parler lors de cette intervention. Nous considérons que cette proposition de loi suit une constitue une première étape dans un contrôle à l'accès d'Internet pour nos plus jeunes et c'est dans cet état d'esprit qu'avec mon groupe nous voterons favorablement à ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Jean hein xer du groupe Union centriste pour 4 minutes.

madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tenais tout d'abord, et nous tenions. Le groupe centriste, né à à vous féliciter madame la rapporteure pour cette proposition de loi dont nous entamons l'examen le numérique. L'Internet les réseaux sociaux, les tablettes, les smartphones ont pris une place centrale dans la vie des enfants et des adolescents. Je ne reviendrai pas trop longuement sur l'impact extrêmement inquiétant que ces nouvelles technologies parfois utile on sur notre jeunesse. Notre rapporteur que je félicite au passage pour l'excellence de son travail. On a déjà fait un bilan pour le moins éclairant, 60% des jeunes âgés de 11 à 18 ans sont inscrits sur au moins un réseau social. Ces inscriptions interviennent de plus en plus tôt. 80% des parents déclarent ne pas savoir ce que font leurs enfants en ligne. Concernant ce dernier chiffre en commission l'une de nos collègue faisait remarquer qu'il y a surtout 20% des parents qui ne savent pas. Qui ne savent pas ce que leurs enfants font en ligne j'ai malheureusement trouvé cette réflexion frappée au coin du bon sens. Nous le savons depuis longtemps. Il faut protéger les mineurs de l'ensemble des dangers auxquels le numérique les exposent et ils sont nombreux, telle est l'objet de ce texte, dont la proposition centrale est double, d'une part obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge du des utilisateurs et d'autre part, garantir le consentement des titulaires de l'autorité parentale, pour les moins de 15 ans. Ce texte est d'autant plus partisans, qu'il a été simplifié en commission. L'Assemblée nationale avait en effet prévu un dispositif plus compliqué entre 13 et 15 ans, les jeunes n'aurait pu avec le consentement de leurs parents s'inscrire que sur des sites labellisés. On comprend l'intention, elle est louable mais cela soulever encore trop d'interrogations. Qui la abbé liseré sur quels critères. C'est pourquoi nous pensons que notre commission de la culture a bien fait de supprimer ce dispositif. Le présent texte fait écho aux travaux de notre collègue Annick Billon sur la protection des mineurs contre la pornographie en ligne dont elle dira un mot dans quelques instants. Il fait aussi écho très au travail depuis fort longtemps de notre collègue Catherine Morin-Desailly qui militent pour une régulation des plateformes et c'est bien là le nerf de la guerre. Mais c'est aussi là que le bât blesse en commission la proposition de loi majorité numérique haine en ligne a été presque unanimement plébiscitée. Mais dans le même temps, tout le monde reconnaissait que si l'on ne contraint contraint pas les plateformes à l'accompagner à jouer le jeu. Ce que nous sommes en train de faire pourrait avoir tout d'un acte performatif un geste aussi beau et politique que platonique. Tout le monde sait que proclamer des principes sans être capable de les faire appliquer ne servirait à rien. Heureusement, les choses semblent enfin évoluer dans le sens d'une véritable régulation des plateformes. Au niveau européen d'abord avec le Digital Service Act qui renforcera la responsabilité des plateformes sur les politiques de modération des contenus mis en ligne et le Digital Markets Act qui rééquilibrera les relations entre les plateformes et les entreprises qui recourent à leurs services. Et bien sûr ensuite au niveau national avec le futur projet de loi sereine qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique pour permettre. Pour mettre en oeuvre. Oh pardon. Ces principes au mieux et au plus vite. Vous l'aurez compris. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le groupe Union centriste votera la présente, proposition de loi en ayant en ligne de mire, l'examen du texte Rennes qui lui donnera tous les moyens de réussir et de se concrétiser. Je vous remercie. Madame la présidente. Madame, monsieur les ministres, madame le rapporteur. Mes chers collègues. Si la petite poussette de Michel Serres a la chance d'avoir au bout de ses doigts l'accès à l'ensemble des données universelles répertoriés dans les encyclopédies. Gratuitement. Nous savons que les enfants ont aussi entre les mains en risque élevé d'addiction aux réseaux sociaux qui leur colle au doigt. Le caractère addictif des réseaux sociaux accentuée par une course effrénée à l'engagement est un danser. J'ai pour la santé et la société. Sans régulation. Les algorithmes augmente l'emprise sur le cerveau des enfants contre laquelle les parents ne peuvent pas toujours lutté. Les chiffres sont là. Selon la CNIL. 82% des 10 14 ans consultent Internet sans leurs parents et 46% des 6 10 ans disposent de leur propre smartphone selon selon et La consultation de contenus inappropriés par les enfants et les jeunes adolescents à de lourdes conséquences psychologiques et sociales allant de l'addiction au suicide comme on l'a dit, en passant par une baisse de l'estime de soi. Il y a des on pas raison avec des influenceurs des mauvaises rencontres ou du cyber harcèlement. Pour toutes ces raisons, la régulation des réseaux sociaux est nécessaire et urgente. À ce titre j'avais déposé un amendement prévoyant que les réseaux sociaux affiche un message d'avertissement sur les conséquences néfastes que peut engendrer leur utilisation sur la santé physique et mentale. Cette proposition de loi ne vise ni à punir les plus jeunes ni à provoquer des relations conflictuelles avec les parents. Au contraire. Elle aspirent à remettre le parent au coeur de la relation entre le mineur et l'outil Nîmes numérique. Ce texte constitue une avancée en matière de protection numérique. Il s'inscrit dans la lignée de l'article 8 du règlement général de l'Union européenne relatif à la protection des données, lequel fixe déjà l'âge de 15 ans pour consentir au traitement de ces données personnelles. Ainsi, en prévoyant une autorisation parentale pour l'inscription d'un mineur de moins de 15 ans sur un réseau social la présente proposition prolonge et améliore le RGPD. Toutefois, le numérique est une technologie en telle évolution que le 100% n'existe pas. Et caché derrière son écran la tentation de jouer avec les règles et grande. En ce sens. Il faut, sur la base d'un référentiel élaboré par l'Arcom et la CNIL à mettre en place un outil technique permettant de contrôler l'âge des inscrits et des futurs inscrits. Aucune solution technique ne répond à ce jour à ce défi à l'échelle de la population. Toutefois, nous pouvons espérer dans des initiatives telles que eux-consente par exemple soutenue par la Commission européenne. Les réseaux sociaux doivent aussi prendre leur part dans la lutte contre la haine et les dérives en ligne. Ils doivent empêcher la consultation de contenus inappropriés au moyen de leurs algorithmes. Qui savent déjà très bien orienté leur contenu vers des publics ciblés. S'il ne joue pas le jeu de la collaboration et de la prévention. Les pouvoirs publics seront en mesure de prononcer des sanctions dissuasives sur leur chiffre d'affaires mondial. Cette proposition vise à lutter contre toutes les formes de haine en ligne. En ce sens. Elle n'ignore pas le cyber Arte seulement. Un fléau qui touche plus d'un million d'élèves chaque année. Aussi. Si la mise en place des numéros 38, 20 et 38 18 va dans le bon sens. Il sera à mon avis plus simple et plus efficace de ne proposer qu'un seul numéro bien repérable parce qu'on sait qu'ils sont difficilement. Repéré et qui orienterait le jeune vers un standard unique. Lequel pourrait orienter vers l'entité. Compétente. Parce que les deux ça ne doit laisser aucun enfant Sol en détresse et apeuré derrière son écran. Le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition.

Madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi du député Laurent Marcangeli, dont l'objectif est de mieux encadrer l'usage des réseaux sociaux pour nos jeunes en instaurant une majorité numérique à 15 ans et lutter contre la haine en ligne. En effet nous constatons chaque jour certains effets délétères et toxique que peuvent provoquer les plateformes de réseau social sur les enfants et les adolescents avec des expositions à des contenus inadaptés. Vous l'avez dit, monsieur le Ministre. Le défi à relever est de taille. Il suffit de lire les différents chiffres cités dans le rapport de notre collègue. Alexandra Borchio-Fontimp, dont je salue l'excellent travail. 82% des 14 des 10 14 ans consultent Internet sont leurs parents, 46% des 6 10 ans disposent. De leurs propres smartphones. 28% d'entre eux se rendent régulièrement sur un réseau social 60% dès 11 18 ans se réinscrit sur TikTok. Ces chiffres sont alarmants et cachent parfois des situations particulièrement inquiétante, dépression, anxiété sédentarité isolement isolement troubles du sommeil de l'humeur et de la mémoire ou encore cyber harcèlement. La CNIL rappelle ainsi que 6% des collégiens serait harcelé jusque dans leurs chambres via leur smartphone ou les réseaux sociaux, ce sont 6% de trop. De leur côté les parents ignorent ou n'ont pas toujours les moyens ni le temps pour superviser la vie numérique de leurs enfants. Ces derniers sont pourtant très vulnérables. Face aux stratégies commerciales de plus en plus agressive et ciblée des plateformes qui sur sollicitent leur attention. Dans ce contexte, la régulation de l'accès Internet pour nos jeunes constituent un véritable enjeu de santé publique. Le texte de monsieur Marcangeli tente d'y apporter une réponse en fixant un âge à 15 ans, en dessous duquel les mineurs aura besoin du consentement de l'un de ses parents pour s'inscrire sur un quelconque réseau social cette borne doit à la fois servir de boussole pour les parents et obliger les réseaux sociaux à repousser l'âge d'entrée est fixé jusqu'à présent à 13 ans. Le but est d'envoyer un signal fort au moment où certains de nos voisins européens encadre plus strictement l'usage des outils numériques. Ce texte contribue également à restaurer l'autorité parentale. La remise d'un rapport du gouvernement au Parlement permettra par ailleurs de mieux évaluer l'impact des réseaux sociaux sur le développement cognitive de nos enfants et adolescents cela contribuera aussi à animer un débat public sur ce sujet de société. Du point de vue technique ce texte incite vivement les plateformes a contribué à l'encadrement de l'usage des réseaux sociaux pour les mineurs en développant des solutions technologiques permettant d'identifier l'âge de la personne s'inscrivant un réseau social et de recueillir l'accord de l'un des deux parents. Il s'agit aussi pour elle de respecter plus rigoureusement le cadre national et européen sur la protection des données personnelles des mineurs, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se leurrer, la mise en oeuvre de cette proposition de loi sera complexe et longue. Il faudra compter sur la bonne volonté des plateformes. Si la perspective des sanctions devraient aider à avancer assez rapidement la rapporteure a tout de même souhaité rend le texte plus opérationnel. Par le biais de précision technique bienvenue. Concernant les conditions de la majorité numérique l'accord d'un seul des titulaires. De l'autorité parentale suffira pour accepter l'inscription d'un mineur de 15 ans sur un réseau social. Un nouvel article décale également l'entrée en vigueur de la loi afin de respecter l'obligation de consultation de la Commission européenne et d'augmenter le délai permettant de travailler à des solutions techniques. Ainsi cette proposition de loi ambitieuse constitue une partie de la réponse aux enjeux de santé publique et de protection de l'enfance qui nous préoccupe tous, si elle est adoptée, ce que le groupe Les Républicains souhaitent elle devrait encore faire face à de nombreux obstacles. D'autres mesures sont en effet nécessaires pour préserver les mineurs des dérives d'internet, c'est d'ailleurs dans cet esprit que le Sénat s'est mobilisée en adoptant récemment la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérive des influenceurs sur les réseaux sociaux et également avec la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Mon groupe votera donc ce texte, car nous restons convaincus qu'exposer un enfant trop tôt aux écrans et Internet nuit à la construction sereine de sa personne et de son Intelligence. Il faut se donner les moyens d'agir avant qu'il ne soit trop tard et trouver les bons équilibres. Face aux nouvelles technologies du numérique. Je vous remercie. Merci cher que le collègue, la parole est à présent à monsieur Claude Malhuret du groupe les indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues. Nous connaissons tous désormais les dangers des réseaux sociaux pour nos enfants et nos adolescents. Accès au fait que News et au contenu violent Challenge dangereux. Et bien d'autres. Nous sommes bien loin des premiers réseaux qui permettait simplement de conserver des Liens entre famille et amis éloignés les uns des autres. L'utilisation de ces réseaux par des mineurs posent en réalité un double défi de protection de l'enfance et de santé publique. Des millions de jeunes Français les utilisent quotidiennement 55% des 10 14 ans possèdent au moins un compte selon la CNIL. En dessous de 13 ans, les enfants ne sont pourtant pas censé ouvrir un compte sur YouTube Snapchat Instagram TikTok discorde ou encore tu which. Or la première inscription intervient en moyenne vers huit ans et demi. Toujours selon la CNIL. Ces réseaux sont construits sur l'économie de la tension il capte nos données tandis que leurs algorithmes analyse en continu notre comportement en ligne afin de nous proposer du contenu ciblé c'est-à-dire en bon français addictif. Les internautes mineurs ne sont pas épargnés. Confrontés au fait News les plus farfelus et aux théories du complot les plus diverses. Les enfants ne savent pas toujours trier la surcharge d'information à laquelle ils sont exposés. L'IFOP nous apprend qu'un jeune Français sur 6 parmi les 11 24 ans pensent aujourd'hui possible que la Terre soit plate. Un sur 5 des 18 24 ans pensent que les pyramides égyptiennes ont été bâtis par des extraterrestres. Ne jeunes sont également confrontés à des contenus violents inapproprié et choquant, parfois sans le vouloir tout simplement parce que certains sites pour adultes ne verrouille pas l'accès à leur contenu. Il est loin le temps du vidéo club où il fallait passer le contrôle du vendeur pour louer une cassette aujourd'hui le contenu pornographique est accessible gratuitement, sans la moindre vérification d'âge. De millions de mineurs en France sont exposés chaque mois aux contenus pornographiques sur Internet vous l'avez dit tout à l'heure Monsieur le Ministre. Cet état de fait préoccupant nous alerte et doit nous engager à agir. Les réseaux sociaux permettent une liberté de ton et un anonymat qui n'existe pas dans le monde réel il favorise toutes les dérives et toutes les accès tuer toutes les excès comme l'avait souligné notre collègue Colette Mélot dans son rapport sur le harcèlement scolaire elle souligné qu'un enfant sur 10 est harcelé à l'école. Ce harcèlement est loin de se limiter à la cour de récréation, il se poursuit jour et nuit via les réseaux sociaux jusque dans l'intimité du domicile familial. De la même manière. Certains réseaux sociaux participent à l'hyper sexualisation des jeunes particulièrement des jeunes filles. D'autres permettent les échanges Directs de mineurs avec des adultes mal intentionnés tout cela. Pour des enfants qui n'ont parfois même pas atteint l'âge de 10 ans. Évidemment, cela ne peut durer. Permettre à nos enfants de naviguer sur Internet en toute quiétude représente un défi majeur. Cette proposition de loi est une première étape dans la réponse que nous y apporterons ce texte va foncièrement dans le bon sens. Je salue son auteur notre collègue le député Laurent Marcangeli pour son engagement sur ce sujet si important. Je remercie également notre rapporteur Alexandra Borchio-Fontimp de son travail attentif. Notre assemblée de se prononcer avec fermeté sur la question de la responsabilité des plateformes numériques. Dans le même sens lors de l'examen du projet de loi confortant les principes de la République. J'avais déposé un amendement visant à rendre les plateformes civilement et pénalement responsable des informations qu'elle stocke. Cet amendement adopté à l'unanimité au Sénat n'a pour le moment pas été présenté à l'Assemblée nationale et je le regrette. Imposer la mise en place effective d'une solution technique pour vérifier l'âge des utilisateurs et l'autorisation des parents est une avancée certaine. Je rappelle qu'il est également essentiel de sensibiliser les parents il y a des règles d'usages à respecter collectivement. Le nombre de textes relatifs aux enjeux du numérique et à la protection de l'enfance examiner ces derniers mois démontre une fois de plus l'engagement du Parlement sur ces questions. Je pense notamment à la proposition de loi visant à garantir le respect au droit à l'image des enfants ou encore au texte visant à lutter contre les dérive des influenceurs sur les réseaux sociaux. Nous pouvons nous en féliciter, c'est également le sens de la commission d'enquête sur l'utilisation de TikTok que je mène depuis plusieurs mois avec plusieurs de nos collègues. Le débat que nous avons aujourd'hui est essentielle. Au regard de l'immensité du défi d'un internet sûr sain et sécurisé pour nos enfants. Il se poursuivra dans les semaines à venir lors de l'examen du projet de loi sur le numérique dont nous a parlé en introduction à cette séance tout à l'heure le ministre de la transition numérique. Notre groupe les indépendants votera ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Enfin, la parole est donnée à madame la présidente Annick Billon du groupe Union centriste pour 4 minutes, chers collègues. Je n'avais Je n'avais pas l'impression d'être beaucoup plus petite que Claude Malhuret, mais a priori oui. Très bien, madame la présidente madame et monsieur les ministres me madame la rapporteure, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Madame la rapporteure Alexandra. Borchio-Fontimp pour la qualité de ses travaux pendant que nous débattons des jeunes collégiennes et collégiens font l'objet de harcèlement en ligne ou visionne des films pornographiques publie des chorégraphies et La législation européenne impose aux réseaux sociaux de fixer une majorité numérique comprise entre 13 et 16 ans en deçà de 13 ans, les enfants de doivent et ne devrait pas y avoir accès. Français des enfants français de 11 12 ans ont un compte sur au moins un réseau social. Ils ils publient du contenu régulièrement. Doit-on parler de défaillance ou de laxisme. La proposition de loi que nous examinons crée une majorité numérique fixée à 15 ans sous cet âge elle conditionne l'inscription sur les réseaux sociaux à une autorisation parentale. Malheureusement, il suffit d'un clic et d'une fraction de seconde pour transgresser l'interdit numérique et accéder à l'immensité des réseaux sociaux. Contourner l'accord parental est bien plus simple que de copier la signature d'un parent sur un mauvais devoir nous ne disposons actuellement pas des outils de contrôle nécessaires, ce qui met en échec l'intérêt parfois de l'accord parental et l'esprit déréglementation déjà existantes avec la rapporteure et aux côtés de Laurence Cohen et Laurence Rossignol. Dans le cadre d'un autre rapport sur l'industrie pornographique Porno l'enfer du décor. Nous avons formulé des recommandations dont certaines portent sur ses difficultés comme définir dans les lignes directrices de l'Arcom des critères exigeants d'évaluation des solutions techniques ou imposer le développement de dispositifs de vérification d'âge avec un système de double anonymat comme proposé avec le dispositif pérenne et Knin. L'appel du Sénat a été entendu par le gouvernement. En témoignent les premiers articles du projet de loi sur l'espace numérique que vous portez monsieur le Ministre, et qui reprennent. Avec une des améliorations. Une dizaine de nos recommandations sénatoriale au cours des derniers mois, plusieurs solutions de contrôle d'âge ont été évoquées, certaines sont en cours d'expérimentation et nous attendons résolument les premières conclusions. Gardons cependant à l'esprit que les dispositifs qui seront déployés pour les sites pornographiques ne seront pas pour autant facilement transposable aux réseaux sociaux du fait de la différence de l'âge minimum requis 18 ans pour les premiers 13 ans pour les seconds. D'autre part pour une réelle efficacité. Les mesures en faveur de la protection des mineurs doivent se penser c'est à l'échelle du réseau. À défaut, le recours à des dispositifs VPN permet déjà de contourner. La loi française. Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience générale et international du danger que peuvent représenter les réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes. Nous sommes face à un enjeu de santé publique, l'Exposition aux écrans et plus particulièrement aux réseaux sociaux, a des conséquences avérées sur la concentration, la diction, l'estime de soi, le rapport aux autres, la liste est longue. C'est pourquoi il y a urgence à combler les vides juridiques. Ce que nous faisons aujourd'hui mais aussi à mettre en oeuvre des dispositifs Il s'agit de protéger les enfants les futurs. Adultes, il est aussi question de protéger notre modèle de société. Nous devons tout tenter tout expérimenté pour enfin réussir à contrôler l'accès de la toile contrôler sanctionner éduquer former au numérique. Beaucoup de travail c'est un 1er pas merci. Madame la présidente madame la rapporteure chers Alexandra Madame. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. tout droit doit sans cesse s'adapter face au développement des pratiques sur Internet. Cela est parti mon vrai concernant le sujet de la protection des jeunes à peine voté la proposition de loi sur le respect du droit à l'image des enfants. Nous sommes de nouveau réunis ce soir pour légiférer sur l'accès aux réseaux sociaux. Or, l'évolution des technologies de caractère international de l'économie numérique rendent difficile la mise en oeuvre concrète des mesures que nous adoptons. À l'espèce nous sommes bien conscience. Des difficultés techniques qui se posent euros pour rendre effective l'interdiction d'accès des mineurs de 15 ans aux réseaux sociaux. Comment les plateformes pourront-elles s'assurer que l'âge communiqué hé bien l'âge effectif de la personne qui s'inscrit. S'il est établi que le l'usager. Eh bien, un mineur de 15 ans. Comment l'accord des parents sera-t-il recueilli les auditions ont montré que pour le moment les plateformes ne dispose pas des moyens techniques nécessaires pour autant soyons persuadés que si elles le souhaitent, elles seront en capacité de le faire. Alors pourquoi légiférer tout d'abord les des plateformes ont toutes évoqué des hypothèses de travail et des pistes prometteuses pour trouver des solutions technologiques. La proposition de loi les y incite fortement en engageant leur responsabilité et en prévoyant des sanctions ensuite ce texte marquer notre volonté politique d'édicter des règles pour l'usage des réseaux sociaux et la protection de nos jeunes et c'est ce qui est d'ailleurs dans une démarche générale des pays européens visant à donner un cadre à l'usage du numérique. La France ne doit pas avoir un temps de retard mais au contraire donner l'exemple. La protection des mineurs, a une longue histoire, notre pays et c'est son honneur. Elle doit désormais s'adapter à leur environnement numérique. Pour autant, je pense que la protection de nos jeunes doit aussi passer par d'autres actions notamment de prévention et que nous devons également inscrire dans notre droit, la place que les parents devraient être occupés dans le processus d'inscription sur les réseaux sociaux. Car les chiffres cités ce soir plusieurs fois sont édifiants. Les enfants sont massivement connectés aux réseaux sociaux et s'y inscrivent de plus en plus tôt, selon la CNIL, 82% des enfants de 10 à 14 ans, indique consulter régulièrement Internet sans leurs parents la première inscription sur les seaux sociaux intervient en moyenne vers huit ans et demi et plus du quart des 7 10 ans les étudie régulièrement le phénomène a été renforcé récemment par la crise sanitaire et les confinements successifs. Parallèlement, les parents supervise peu ou pas. Les activités en ligne de leurs enfants par méconnaissance mais également par un sentiment d'impuissance. Selon une enquête menée Paris enfance à peine plus de 50% des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 83% des ne pas savoir exactement ce que leurs enfants sont en ligne. Un nombre croissant d'études scientifiques attestent des risques induits par cette surexposition risque pour le développement des enfants pour leur construction sociale pour leur santé mais également risque de harcèlement et de cybercriminalité. Dans l'actualité nous rappelle qui peuvent conduire à des drames. Certes. L'expérience vécue sur internet de se résume heureusement pas à ces effets néfastes. Ce vaste. Il s'agit également de formidable outil de connaissance et de communication mais il nous faut constater que notre société se trouve confronté à un double défi de santé publique et de protection de l'enfance qui n'a pas été suffisamment anticipé le présent texte a le mérite d'impliquer les plateformes et de donner aux parents le cadre nécessaire pour mieux contrôler les usages de leurs enfants. Il permet par ailleurs d'intégrer enfin la définition européenne des réseaux sociaux. Diverses règles concernant la diffusion de messages de prévention et des numéros verts ou encore la procédure de réquisition judiciaire de contenus électronique. Le travail de notre rapporteure donc je tiens à saluer l'investissement sur cette PPL et au-delà sur la protection des mineurs dans l'environnement numérique, s'est attachée à rendre le texte C'est donc le texte abouti qui nous est proposé d'adopter aujourd'hui et notre rapporteur a décidé avec raison de lui laisser sa chance. Merci cher Alexandra pour que Fontaine pour votre engagement aussi, comme l'a dit, Guillaume Chevrollier, le groupe Les Républicains apportera son soutien à ce texte, tout en soulignant Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, que vos échanges avec les fournisseurs de services de réseaux sociaux seront essentielles pour le que le cadre fixé aujourd'hui devienne effectif en fait il. La balle est désormais dans leur camp et je suis persuadé, comme je le disais il y a un instant que s'ils le veulent vraiment, ils trouveront les moyens de donner du contenu à ce texte qui les y incite et c'est ainsi une bonne chose que nous faisons ce soir. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Cyrille pelle va du groupe les républicains pour 4 minutes. mais la présidente Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Depuis de trop nombreuses années. La législation française n'est pas à la hauteur des enjeux de santé publique et de protection de l'enfance qu'induisent l'utilisation d'Internet par des mineurs. Exposition à la haine en ligne et prolongement du harcèlement scolaire au sein même du foyer qui devrait pourtant être un refuge déformation de l'image de soi. Hausse des tendances suicidaires et des comportements addictifs risque de Revenge porn ou encore de prédation sexuelle, nombreux sont les impacts de dangers auxquels les enfants sont confrontés. Du fait de leur présence sur le Net et nous l'avons tous rappeler sur ces bancs. Certes le droit européen, a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans avec une possibilité laissée à la discrétion des États membres de porter l'âge minimal jusqu'à 16 ans. De même, nous avons légiféré afin d'acter l'obligation pour certaines plateformes de refuser aux mineurs de s'y inscrire ou de les consulter. Je pense notamment aux sites pornographiques. Mais le bât blesse. Concernant la vérification de l'âge des utilisateurs par les éditeurs, la plupart exige une simple déclaration sans aucun contrôle de sa véracité. Ce qui laisse toute latitude à l'internaute pour mentir demandé d'entrer des informations d'une carte bancaire ne suffit pas non plus puisqu'il est possible pour un enfant de obtenir une d'en obtenir une des 12 ans août utiliser celle de ses parents. De même la reconnaissance faciale présente des lacunes et le portefeuille européen d'identité numérique hein qui ambitionne de pouvoir identifier authentifier et vérifier des données telles que l'âge. Ou des documents officiels ni lui aussi pas encore au point. Faute de solution techniques éprouvées pour effet vérifier l'âge les plateformes ne respectent pas leurs obligations ne sont donc pas à ce jour, ils ne sont donc, à ce jour pas sanctionner. Ces derniers mois des avancées technologiques ont toutefois été constatés et une ou plusieurs solutions permettant d'obtenir un système de vérification satisfaisant et sécurisé devrait être trouvé un moyenne un moyenne voire courte échéance. Considérant ces avancées au regard de l'urgence qu'il y a un médecin fin à cette situation de non-droit au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant c'est ici contre Angers. La proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui. D'une part elle vient fixer une majorité dite numérique pour l'utilisation des réseaux sociaux là pourtant à l'âge de 15 ans. Les réseaux sociaux seront alors obligés de refuser l'inscription des utilisateurs n'ayant pas l'âge requis sauf accord Express de l'un des représentants les cours. D'autre part, il prévoit la création d'un référentiel par l'Arcom relatifs au système de vérification de l'âge. Des réseaux sociaux devront alors mettre en place une solution technique conforme à ce référentiel. En l'absence de vérification en cas de non-conformité l'Arcom pourra saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir une sanction à leur compte du réseau social. L'entrée en vigueur de cette possibilité de saisine de la justice est toutefois reporté un an dans le but de laisser le temps aux solutions techniques de se perfectionner. Ce compromis apparaît satisfaisant et je voterai donc à l'instar de mon groupe en faveur de cette proposition de loi. Mais je tiens toutefois à souligner qu'elle comporte et des angles morts. Le premier m'apparaît être la question des sites de rencontres. Ils sont des réseaux sociaux aux choses est la définition introduite par la proposition de loi, mais il me semble que la limite d'âge est ici inadapté. Certains sites de rencontre ont volontairement interdit l'accès à leurs services aux mineurs de 18 ans mais n'existera pas de sanctions pour celui qui donne accès au plus de 15 ans. La la question de l'accès aux mineurs à ce service peut être discutée mais je n'ai pas l'impression qu'elle a été posée. En outre, la proposition de loi se concentre sur les réseaux sociaux hors des services en ligne qui ne peuvent être qualifiés comme tel doivent eux aussi être interdits d'accès aux enfants de moins de 15 ans comme les sites de location de trottinettes électriques, voire des 18 ans pour les suites où il est possible d'acheter de l'alcool ou d'autres produits interdits aux mineurs de location de scooter ou de voitures les jeux d'argent en ligne et les sites pornographiques. Ces sites numériques qu'ils soient légalement obligé d'interdire l'accès ou qui l'interdisent de manière volontaire ne sont pas soumis à cette obligation de vérifier l'âge et de respecter le référentiel faut d'être qualifié comme des réseaux sociaux. Pour les sites pornographiques. Le projet de loi visant à sécuriser régulariser et régulé pardon l'espace numérique met en place une solution similaire au dispositif de la PPL n'a rien n'est prévu pour les autres services numériques. Je tiens donc à souligner pour conclure qu'il nous faudra être attentif à ces questions à l'avenir, je vous remercie. Merci cher collègue. La discussion générale est Close, nous passons à la discussion du texte de la commission article 1er une demande de prise de parole par notre collègue Madame Marie-. Pierre Monier. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous permet d'affirmer un principe sur lequel nous nous rejoignons toutes et tous, celui de l'accord préalable des parents pour l'inscription sur un réseau social pour les mineurs de moins de 15 ans. C'est un signal salutaire à l'heure où 46% des 6 disant disposent de leurs propres smartphone et au 28% des 7 10 ans se rendent régulièrement sur un réseau social. Il nous apparaît toutefois de façon aussi évidente que ce principe, une fois votée se heurtera à des difficultés pratiques dans sa mise en oeuvre. Mes collègues de la délégation aux droits des femmes qui ont travaillé pendant des mois dans le cadre de leur rapport porno l'enfer du décor sur la complexité d'interdire, conformément à ce qu'énonce l'article 227 tiré 24 du code pénal dont la première version remonte à 1994. Donc complexité d'interdire l'accès des mineurs à des contenus pornographiques pourront ainsi vous témoigner du gouffre entre l'intention du législateur et la réalité sur le terrain du numérique. Ainsi, si la loi du 30 juillet 2020 sur les victimes de violences conjugales, a rendu l'Arcom compétente pour intervenir auprès des sites qui ne vérifie pas la je leur utilisateur. Il a fallu attendre plus d'un an pour la publication du décret rendant opérationnel cette disposition sur le fondement de ce décret. Plusieurs sites pornographiques ont été effectivement mises en demeure par l'Arcom. Nous devons encore attendre pour 5 d'entre eux a signé pour être bloqué un verdict de la justice. Le 7 juillet prochain sera rendu suite à la saisine du tribunal judiciaire de Paris. Ce parcours du combattant a poussé le gouvernement à prévoir dans le cadre au projet de loi sécuriser, réguler l'espace numérique de donner à l'art comme la possibilité sans passer par une décision judiciaire de se prononcer sur le blocage et de déréférencement à la et de la mise une mise à l'amende. Des sites ne respectant pas cette obligation. C'est un pas dans la bonne direction qui rejoint d'ailleurs les recommandations mises en avant dans le rapport de la délégation, j'évoque aujourd'hui cet épisode car il doit nous alerter sur la solidité des garde-fous à mettre en oeuvre pour faire passer la protection du bien-être et de la santé de nos enfants avant les intérêts des plateformes privées. Cela suppose aussi d'ailleurs au au-delà de belles intentions de doter une structure comme l'art comme des outils administratifs et des moyens humains nécessaires pour faire vivre

Mes chers collègues par cet amendement. Nous proposons d'inscrire une nouvelle obligation pour les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne. Elle consiste à délivrer une information à l'utilisateur sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention aux mineurs de moins de 15 ans ainsi qu'à leurs parents. L'exposé des motifs de la proposition de loi indiquait je cite que les parents ignorent souvent le contenu et vous l'avez beaucoup dit de la vie numérique de leurs enfants et ne super pas leur activité. Il serait ainsi à peine plus de 50% à décider du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 80% déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants ce que leurs enfants font sur Internet ou les réseaux sociaux. Ces chiffres font prouve donc l'impuissance des parents face à des pratiques que leurs enfants maîtrisent souvent beaucoup mieux que sans en maîtriser les conséquences. Il est donc proposé d'inclure dans le dispositif de la proposition de loi, une obligation d'information des familles lors de l'inscription, information qui pourrait prendre la forme de conseils sur les risques liés à l'utilisation d'Internet et des moyens de les aborder du droit à l'oubli, la protection des données, la surexposition aux écrans ou même de l'indication du numéro Vert dit en France le 30 il est le numéro que vous connaissez pour les enfants victimes de violence numérique et pour leurs parents le décret d'application de l'article 6 7, précisera les caractéristiques et modalités de cette information afin que le même niveau de protection soient offerts par tous les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans et à leurs parents. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure votre avis sur cet amendement. je sa visibilité joue l'accord doit être améliorée, elle devrait d'ailleurs par ailleurs de préciser par le DSA, que nous examinerons prochainement mais je crois que notre assemblée doit privilégier l'intérêt des mineurs par rapport aux simples considérations d'articulation des normes entre elles, donc vous l'aurez compris. C'est donc un avis favorable en espérant que le gouvernement fasse le même choix que notre chambre c'est-à-dire protéger nos mineurs envers et contre. Merci Monsieur le Ministre, votre avis. Merci madame la la la présidente l'argumentation de Madame la rapporteure est parade néanmoins il m'appartient d'être. Défenseur. Si l'on peut dire. De la ligne de crête. Que nous devons emprunter pour ne pas trop empiéter sur le DS pourquoi parce que le DSA est le fruit d'un compromis. Que la France a. Dont la France a obtenu qu'il soit exigeant. Et. Et qui évidemment n'a, n'a pas permis d'intégrer. Dans la version finale du texte l'intégralité des desiderata de la France. Néanmoins, il a atteint un équilibre. Qui qui permet à l'Europe d'imposer sur l'ensemble de son territoire un certain nombre de règles et donc le gouvernement sera toujours très prudent lorsque. Les les propositions. D'amendements parlementaires viendront empiéter sur le champ. Définitif. Du DSA en tout cas telle qu'il, il est apparu à l'issue des des discussions. Ceci étant dit sur sur cet amendement numéro 8 au qui qui a l'article 35 à l'article 14 du. Du DSA. Et à notre avis satisfait je le. Le gouvernement va émettre un avis de de sagesse, la vie sera un tout petit peu plus sévère. S'agissant de l'amendement suivant considérant que dès lors que l'amendement numéro 8 et. Est adopté par l'Assemblée. Alors le l'amendement numéro 9 est satisfait doublement d'une part par le DSA et d'autre part par l'amendement que vous aurez adopté juste préalables et je vous demanderai donc peut-être de retirer l'amendement numéro. Madame la sénatrice, je mets aux voix. Avec. Un avis favorable de la commission. Défavorable du gouvernement qui va sagesse pardon sagesse. C'est pour ça que je vous posais la question. Tu as bien suivi. Désolé. Donc un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement je mets aux voix cet amendement qui vote pour. Contre, abstention il était adopté. L'amendement numéro 9. merci madame la présidente, je sais déjà la position du gouvernement mais je vais la je vais quand même présenté cet amendement qui propose de suivre une recommandation de la CNIL. En effet, la Commission a précisé que le RGPD impose de fournir aux personnes concernées une information sur les conditions d'utilisation de leurs données et sur leur droit qui soit compréhensible aisément aisément accessibles en des termes clairs et simples en particulier pour toute information destinées spécifiquement un enfant pour ceux-là pourtant il suffit de naviguer sur certaines de ces plateformes massivement utilisé par les mineurs, pour se rendent compte que cette information sur les données est loin d'être une pratique généralisée. La CNIL avait néanmoins indiqué que cette je cite obligation d'une information adaptée et pourtant la clé de voûte du dispositif de protection des mineurs. Elle conditionne la possibilité même d'un consentement éclairé ainsi que la connaissance des droits dont ils disposent dont il te pourrait évidemment pas se saisir s'il les ignore où n'en comprennent tout simplement pas le sens et l'intérêt je vous remercie. Merci madame la rapporteure votre avis. Alors cet amendement suit la même logique que le précédent le le numéro 8 et emporte donc une même appréciation de la part de la Commission, c'est donc un avis favorable parce que cela va dans le sens d'une meilleure protection des mineurs. Merci Monsieur le Ministre votre avis s'il vous plaît. Comme précédemment évoqué, c'est une demande de retrait à défaut défavorable puisque. Cet amendement, nous semble doublement satisfait d'une part par le DSA, qui prévoit explicitement que les conditions générales d'utilisation doivent être. Conçus de manière à être facilement compréhensibles par les enfants, et d'autre part parce que vous avez adoptée il y a quelques instants un excellent amendement l'amendement numéro 8. Qui prévoit déjà qu'une information est donnée au moment de l'inscription. Merci. Je je vois cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour. Abstention il était adopté. L'amendement numéro de monsieur Merci madame la présidente. Donc cet amendement a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne d'empêcher les mineurs numérique de consulter des contenus inappropriés. Parce que si certains fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne ont mis en place des outils afin de limiter la consultation telle que tenu par les jeunes grâce notamment au mode restreint poser cette obligation de résultat forcerait les fournisseurs de service à améliorer le fonctionnement de leurs algorithmes qui tendent qui tendent à enfermer l'utilisateur dans une niche. On a notamment pu assister à une augmentation des actes d'automutilation chez des adolescents orienté par l'algorithme vers une bulle dépressive. Je rappelle exhale également. Que le règlement européen sur les services numériques ou le DSA. N'entrera en vigueur que le 17 février 19, 2024 et le 25 août 2023 pour les très grandes plateformes en ligne. Il dispose notamment à son article 42 que ce sont aux États membres de fixer de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services aussi par cet amendement. La sanction applicable aux fournisseurs de services de réseaux sociaux, laissant une libre-consultation mineur de moins de 15 ans à des contenus inappropriés permettrait ainsi d'être fixé à une amende ne pouvant excéder 1% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent du fournisseur de services de réseaux sociaux. Merci madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. Alors cet amendement. Par et on en a déjà parlé d'une réalité incontestable largement développé hein d'ailleurs dans le rapport. C'est-à-dire que les jeunes sont confrontés à des contenus douteux sur les réseaux sociaux. Alors toutefois de problèmes se posent. Premièrement, un problème juridique puisqu'il n'a pas de définition de contenus inappropriés. Comme vous savez si la pédo-pornographie ou le terrorisme ne font pas débat. Hé bien la frontière est souvent beaucoup plus flou finalement sur d'autres sujets en complément. Il est à noter qu'une procédure de signalement des contenus manifestement illégaux existent déjà, alors si bien sûr, nous ne pourrons pas pleinement nous en satisfaire avec le chemin est encore long. Je crois qu'il faut travailler plus en profondeur pour ne pas fragiliser justement une protection qui existent déjà et puis deuxièmement il y a un problème on va dire juridico-pratique puisqu'il n'est pas question de contrôler a priori les contenus postés par les internautes sur les réseaux de fait leur classement en approprié ou non, étant en pratique irréalisable à nouveau. Je répète que le DSA sera examiné prochainement par le Sénat et devrait comporter une palette de mesures en matière de régulation des contenus en tout cas je l'espère. C'est donc, vous l'aurez compris, un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame la présente Mesdames et messieurs sénateurs à satisfaire satisfaire l'intention qui est la vôtre, à la fois sur la question du retrait des contenus, même si. Ce que prévoit le DSA, c'est que chaque plateforme devra disposer d'un processus. De signalement par les usagers mais aussi par des tiers de confiance identifiée identifiée sous le vocable de signer alors de confiance seront des associations notamment étaient des associations de protection de l'enfance des sa prévoit également un régime de sanctions puisque c'est en cas de manquement aux obligations 6% du des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires qui seront prononcées. Merci. Il est retiré. De patient l'amendement numéro 10, madame Robert. Oui merci madame la présidente. Bien. Cet amendement va rentrer dans la même logique que le suivant qui vise à permettre aux mineurs de 15 ans au mieux de mieux exercer leurs droits numériques. Seule une différence de degré distinguera ces deux amendements. Vous verrez car ce tu amendement s'inscrit pleinement, celui-ci dans le dispositif prévu qui octroie aux mineurs de 15 ans, en plus de l'autorité parentale, le droit de demander la suspension de son compte les fondements de cette proposition, sont de 2 ordres principe y a les pratiques comme il a été souligné dans le rapport de l'acné de 2021 sur les droits numériques des mineurs le RGPD invite à vite a favorisé cette autonomisation autant que faire se peut, selon l'âge et le degré de maturité des mineurs à cet égard. Rappelons que l'article 1 du RGPD garantit le droit à l'autodétermination informationnelle. Donc c'est toute personne qui doit être mise en capacité de maîtriser les données qui le concerne 100 cette faculté point d'apprentissage et point d'autonomisation. D'un point de vue plus fonctionnel et parents de sont pas nécessairement au courant des violences que peut subir par exemple leurs enfants dans l'espace numérique. Vous l'avez beaucoup dit, autrement dit en s'assurant que les mineurs de 15 ans puisse directement sollicité la suspension de leur compte, nous les protégeons plus efficacement. Loin d'être antinomique et je ne veux pas que cet amendement le soit avec l'exercice de l'autorité parentale, ce droit accordé complète donc le dispositif pour lui apporter une protection supplémentaire et traduit une des recommandations de la CNIL. Alors vous allez me répondre et je termine là mais aujourd'hui madame la sénatrice, c'est possible. Je vous répondrais oui dans les faits c'est possible mais en droit, j'aimerais bien que vous me précisiez car si un jour un réseau social parce qu'il faudra l'autorité parentale. Hé bien. Dès lors qu'on l'a on l'introduit dans la loi. Pourrait empêcher un un jeune finalement de suspendre son compte. Donc c'est vraiment un amendement qui vise à le protéger encore plus efficacement. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure votre avis. Alors la faculté de suspendre son compte existe sur toutes les plateformes hein je l'ai d'ailleurs vérifié personnellement en tout cas sur les réseaux sociaux les plus importants. Je profite de cet amendement pour vous dire bien sûr que je partage votre préoccupation, vous le savez qu'évidemment je serai très attentive, en tout cas sur les plus texte pour qu'il ne puisse jamais remettre en tout cas cette possibilité en cause en l'état donc l'amendement et donc sur le fond déjà satisfait par la pratique. Donc ce sera un avis défavorable. Monsieur le Ministre. Même avis. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro trois Madame Robert. Oui, donc vous l'avez compris, madame la présidente, chers collègues, finalement c'est un amendement qui. Est un peu similaire à à à l'autre, sauf que il va plus loin en termes de graduation, d'abord je voudrais dire que la protection des mineurs recouvre un triple enjeu, un enjeu de santé publique bien sûr un enjeu éducatif mais aussi un enjeu sécuritaire. Puisque il faut donc établir ce code, pas un appel un ordre public numérique, c'est-à-dire. Finalement que la protection des mineurs et en est une composante essentielle l'édifice juridique est en cours de construction, comme le démontre l'actuel foisonnement des textes législatifs, on a parlé du DMA du DSA des règlements européens, il veut son et discuter bien sûr prochainement à l'occasion du passage. En en séance publique. Ces propositions doivent la proposition la vise visant à réguler l'activité d'influenceurs à garantir le droit à l'image viennent aussi d'être votée par notre assemblée et nous débattrons bien sûr prochainement d'autres projets de loi. je regrette un peu l'éclatement de ces différentes initiatives qui rend difficilement lisible et saisissable ensemble du corpus juridique élaboré. Il n'en demeure pas moins qu'elles permettent d'adapter notre droit aux nouveaux usages numériques et appelle bien sûr de notre part. Vigilance et anticipation cet amendement vise donc à répondre à ces triple enjeu hé bien sûr. En l'état la PPL ne prévoit que la possibilité de suspendre le compte. Ce qui apparaît sur demande de l'autorité parentale. Ce qui apparaît peut être insuffisant afin de conférer au droit à l'oubli, une pleine portée conformément à l'article. La lettre de l'article 51 de la loi Informatique et Liberté. Le mineur de 15 ans doit pouvoir supprimer librement son compte ainsi que toutes les informations afférentes ce droit numérique lui appartient, c'est la philosophie de cet amendement, je vous remercie. Merci madame la rapporteure votre avis. Alors comme pour la suspension évoqué hein à l'amendement précédent la faculté de supprimer son compte existe. Là aussi sur toutes les plateformes et j'ai envie de dire heureusement. En tout cas j'ai pu vérifier là aussi. Dès lors, mon avis reste le même, l'amendement est déjà satisfait par la pratique, donc ce sera un avis défavorable. Monsieur le Ministre même avis. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorable qui est pour. Contre. Abstention il n'est pas adopté. Un amendement et un sous-amendement le l'amendement numéro 4, madame Robert. par cet amendement. Nous proposons que les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne soit légalement tenus de proposer un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services. Lors de l'inscription d'un mineur, la surexposition aux écrans entraîne selon l'association, il en France des problèmes de concentration et de mémorisation, avec une baisse des risques Utah scolaire et bien sûr parfois un repli sur soi. Elle a également des conséquences sur le sommeil car la lumière bleue des écrans, vous savez bloque la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, l'horloge interne et les cycles de sommeil s'en trouve donc parfois perturbé. Cette association relève aussi des troubles du comportement et des conséquences psychologiques et de parfois même des conséquences physiques, la surexposition aux écrans peut entraîner l'addiction aux jeux vidéos, aux jeux de hasard en ligne à un risque accru d'Exposition aux contenus choquants ou inadapté ou encore bien sûr aux mauvaises rencontres en ligne cet amendement tend donc à ce que chaque entreprise de service de réseau social propose un décompte du temps d'utilisation quotidien pour les utilisateurs mineurs qui leur seraient envoyés prendre conscience du temps passé sur un réseau social est un 1er pas pour lutter contre l'addiction à ces plateformes. Je suis heureuse que notre rapporteur et par son sous-amendement rendu plus contraignant. Le dispositif de notre amendement les mineurs doivent effectivement prendre conscience du temps passé sur les réseaux, et une information régulière obligatoires obligatoires pardon et automatique de leur part en constitue la meilleure garantie. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure votre sous-amendement. Cet ajout donc pourrait effectivement constituer une fonctionnalité utile je pense donc cependant qui sera encore plus. Pertinent de Laurent donc obligatoire avec le sous-, amendement numéro 15 que je vous propose. Je vous propose donc ce sous-amendement donc c'était l'amendement quatre hein notamment de David Assouline. Donc c'est un amendement qui prévoit un dispositif optionnel de contrôle du temps passé par les mineurs sur les réseaux sociaux qui vient de s'appliquer par notre collègue Sylvie Robert, je propose donc d'aller plus loin avec ce sous-amendement afin de rendre cette information n'ont pas finalement optionnel et passive avec un utilisateur qui devrait aller chercher dans les paramètres pour consulter son temps passé sur les réseaux, parce que finalement personne le fait mais plus active, c'est-à-dire que l'utilisateur recevrait directement l'information sous forme de notification régulière, je trouve cela en tout cas plus pédagogique car on oublie trop souvent, le temps passé sur les réseaux sociaux et les biens que les mineurs puissent surtout en prendre conscience. Voilà, c'était l'objet de ce sous-amendement que je vous propose d'adopter. Merci Monsieur le Ministre, votre avis sur le sous-amendement et l'amendement. Merci madame la présidente. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le le gouvernement veille à ce que. Le. La loi nationale ne viennent pas. Fait à commettre des entorses. Au Auchan qui a été délimité par le législateur. Européen. S'agissant. Du, du mode de fonctionnement des des réseaux sociaux le le DSA prévoit d'ores et déjà que. Les plateformes où les éditeurs de réseaux sociaux doivent garantir le plus haut niveau de sécurité, de sûreté de protection de la vie privée des mineurs, y compris en mettant en place un certain nombre de paramètres On est là. Clairement dans le dans le Champ du DSA mais comme je l'ai fait tout à l'heure je m'en remettrai à la sagacité du Sénat pour savoir si effectivement l'articulation entre

Sagesse. J'avais bien compris. Merci Monsieur le Ministre. Je mets aux voix le sous-amendement. De la commission avec un avis sagesse du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient. Il est donc adopté je mais aux voix l'amendement numéro 4 ainsi modifiée avec donc un avis de sagesse de la part du gouvernement qui votent pour, contre, abstention-il être adopté. L'amendement numéro 5 Madame Robert. merci madame la présidente par cet amendement. Nous proposons que les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne soit légalement tenus de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu'un contenu est signalé par un mineur ou qu'il concerne un mineur, compte tenu du public extrêmement spécifique constituent les mineurs par nature plus influençables, plus vulnérables que les adultes. Il est important que dans ces 2 cas, une personne humaine et non un algorithme traite du problème. On ne peut ainsi se permettent de traiter ou de régler un signalement de harcèlement dont on connaît les conséquences souvent dramatiques. Par le biais d'un algorithme. Alors j'entends les arguments de notre rapporteur selon lesquelles un traitement mixte associant à la fois traitement algorithmique mais aussi traitement humain avec un 1er tri par algorithme serait plus rapide et donc plus efficace et qu'il serait déjà à l'heure. Je m'interroge dont en plus sur son efficacité. Alors que l'on assiste à une recrudescence d'actes dramatiques allant jusqu'au suicide, parfois vous l'avez entendu de la part de jeunes victimes des pratiques de réseaux sociaux, et principalement bien sûr de harcèlement je maintiens donc Monza mon amendement pour demander que davantage de personnes humaines rentre dans la gestion de notre cybermonde aujourd'hui. Merci madame la rapporteure votre avis. Alors on comprend. Eh bien l'idée des auteurs de l'amendement hein qui insiste sur l'importance d'un traitement spécifique. Des signalements relatifs à un mineur. Mes chers collègues, si nous partageons le fait que des algorithmes ne doivent jamais remplacer en tout cas à l'appréciation des hommes. Votre amendement serait in fine et contre-productif puisque premièrement cela va rallonger considérablement les délais de traitement d'une part, car le nombre de signalements ne cesse d'augmenter et d'autre part, car des esprits mal intentionnés pourraient se servir finalement de cette mesure pour submerger les équipes en charge ces traitements et puis deuxièmement et cet argument Éric beaucoup les, les mesures de ce texte, vous l'aurez compris, il s'agit de mesures européennes, que nous examinerons là aussi bientôt. Le règlement DSA d'application directe prévoit comme vous le savez déjà des procédures de modération spécifique et proportionnée, en fonction des besoins identifiés donc parce que déjà satisfait par le droit européen, ce sera donc un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame présente même avis que que la rapporteure. Effectivement il faut garantir. Que dans le cas des 10 décisions les plus difficiles. Une personne humaine puisse effectivement réagir. Et et prendre cette décision, mais il ne faut pas négliger que parmi les éléments positifs qui viennent avec l'Intelligence artificielle, qui s'est invité. Désormais quotidiennement dans. Dans, dans les médias et en réalité, dans la salle à manger des des Français, hé bien il y a la capacité à à modérée beaucoup plus efficacement les réseaux sociaux, puisqu'il y a des contenus qui sont de toute évidence illicite de toute évidence inappropriée et que l'Intelligence artificielle peut repérer beaucoup plus rapidement et et exclure beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc voilà les raisons pour lesquelles le gouvernement est défavorable à cet amendement. Merci je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour, contre, abstention il n'est pas z'adopté l'amendement numéro 12 me Oui madame la présidente par cet amendement. Donc on on vise à obliger les fournisseurs des services de réseaux sociaux en ligne de diffuser des messages d'information contenant un avertissement général quant au risque d'externalités négatives dont sont à l'origine, les réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des jeunes notamment des mineurs. Si l'article 1er, terre de cette proposition de loi prévoit la mise en place d'avertissement spécifique pour le cyber harcèlement qui se traduirait notamment par la diffusion de messages de sensibilisation et de prévention. Pourquoi ne s'arrêter qu'à sept externalités négatives et ne pas les compléter d'autres. Cette liste pourra d'ailleurs être complétées, notamment après la sortie du rapport prévue à l'article IV. On sait comment ça se passe pour le le tabac hein des avertissements à apposer sur les paquets de cigarettes et autres produits du tabac améliore l'information sur ces dangers, donc nous pouvons ainsi facilement faire un parallèle avec les risques que portent les réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des jeunes et améliorer la visibilité et l'accès quotidien au risque d'externalités négatives de ces réseaux doit nous préoccuper et des solutions doivent être trouvées. Merci madame la rapporteure votre avis. Le présent amendement semble déjà partiellement satisfait avec les amendements numéro 8 et 9 qui renforce donc les obligations d'information des des mineurs au moment de l'inscription sur les risques des réseaux sociaux et sur l'usage des données personnelles son Champ et par ailleurs plus large puisqu'il ne concerne pas exclusivement les mineurs mais l'ensemble des inscrits. Par ailleurs, il ne dit rien finalement sur le moment où ces messages devront être diffusé. Vous l'aurez compris, en tout cas ce n'est pas l'objectif de l'eau de, de l'amendement qui me pose problème mais plutôt sa faisabilité. Donc pour rester dans le Champ du texte. Je propose un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame la la présidente, simplement pour dire que, effectivement, est très important que l'import l'information parvienne. Jusqu'aux utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier les mineurs et leurs parents. Que c'est la raison pour laquelle nous avons. Généralisé où nous allons généraliser dès la rentrée prochaine. Le passeport numérique en sixième de manière à ce que tous les élèves de 6ème puissent bénéficier d'un Module. De prévention aux risques et et d'éducation aux gestes à adopter en ligne et par ailleurs. Le le le gouvernement soutient et encourage l'action d'un certain nombre de réseaux associatifs très engagé dans la prévention, à la fois à destination des. Des enfants et des parents, je pense à l'action de l'UNAF. Des associations Tralalère. Open de génération numérique ou de il en France qui a été cité à plusieurs reprises à la tribune tout à l'heure. Mais pour les mêmes raisons que Madame la rapporteure sera un avis défavorable. Merci je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Abstention il n'est pas adopté. L'amendement numéro 16 de madame la rapporteure. je vous propose avec cet amendement, de répondre aux préoccupations exprimées par nos collègues Sylvie Robert et Catherine Morin-Desailly sur les encyclopédies en ligne à but non lucratif et les répertoires éducatif et scientifique à but non lucratif, je pense notamment à Wikipédia, il serait en effet très regrettable évidemment de restreindre leur fréquentation alors qu'ils constituent des des sources d'informations très utiles. Il est donc proposé avec cet amendement, de les exclure explicitement du Champ de la proposition de loi. Alors je travaille à cette rédaction afin de la rendent plus compatible avec le droit européen on ne touchons pas à la définition des réseaux sociaux qui est l'objet de l'article 1er qui est issu de DSA. Je vous propose donc d'adopter cet amendement qui règle une question importante. Et je remercie bien sûr. Mes collègues d'abord soulevé cette problématique. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Et effectivement, merci à, à Sylvie Robert Catherine Morin-Desailly est à madame la rapporteure. Pour ce travail collaboratif qui conduit à une précision très utile pour le texte, un avis favorable. Merci je mets donc on voit cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui vote pour. Contre. Abstention il être adopté je mets aux voix l'article de ainsi modifié qui est pour. Contre, abstention et être adopté l'amendement numéro 14. Madame Billon. et qui prévoit de bloquer systématiquement le téléchargement par les boutiques d'applications logicielles telles qu'elles sont définies au sens du règlement de 2022 1925 donc. Il vise à rajouter une protection supplémentaire en obligeant ses boutiques d'applications logicielles à bloquer systématiquement le téléchargement des applications au service. Des réseaux sociaux réservés aux personnes majeures et mineures en effet ces boutiques d'applications logicielles connaissent l'identité et l'âge de leurs utilisateurs puisque ce sont des informations demandées dans le cadre de la création d'un compte pour télécharger 16 application. L'objectif n'est pas de remettre évidemment en question les obligations imposées aux fournisseurs de réseaux sociaux mais de les compléter avec une mesure qui interviendrait en en amont pour un type d'application bien précis en l'occurrence les applications conçues pour un usage pour des personnes de 18 ans et plus. Donc les téléphones connectés sont le principal moyen pour les mineurs de télécharger des applications, réseaux sociaux et et donc c'est un moyen supplémentaire qui permettrait ce contrôle, je vous remercie. Si madame la rapporteure votre avis. Qui est la place donc des magasins d'applications, je vais pas les citer, vous les connaissez tous. Et puis la responsabilité des systèmes d'exploitation, alors c'est un amendement qui est sans doute celui sur lequel je me le suis plus interrogé. Lors des auditions cet enjeu nous a été soulevé. L'idée est apparu plutôt intéressante. Si la vérification de l'âge par les plateformes pose déjà de nombreux problèmes l'adoption en tout cas de cet amendement qui vise donc à faire peser ce contrôle également sur les boutiques d'applications entraînerait finalement des difficultés supplémentaires qui viendraient complexifier une procédure déjà lourde à mettre en oeuvre mais qui repose exclusivement donc sur les plateformes. Par exemple, on pourrait se poser la question de savoir si ce qu'au partage de responsabilités finalement n'ouvrirait pas la voie son délaissement par les 2 parties qui seront verrez un peu la balle à chaque fois. De plus, l'adoption de cet amendement ne semble pas compatible avec le dispositif porté par l'article 2 de cette proposition de loi qui prévoit, je le rappelle, le recueil d'une autorisation parentale pour une inscription sur un réseau quand le mineur à moins de 15 ans. Toutefois et ce malgré ses arguments. Je souhaite tout de même. Comme on demandait l'avis du gouvernement, car je pense sincèrement que. La question de l'implication un des systèmes d'exploitation doit vraiment et travailler en concertation avec toutes les parties. D'ici l'examen du projet de loi sur l'espace numérique.

à une question importante. Madame la rapporteure la la rappeler qu'il a la responsabilité des magasins d'applications dans la vérification d'âge. C'est peut être effectivement. L'une des solutions à ce problème qui concerne le sujet qui nous rassemble aujourd'hui la majorité numérique, c'est-à-dire la vérification d'âge à l'entrée sur les réseaux sociaux mais aussi. Le problème de la vérification d'âge pour les contenus qui sont réservés aux adultes, c'est-à-dire la barrière si l'on peut dire des 18 ans. je vous remercie madame les sénatrices. D'avoir consacré du temps à la rédaction de cet amendement. Cet amendement pourrait encore être. Améliorée. Et qu'il. Aurait. Toute sa place dans le débat qui va entourer l'examen. Du projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique pour 2 raisons, la première c'est que, comme je le disais à l'instant. La proposition de loi qui nous rassemble aujourd'hui traite de la question de l'accès aux réseaux sociaux au dessus ou en dessous de l'âge de 15 ans, notamment avec la question qui se pose du recueil du consentement parental. L'objet qui est visé par votre amendement. Et qui en quelque sorte évoque la question. des contenus réservés aux adultes comme celui qui a été traitée dans le rapport que vous avez commis avec madame la rapporteure, c'est celui des applications de rencontre qui sont réservés aux adultes et qui exclut tous les mineurs de 18 ans, c'est ce qui est une question légèrement différente de celle de l'accès aux réseaux sociaux auxquels certains mineurs peuvent avoir droit. Le projet de loi qui vise à réguler et sécuriser les l'espace numérique traite. De ces questions en en allant chercher les les les les propositions du rapport sénatorial c'est la raison pour laquelle ce débat de la vérification d'âge au niveau des magasins d'applications pour l'accès à des services réservés aux adultes aurait sa place dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. D'autre part la la rapporteure a fait état de quelques améliorations techniques qui pourraient être apportées au dispositif que vous proposez et que je m'engage à travailler avec vous si vous le si vous y conforter madame la sénatrice, ainsi qu'avec Catherine Morin-, Desailly. D'ici là puisque nous avons encore quelques semaines. Pour le faire. Je vous propose donc de retirer l'amendement en contrepartie des engagements que je viens de de prendre. Et et vous remercie une nouvelle fois pour pour cette proposition. Merci madame la présidente. Merci madame la rapporteure et Monsieur le Ministre, pour les explications. On le sait. Tout mettre en oeuvre pour éviter que les mineurs, mineurs pardon et des contenus auxquels ils n'ont pas le droit d'accéder, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que je, je regarde la rapporteure lorsqu'on a rendu nos conclusions porno l'enfer du décor. On a fait plus d'une vingtaine de propositions. On voyait bien qu'elle nécessitait encore du travail pour pouvoir être abouti. C'est pour ça que nous avions été vous voir Monsieur le Ministre, c'est pour ça que nous avions été aussi voulait présenter Madame la Ministre parce que nous souhaitons, ce travail de construction. Donc oui c'est difficile de trouver les bons dispositifs réussir à bloquer les sites pour réussir à bloquer l'accès des mineurs et bien entendu Monsieur le Ministre, avec ma collègue Catherine Morin-Desailly nous serons tout à fait disposé d'ici début juillet à travailler à améliorer cet amendement parce que c'est un dispositif qui est proposé, qui peut permettre de compléter tous les dispositifs qu'on essaye de mettre en place mais ce ne sera pas suffisant, on le sait, donc comme je disais dans la discussion générale, tout doit être tenté. Tout doit être expérimenté. Tout doit être essayer pour qu'on avance sur ce suis sujet d'évidemment de contrôle de l'accès. À ces contenus normalement interdit aux mineurs notamment merci donc, bien entendu je parle pour Catherine Morin-, Desailly qui n'est pas là mais je, j'imagine qu'elle s'associer Sierra à mes propos.

Madame la présidente. Donc il y a pas de problème, il est donc retiré jamais aux voix l'article 3 qui n'pas zut d'amendements qui est pour. Qui est contre il était adopté des amendements à l'article 4 le l'amendement numéro 6, madame Robert. Oui merci madame la présidente. Il s'agit simplement par cet amendement de compléter la demande de rapport on a hâbleur dans un angle mort de la proposition de loi, mais on en a beaucoup parlé ce soir c'est l'accompagnement des parents. Quant aux usages des plateformes en ligne par les mineurs. Merci madame la rapporteure. Il a été élaboré dans le cadre d'un partenariat national qui vise à fédérer les acteurs publics et privés cette cette plateforme propose je le rappelle déjà des outils et des conseils et des ressources Patrick pour mieux informer et accompagner les parents afin qu'ils protègent leurs enfants ils ne paraît donc pas utile, à mon sens de surcharger encore un peu un rapport qui a déjà été largement complété lors du passage du texte à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison, donc que je donnerai un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre, Madame la Ministre pardon. Simplement pour rappeler que le gouvernement est engagé dans une politique complète stratégique à destination des familles avec plus que un simple rapport puisqu'on est, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs dans une logique de diffusion de d'ateliers parentalité dans des d'illogique de diffusion de documents donc c'est au-delà du rapport, le gouvernement rendra compte régulièrement de sa stratégie à l'égard des familles. Nous ne pouvons pas régler les problématiques de nos enfants sur Internet sans les parents, c'est une conviction que nous avons avec le ministre. Nous sommes très régulièrement en contact avec les associations et avec les parents eux-mêmes sur le, sur Merci je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre. Abstention il n'est pas adopté, je mais aux voix l'article IV qui est pour,

Je reviens sur le le la proposition de numéro unique hein qui vise à ce que les victimes de harcèlement scolaire et de harcèlement en ligne n'est plus qu'à composer qu'un seul numéro pour avoir accès à l'ensemble des plateformes d'aide et d'écoute. Je rappelle qu'actuellement, les victimes de harcèlement peuvent appeler soit le 30 20 en cas de harcèlement scolaire soit le 30 18 en cas de cyber harcèlement. Alors que le cyberharcèlement et bien souvent liés au harcèlement scolaire. La réunion de ces plateformes apparaît comme adapté cohérente et source de simplicité donc de rapidité et d'efficacité dans la prise en charge des victimes. Si la demande de rapport visant à demander au gouvernement la remise au Parlement d'un rapport sur l'opportunité d'un rapprochement entre les plateformes téléphoniques d'aide en ligne compte le harcèlement scolaire et de cyberharcèlement a été supprimé en commission ce numéro unique donnerait accès à un standard téléphonique automatisé qui orientera la victime vers l'entité co-compétente soit l'association Enfance en cas de cyber harcèlement soit l'école des parents et des éducateurs d'Île-de-France en cas de harcèlement scolaire. Le flux d'appels importants ne saurait être un obstacle à cette fusion, car je le rappelle. Il ne s'agit pas ici de limiter les effectifs des plateformes d'aide et d'écoute aux victime de harcèlement scolaire et de harcèlement en ligne, mais seulement de simplifier et faciliter leur accessibilité par le recours à un seul et unique numéro, je crois qu'on croule sous les les les les numéros. D'appel je pense que plus on simplifierait surtout pour des gens en détresse. L'accès à ses plateformes serait le bienvenu. Merci. Cher collègue, Madame la rapporteure votre avis s'il vous plaît. Alors notre collègue propose donc un numéro unique. Hein qui orienterait vers l'un des deux services. Alors je rappelle que ça t'article 5 initialement demandé la remise d'un rapport pour rapprocher donc c'est de services, à savoir le 30 20 sur le harcèlement scolaire, et le 30 18 sur le cyber harcèlement alors pour mes noirs. Je voudrais quand même le rappeler pour rappeler la distinction entre ces 2 services il y a le 30 18 qui est opéré par l'association et enfance avec le soutien d'ailleurs du ministère de l'Éducation nationale, il apporte une aide aux personnes victimes de violences numérique. Donc par exemple du cyber harcèlement des expositions à des contenus violents usurpation d'identité ou encore violences à caractère sexiste et puis il y a eu 30 c'est un numéro d'appel gratuit opérée par l'école des parents et des éducateurs d'Île-de-France subventionner là aussi par le ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci fait appel à donc aux professionnels témoins ou victimes d'une situation de harcèlement entre élèves. En tout cas les auditions que j'ai pu mener mon conduit à penser que les 2 services ne concerne pas tout à fait les mêmes publics ni les mêmes problématiques mais elles apparaissent en tout cas elles De de de notamment de Revenge porn sont pas finalement confronté quand même au même problème car harcèlement scolaire c'est pas tout à fait le même sujet. Il me semble donc que l'idée sous-jacente de rapprocher les 2 services devraient être soigneusement pesés, ce qui relève au demeurant et comme je l'indiquais en commission plus du gouvernement, en tout cas que du législateur donc je donnerai un avis défavorable. Merci madame la ministre. J'ai moi même un ami défavorable, ça fait longtemps que je suis interpellé sur le fait qu'il y a en fait trois numéro le 119 le 30 18 et le 30 20 c'est une étude que j'ai moi même conduite en réalité on n'est pas du tout sur les mêmes publics on n'est pas du tout sur les mêmes réponses et on n'est pas sur les mêmes écoutant le 30 20 et en réalité énormément mobilisées par les familles et par les familles, dans les écoles primaires pour du harcèlement. Le harcèlement physique et des problématiques qui sont réels au sein, au sein des écoles. Je rappelle que dans le 30 20. D'ailleurs les écoutants, qui sont issus de l'éducation nationale qui sont pilotés par l'éducation nationale ont l'obligation d'ailleurs de prendre attache avec l'école C'est ce qui fait un obstacle majeur pour des adolescents notamment qui voudraient saisir pour du Revenge porn ou pour des problématiques de contenus qui porte atteinte à leur intimité, le 30 20, même si son cyber. Sur ça parce que il y a la question de la confidentialité et de la confidentialité, tant à l'égard parents qu'à l'égard de de l'école donc fusionner le 30 20 et 30 18 sait fusionner des des démarches des publics et des problématiques différentes et des acteurs différents. Il y a une vraie formation une vraie compétence dans le train voilà dernière élément extrêmement aussi important pour moi, le 30 18 est considéré comme un signal heures de confiance au niveau européen, c'est ce qui lui permet de signer des conventions avec l'ensemble des plateformes et d'obtenir des retraits de contenus extrêmement rapide, ce qui n'est évidemment pas le rôle de l'éducation nationale qui a fort à faire déjà avec nos enfants, donc on a vraiment 2 démarches différentes, je souhaite vous rassurer le 119 le 30 18 et le 30 20 ont ont des mécanismes de relais quand il y a une erreur de d'embranchements pardonnez-moi et ont des mécanismes de relais aussi compte le le le la problématique est à cheval sur 2. Sur de situations, il était évident que par exemple 30 18, invite l'enfant à prendre attache avec ses parents ou ou ou peu signaler des Arctic 40 notamment au niveau de la justice, il faut que l'école et les parents se mobilisent donc les mécanismes on les on les travaille, on ne peut pas enfin aujourd'hui en tout cas on ne peut pas fusionner ses numéros il y a vraiment des démarches différentes entre l'enfance en danger l'ado qui a besoin d'aller signaler quelque chose sur le 30 18 et les familles qui constate un harcèlement notamment pour les plus jeunes. Donc je suis défavorable à cet amendement. Monsieur le sénateur pour explication de vote. Oui et je ne sais pas si je me fait mal comprendre parce que moi je ne souhaite pas du tout que les services soient fusionnées les réponses sont bien sûr spécifique, ce que je dis simplement, c'est qu'on doit quand même être capable aujourd'hui d'avoir un numéro unique qui soit très simple pour pour que tout ce qui touche autour du harcèlement scolaire du cyber harcèlement et cetera soit unique et ensuite c'est la plateforme qui dispatche rail qui enverra vers une réponse qui soit différente. on va plus avoir, il va nous faudra effectivement un smartphone supplémentaires pour pouvoir noter tous les numéros d'appel qu'on aura à faire en cas d'urgence ou c'est simplement est-ce qu'on peut simplifier les choses sais ce que je demandais. Et j'insiste pour qu'on puisse essayer quand même de concevoir un numéro unique qui sera capable quand même après d'orienter vers des réponses et des services différents. Merci, chers collègues, je mais aux voit cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient. Il n'est pas z'adopté je mais je vois l'article 6 qui votent pour, contre, abstention il être adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, il y a-t-il de demandes d'explications de vote.

favorable à une proposition de loi pour protéger nos enfants, pour protéger nos enfants, en particulier de ce monde numérique qui nous échappe et qui échappe aux adultes. Je souhaite que ce soit évidemment applicable l'amendement que j'avais fait voter dans la loi du 30 juillet 2020. Donc il y a plus de 3 ans, cette loi n'est toujours pas appliquée. Probablement que c'était difficile, mais c'était une loi pour protéger nos enfants de contenus qui sont destinés à des adultes. Tout le monde est d'accord pour les protéger. À partir de quel moyen, c'est là où on se demande comment on va faire, donner des moyens supplémentaires à l'art comme on se passe en 2 juges, pourquoi pas, mais je voudrais vraiment insister sur un point, on peut. Effectivement mettre en place des outils faire le contrôle parental mais s'il vous plaît, ne pas oublier de garder la responsabilité au site. Il ne faut pas exonérer les sites qui diffusent ce genre de. De leur responsabilité, c'est destiné à des adultes, pas à des enfants, ça doit donc être interdit aux enfants et on doit contrôler l'âge des usagers. Merci, chers collègues, je mets donc aux voix. Cette proposition de loi. Qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient. Elle était adoptée. Madame la rapporteur. Vous avez demandé la parole. Oui j'ai demandé la parole, tout simplement pour adresser des remerciements. D'abord à vous tous chers collègues ici présents. Merci pour votre mobilisation et pour votre confiance dans le vote de cette proposition de loi, je voudrais adresser plus particulièrement remerciements au président de la commission Culture Laurent Lafon à mon ami Max Brisson et aussi à mon administrateur. Bertrand Pelé. Merci à vous Monsieur le Ministre Madame la Ministre pour la qualité de nos échanges sur ce sujet transpartisan avec comme seul objectif évidemment la protection des enfants qu'on vient de le rappeler ma collègue Marie Mercier et puis des remerciements également pour la séance. Merci infiniment, parce que vous aussi vous avez vous trois, merci à tous, c'était ma, ma première fois au banc. Je suis ravi. Merci madame la rapporteure. Félicitations. Pour ce. Rapport. C'est pas fini en fait. J'ai quelques communications désolé. Oui. Par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande l'inscription à l'Ordre du jour du jeudi 8 juin le matin en 1er Point de l'ordre du jour des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Acte est donné de cette demande. Le délai limite pour les inscriptions de parole sera serait fixée au mercredi 7 juin à 15h, sauf si vous avez des observations. Il n'y en a pas, il en est ainsi décidé par ailleurs à la demande de plusieurs groupes nous pourrions fixer à 1h30 le temps réservé au groupe dans la discussion générale commune sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice. 2023 2027. Et le projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps du site judiciaires pardon, prévue le 6 juin, ainsi que dans la discussion générale sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense prévu le 27 juin prochain, y a-t-il des oppositions. Je n'en vois pas. Il en est donc ainsi décidé mes chers collègues, je vais enfin levé la séance prochaine séance mercredi 24 mai 2023 à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. Bonne soirée, bonne appétit. La séance est levée.